La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point. Le procès verbal est donc adopté sur les réserves d'usage. Notre ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Je vais immédiatement donner la parole. Au président Combo. Je suis saisi d'une demande de la commission tendant réserver l'examen de l'article 2, qui inclut les amendements déposés sur le rapport annexé afin qu'il soit examiné à la fin du texte, vous avez tout dit, monsieur le président. Selon l'article 44 alinéa 6 de notre règlement. C'est bien cela. Vous le confirmez, monsieur le président. La commission des affaires étrangères et de la Défense et des forces armées souhaite effectivement que l'article que l'examen de l'article 2, qui inclut les amendements rapport annexé puisse être examiné à la fin de notre texte. La de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond sauf opposition du gouvernement. Je vois que le gouvernement étant déjà dans une forme de sagesse. Et je je m'en réjouis. La réserve et donc ordonné. Et maintenant, nous allons aborder la discussion générale et je vais donner la parole en

Le président du Sénat. Monsieur le président de la commission des Affaires étrangères et des forces armées et rapporteur de la loi de programmation militaire mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis mesdames et messieurs les sénateurs salue également Madame la Ministre j'ai l'honneur de vous présenter cet après-midi. Un projet de loi de programmation militaire pour la période 2024 2030. Le quinzième depuis le début de la Ve République et depuis que ces lois de programme en matière de défense nationale, spécificité bien française existe. Ce texte de loi pour lequel nous armer les directions et services du ministère travaille depuis un an a été préparé sous l'autorité du président de la République, chef des armées en lien étroit et très en amont avec le Parlement, les acteurs du monde de la Défense, il cherche à traduire une conviction simple, la seule qui vaille les menaces qui pèsent sur la nation française n'ont jamais été aussi diverse et protéiforme que depuis la fin de la guerre froide. À bien des égards et nous place face à un défi aussi important que celui qu'ont dû relever les gouvernements de la fin de la IVe République et plus encore les gaullistes dans les années 60 cette programmation. Acte en effet du retour d'une compétition plus dure entre les grandes puissances sur fond de prolifération nucléaire de la permanence d'un risque terroriste qui n'a pas disparu, et dont malheureusement on ne parle plus assez. Ce qui me donne l'occasion de remercier le Sénat pour le débat que nous avons eu il y a quelques jours sur l'Afrique mais aussi de l'émergence de nouveaux espaces de conflictualité qui découle ou qui sont le reflet de sauts technologiques rapides et brutaux comme en témoigne la militarisation du cyber de l'espace ou des fonds marins. Ces menaces entendent autant dans leur approche classique mais aussi et surtout pour une puissance nucléaire comme la nôtre dans une hybridité qui nous invite à penser nécessairement différemment. C'est là où la dimension de transformation de cette LPM. Ce qui ne signifie pas rupture intervient plus que jamais. Ces menaces nouvelles ou anciennes se cumule désormais plus qu'elle ne se succèdent. Cette programmation militaire a été construite en les regardant et en les analysant froidement en y intégrant les spécificités françaises avec nos forces mais aussi faut le reconnaître nos vulnérabilités. Elle n'a pas pour but de tirer les conclusions comme certains commentateurs ou se experts nous y ont souvent incité de conflits qui ne sont pas les nôtres et qui structurellement ne pourront jamais être les nôtres. La France a un modèle de défense singulier qui lui est propre. Fruit d'une construction historique gaullienne, reposant sur une autonomie stratégique française qui va bien au-delà de la seule dissuasion nucléaire et puis sa force dans le sentiment profond que notre pays n'aurait jamais dû perdre. La drôle de guerre du 19.140 n'aurait jamais dû connaître les difficultés de l'expédition de Suez n'aurait jamais à connaître de nouveaux les guerres d'Indochine et d'Algérie. Cette loi de programmation militaire doit permettre non seulement de poursuivre une réparation d'un outil de défense et là, s'abîmer dans le passé par des politiques parfois court-termiste et une forme de déni, il faut le reconnaître sur la réalité du monde mais aussi de transformer nos forces sur des fonctions militaires concrètes avec des objectifs opérationnels précis. Cette programmation militaire ne propose pas une rupture fondamentale avec notre modèle historique. Au contraire, elle propose à sa manière d'y revenir, dans sa force conceptuelle initiale, c'est-à-dire dans sa capacité à s'adapter vite en prenant en compte les défis du monde actuel et donc les menaces sécuritaires actuels ainsi qu'aux sauts technologiques qui emmène avec eux inévitablement des Sceaux stratégique ou tactique dans le Champ dont le Champ de l'hybridité. À cela. S'ajoute la nécessité d'articuler ces nouveaux domaines de lutte autour notre dissuasion nucléaire et nos capacités expéditionnaires. Permettez-moi de former le voeu. Qu'on ne perdent jamais de vue notre modèle global de défense dans cette discussion parlementaire par de nombreux détails techniques sémantique ou budgétaire qui peuvent toujours évidemment à avoir leur intérêt mais qui ne doivent pas nous écarter de l'essentiel, c'est-à-dire l'exigence de cohérence et l'efficacité opérationnelle. Autre modèle d'armée qui reste et doit rester une armée d'emploi. C'est là l'enjeu c'est là l'héritage que nous avons reçu de nos anciens et que nous devons protéger et laisser aux générations futures ce que nous avons souhaité faire primer dans cette loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, c'est notamment un impératif de cohérence sur lequel je suis revenue longuement ici dans nos travaux en commission comme à l'Assemblée nationale entre les livraisons capacitaire les stocks de munitions de pièces détachées le renforcement des soutiens le maintien en condition opérationnelle et la formation qui accompagne nos soldats sur le terrain. Certains ont parfois le goût de la masse de cibles capacité généreuse, la tentation d'acheter en grand nombre des équipements sans y intégrer leur vie opérationnelle est un piège dans lequel beaucoup de pays voisins et là, sont tombés et encore récemment. Nous avons parfois privilégiés dans le passé pour des raisons d'affichage ou industriels à nombre d'hélicoptères livrés aux armées, alors qu'il aurait été préférable pour elle de fixer le nombre d'hélicoptères en capacité réelle de voler. Nous devons apprendre de nos erreurs passées collectivement, même si je note chez les uns ou les autres, parfois une forme de facilité ou en tout cas un refus d'obstacle intellectuel à considérer cette question dans son ensemble. Une loi de programme n'est pas qu'un tableau capacitaire. Tout cela forme un tout logique efficace qui s'appuie d'abord d'ailleurs sur le tableau des contrats opérationnels. La vraie transformation est à chercher dans ces contrats aux missions détaillé dans le rapport annexé, c'est notre capacité demain à concevoir et à déroulé des opérations, terre air mer cyber espace informationnel cohésion nationale de manière combinée merci aux parlementaires qui ont pris le temps d'intégrer cette dimension nouvelle de transformation notamment Monsieur le président Cambon via l'exercice particulièrement visible d'Orion qui à bien des égards faisait oeuvre de pédagogie en la matière. C'est cela, je le crois, la véritable sont de la guerre en Ukraine à tirer pour nous même si nous devons donner de la visibilité notre BITD si nous devons la protéger la promouvoir, nous y reviendrons la LPM doit demeurer le moment où le Parlement doit se pencher sur l'effectivité opérationnelle ce qui a trop souvent et là c'était négliger dans le passé et a pu placer nos forces en situation de vulnérabilité face aux menaces car précisément, je sais que ce, ce constat est partagé. Nous ne tenons pas ces menaces, pour illusoire. Ces choix pour notre modèle de défense nationale répondent à la volonté du président de la République exprimé lors de sa première élection en 2017 mais aussi aux besoins exprimés par nos armées depuis lors. Après un long travail d'introspection demander aux états majors et à la délégation générale pour l'armement. Cet exercice assez inédit n'a pas été sans difficulté. Je tiens à remercier les chefs d'État-Major le CEMA le DG se parce que as général pour l'administration et le DGA pour s'être livré à cet exercice toujours délicat. Ils ont abouti au projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter et sur lequel vous aurez à vous prononcer en responsabilité. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Le Parlement a un rôle majeur dans les choix stratégiques qui assureront notre défense nationale au cours des 7 prochaines années. Ce rôle a d'ailleurs été largement renforcé par l'Assemblée nationale en lien étroit et en amont avec votre président rapporteur ainsi que par des amendements adoptés dans votre commission ici même de la Défense. Ces dispositions relativement inédite. Il faut le reconnaître dans notre histoire, sous la Ve République et viendront renforcer le contrôle du Parlement sur l'exécution et l'actualisation de cette programmation notamment chaque année en amont l'examen des projets de loi de finances qui reste, on le sait les véritables actes parlementaire pour engager concrètement les moyens dans le respect des grands principes de la Vème République, il est évident que le moment dans lequel nous nous trouvons doit être celui du Parlement. Depuis que je suis ministre des armées. Ah non à votre contact lors des nombreuses auditions que j'ai pu faire ma conviction sur l'importance du rôle des deux chambres n'a cessé de croître. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur les enrichissements, de la copie que vous avez décidé d'intégrer en commission. Je pense notamment aux nouvelles dispositions introduites pour densifier le bilan annuel sur l'exécution de la loi de programmation militaire, que cela soit sur l'inflation sur les stocks de munitions sur les commandes capacitaire sur la réalisation des objectifs de préparation opérationnelle ou sur les moyens pour parvenir à nos objectifs en matière d'accroissement des réserves. Je pense aussi aux nouvelles dispositions qui permettront à la délégation parlementaire au renseignement. Monsieur le Président de mieux contrôler les politiques publiques de renseignement et c'est tout à l'honneur du Sénat que de montrer que la France est une grande démocratie, à ma manière et lors d'une récente audition. À la DPR d'accorder plus de visibilité et en confiance dans le respect du secret défense aux politique je cite mais aussi au sujet, je cite, de renseignement et cela va dans le bon sens. Par ailleurs, comme messieurs en commission devant le président mais devant les différents rapporteurs des différents programmes nous ferons preuve d'une plus grande transparence envers le parlement en communiquant aux présidents de commission en charge de la défense des deux chambres la disponibilité technique des matériels et cela dès le prochain exercice budgétaire. Je viens de l'écrire aux 2 présidents. Il s'agit là d'une avancée majeure. Je le crois et je me savais attendu sur le sujet. La communication de ces chiffres permettra de mieux suivre les efforts consentis par la nation et illustreront bien l'équation subtile à trouver entre cohérence et masse. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Les débats que nous nous apprêtons à à voir dans cet hémicycle seront sans doute moins un moment de vérité politique au sens noble du terme qu'à l'Assemblée nationale où au fond on a insisté un véritable choc modèle contre modèle en quelque sorte où chaque sensibilité a pu tenter décliner les choix qu'elle propose pour nos armées en fonction de leur analyse porté sur la situation du monde et ce débat a eu lieu, vous le savez notamment et pour la première fois avec des sensibilités politiques politiques qui ne sont pas représentés ici au Sénat, il n'est pas besoin de les citer. Ce débat est sain, il n'a rien de médiocre, le vote d'adoption par scrutin public de l'Assemblée nationale a été clair, mais il n'occulte pas des visions du monde et donc de notre défense qui sont irrémédiablement. Je le crois divergentes et peut être même irréconciliables entre elles. Néanmoins ce débat avec ses 2500 amendements et ses 90 heures d'examens ont participé à la force du modèle français car il a permis une nouvelle fois au plus grand nombre de se l'approprier et il serait faux de soutenir qu'il a toujours eu dans notre histoire, un consensus sur tout cela n'a d'ailleurs jamais été le cas depuis 1960 et je m'engage naturellement à la même disponibilité à la même ouverture d'esprit pour ce débat au Sénat qui permettront d'enrichir encore le projet de loi. Dans cet exercice. L'examen du texte dans cette navette au Parlement depuis plusieurs mois maintenant essentiellement à l'Assemblée nationale. Ma. Pour l'instant m'a permis de tirer quelques premiers constats que je me permettrai de partager ici tant il me semble important pour notre défense nationale mais aussi pour le débat démocratique. Certaines sensibilités politiques non présentes ici me semble tout d'abord avancé dans une forme de fou. Je ne veux pas dire masqué, mais en tout cas, ils n'ont pas, jusqu'alors formaliser clairement leur modèle d'alliance leur position sur la dissuasion nucléaire et donc in fine et sur le modèle qu'il souhaite pour nos armées, les deux semaines de débats à l'Assemblée Nationale nous ont permis parfois, mais pas toujours de mieux comprendre ce en quoi il s'opposer au modèle français actuel sans pour autant jamais établir une contre-proposition crédible militairement et encore moins budgétairement. D'autres, quant à eux demeurent fidèles à leur position historique depuis la première loi de programmation militaire en 1960 en clarté en cohérence qu'il faut reconnaître au Parti communiste français il n'en demeure pas moins que le modèle d'armée proposé nous exposeraient immédiatement à des risques imminents. Si je ne les partage pas. Je tiens néanmoins publiquement a salué les explications en séance du député Fabien Roussel au nom des communistes sur la dissuasion nucléaire. D'autres encore ne voudrais regarder ces débats que sous l'angle budgétaire sont toujours en définir leur finalité militaire bien qu'il était directement ou indirectement parfois j'ai 10 réduit les Budgets de nos armées quand il était aux responsabilités, je n'y reviendrai pas mais tenons pour l'avenir. Cette approche comme un avertissement. Nos dépenses militaires doivent rester soutenables pour nos finances publiques et être connecté à nos besoins militaires d'abord et industriels ensuite et dans cet ordre, c'est la la condition de la performance opérationnelle dans la durée. D'autres enfin estiment que nous dépensons trop, sans pour autant expliquer comment répondre aux menaces à moins qu'il ne croit pas en leur réalité. Ce qui me semble, ma foi dangereux et naïf. Quoi qu'il en soit, je respecte et respecterait toujours la position de chacun et je m'efforcerai d'défendent cette loi de programme et les convictions qu'elle porte. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Si des sujets crée le débat. Je me réjouis que les discussions à l'Assemblée nationale et dans votre haute assemblée dessine des consensus ferme d'abord sur quelques points précis qu'il faut, je le crois mentionné. C'est notamment le cas pour renforcer le lien entre la nation ses armées leur histoire que nous réaffirmerons Madame la Ministre dans l'article 11 en pérennisant l'activité dans l'ordre national de libération. Citons aussi des efforts que nous proposons également pour l'accompagnement de nos soldats et de leurs familles à travers l'augmentation des moyens dédiés au plan famille de qui entraîne une forme de consensus, tout comme les objectifs de politique salariale qui renforce la progression par les grilles indiciaires notamment pour les militaires du rang et les premiers grades des sous-officiers dès cette fin d'année 2023. Enfin l'importance de l'inscription des conséquences liées au réchauffement climatique dans l'émission que nous confions nos armées est partagé par tous. La programmation militaire acteur a donc notre modèle d'armée devra intégré dans ses missions, les effets du changement climatique, tout comme l'effort de sobriété énergétique dans lequel nous devons collectivement nous engager nous y reviendrons mais cet aspect n'a rien de neutre et notamment pour nos différents territoires d'outre-mer dont je salue les sénateurs ici présent. Il me semble que la convergence, à la lecture des travaux menés par la commission et je remercie une nouvelle fois le président Cambon pour leur qualité va bien au-delà des points que je viens de lister et nous pouvons collectivement tracer un constat. Dans la majorité des groupes politiques ici représentés. Personne ne remet ne remet en cause le modèle d'armée. Dans cette programmation est dans la continuité historique avec un grand H que nous connaissons. La discussion va maintenant devoir nous permet de nous accorder sur les voies et moyens, ce qui est une autre finalité que les débats que j'ai parfois eu à l'Assemblée nationale qui nous permettront d'atteindre les objectifs militaires que nous partageons donc je le crois majoritairement. Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des sujets, l'examen en séance nous permettra d'avoir des discussions approfondies et c'est aussi pour cela que j'ai déposé une cinquantaine d'amendements du gouvernement pour que nous puissions revenir en détail à débattre utilement sur les thématiques qui méritent une attention particulière. Je souhaite prendre maintenant quelques instants. Avant de conclure pour revenir sur les questions sur lesquelles les débats doivent nous permettent de trouver un compromis et un accord, je veux d'abord revenir sur les sujets sur lesquels la version du texte telle qu'elle ressort de la commission crée un potentiel désaccord, on le verra entre le Sénat, le texte issu de l'Assemblée nationale. Je souhaite que une discussion en séance ces jours durant permettent de retravailler le texte pour répondre à la volonté du Sénat, tout en s'assurant de la cohérence du texte final quelque chose que vous souhaitez bien naturellement. Commençons par évoquer l'éléphant milieu de la pièce le sujet budgétaire, il est naturellement structurant l'ambition du texte présenté par le gouvernement était de proposer une trajectoire budgétaire au service d'une ambition militaire documentée et crédible, c'est-à-dire le fait de financer des capacités d'agir concrète en cohérence avec les menaces et la défense de nos intérêts évidemment. À cela s'ajoute notre pratique d'exécution à l'euro près. Et à vrai dire et même de sur exécution sur la fin de période, la LPM actuelle. Je suis déjà longuement revenu et qui doit nous conduire à nous assurer la soutenabilité de la trajectoire et de l'enveloppe globale pour nos finances publiques dans la durée. J'entends dire que nous reportons l'essentiel de l'effort après l'élection présidentielle de 2027. Alors je rappelle qu'en 2017, le budget des armées étaient de 32,3 milliards d'euros qu'en 2023 vous avez voté sur proposition du gouvernement, un budget de 43,9 milliards d'euros qu'en 2027 à la fin du second quinquennat. En l'état, en tout cas de la discussion d'Emmanuel Macron, le budget des armées sera de 56 milliards d'euros, soit une marge d'augmentation de 23,7 milliards d'euros par rapport à 2017 pour finalement aboutir à 68,9 milliards d'euros, ce qui aura permis de plus que doubler le budget de nos armées en de loi de programmation militaire. C'est cela la réalité de l'effort consenti par la nation, pour ses armées. Sous l'impulsion du chef de l'État. Avec l'appui du chef d'État-Major des armées. Nous avons pris le parti de privilégier la cohérence sur la seule masse. C'est au fond l'exigence de regarder dans le rapport annexé autant le tableau des contrats opérationnels que celui des équipements capacitaire, le dernier né tant au service que du premier, je le rappelle une nouvelle fois la même logique s'applique pour nos soutiens comme par exemple le service de santé des armées ou le commissariat. Il en va de même pour notre politique d'innovation qui nous permettra d'être au rendez-vous des sauts technologiques de demain. Je pense notamment aux spatial au cyber à l'Intelligence artificielle au quantique en application militaire et bien sûr, monsieur le sénateur Perrin aux drone. Le Sénat propose au delà même de la seule trajectoire une enveloppe globale financières différentes, nous y reviendrons tout à l'heure sur le terrain plus technique passant l'effort global de 413 à 420 milliards d'euros. Comme je vous le disais, je suis ouvert au débat, et je le redis solennellement ici. Mesdames, messieurs les sénateurs à à la tribune et je serai donc heureux que nous puissions avoir une discussion nourrie précise et cohérente sur ces 7 milliards d'euros supplémentaires votés en commission, mais je le redis la soutenabilité pour nos finances publiques. À ce stade de la rédaction du texte m'interroge. Mesdames, messieurs les sénateurs. Un autre point me tient à coeur et personne ne découvre à ici puisque j'y reviens à chaque fois devant vous depuis plus d'un an. C'est Claude programmation militaire ne doit pas être un carcan qui contraint nos armées et je sais que vous en conviendrez pour défendre par ailleurs plus de liberté pour nos collectivités locales. Comparaison n'est pas raison mais certaines modifications apportées en commission apporte je le crois, une forme de rigidité au texte là où une loi de programmation militaire au sens gaulliste du mot ne doit pas être une loi de prescriptions techniques, mais au contraire prendre de la hauteur et assigné objectifs stratégiques ces prescriptions peuvent créer un cadre trop strict pour nos états majors et surtout ne pas être adapté à la réalité de la ville désarmer. Or, je leur fais personnellement toute confiance et je ne doute pas un seul instant que vous aussi pour réaliser les objectifs qui sont assignés. Je pense particulièrement à la trajectoire de montée en puissance des réserves à la chronique annuelle pour le MCO et pour l'innovation, ce n'est pas eu le rôle d'une LPM, de mon point de vue que de fixer ce niveau de détail. détail. Donc, par voie d'amendement du gouvernement à ce que nous revenions à une épure plus traditionnels de ce qu'à mon sens, doit être une loi de programmation, mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont fait déjà savoir que ces modifications sont aussi des modifications d'appel pour permettre au gouvernement de prendre des engagements. Et donc là aussi évidemment je serais à votre disposition pour nourrir ces débats et les amendements du gouvernement serviront de support pour le faire. Si je suis militant pour que le parlement prenne une place plus importante en matière de défense, il faut en corollaire, que la loi reste crédible dans son exécution et plus encore dans la pratique quotidienne du ministère. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Si nous devons retravailler certains points je veux tout de même affirmé que le gouvernement soutiendra de nombreuses mesures adoptées par le Sénat qui, à mon sens enrichissent profondément le texte et renforce de manière bienvenue notre défense nationale et notre modèle d'armée, c'est en 1er lieu le cas de la mesure qui intègre les objectifs de la politique de défense dans la loi à son article 1er bis nouveau mesdames, messieurs les sénateurs, c'est important de s'y référer et c'est sur cela que l'on s'appuie en partie pour construire le reste les mesures enfin qui viennent sécuriser la trajectoire financière comme les chroniques sur les recettes extra-budgétaires ou encore le mécanisme pour les carburants opérationnels que le Sénat souhaite renforcer vont dans le bon sens même si la copie initiale de mon point de vue était solide. Mais une fois de plus grâce à vos amendements les doutes sont donc complètement dissipé et c'est une bonne chose que la commission introduite sur le sujet du service national universel même s'il nous faudra renforcer la cohérence de la légistique sur l'ensemble du texte au fur et à mesure des différents amendements du rédactionnel en quelque sorte. Vous avez souhaité mettre au clair qui ne figurait pas dans la loi de programmation militaire. C'est ce que je dis depuis le début des discussions. J'ai souscrit donc complètement et là aussi ce sont des modifications qui sont les bienvenus. Je souscris également à la volonté des sénateurs de développer des mécanismes pour mieux financer les entreprises. Monsieur le Président Cambon et et un certain nombre de, de vos collègues en particulier des PME sur lequel vous êtes revenu nombreux soit notre notre BITD, cette loi de programmation militaire ne clôture passe complètement ce chantier mais les réflexions permettront j'en suis certain de trouver des solutions adaptées pour ces entreprises qui font partie de notre modèle de défense en tout cas c'est un sujet d'actualité qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Donc là aussi je suis à votre disposition pour améliorer le texte. Vous avez enfin tenu à développer le patch sur la souveraineté dans nos Outre-mer. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur, ainsi que au président du Sénat. Par ailleurs, nous en avons échangé encore récemment sur ce point et ce sont pour la plupart des engagements que j'avais pu prendre oralement au gré des différents débats et votre version enrichie le rapport annexé. Elle est donc la bienvenue et j'ai su ce qui là aussi pleinement. C'est un signal stratégique particulièrement fort que le Sénat envoie. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Pour conclure, comme je le disais je pense sincèrement que nous sommes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce qui est bon pour nos armées les débats que nous ne manquons pas d'avoir ces prochains jours nous permettront de combler les écarts entre nos positions peut être tout simplement de mieux les expliciter donc mieux les comprendre, donc mieux les accepter qui ne concerne pas tant les objectifs que les voies et moyens pour y parvenir. Si l'on considère que le principe de réalité s'applique à chacun ce que je crois je ne vois rien d'insurmontable et je sais que la qualité du travail de cette chambre confirmera nos convictions communes et l'indispensable cohérence que nous devons préserver entre les objectifs que nous assignant à nos armées pour la protection de la nation et les moyens que nous leur attribuons pour les 7 prochaines années pour nos soldats en ayant une pensée pour les tués et les blessés pour notre nation. Car cette loi de programmation militaire doit garantir notre sécurité en assurant pour les 7 prochaines années et pour longtemps encore le succès des armes de la France, je vous remercie. La parole est maintenant. Président Christian Cambon, rapporteur de la commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Monsieur monsieur le président. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la Ministre, mes chers collègues. La défense, c'est la première raison d'être de l'État. Cette affirmation du général De Gaulle résonne gravement à la lueur des événements survenus ces derniers jours en Russie. En matière de géopolitique en matière militaire. Des bouscule ment soudain violents et imprévisibles se produisent chaque jour sous nos yeux. Et pourtant aujourd'hui il nous faut sortir de l'actualité pour nous projeter dans le temps long. C'est le difficile exercice tout à fait stimulant par ailleurs auquel nous invite l'élaboration d'une loi de programmation militaire. Une LPM ce sont précisément les moyens que collectivement. Nous mettons à leur disposition pour permettre à nos soldats d'atteindre cet objectif. Mais ce sont aussi des moyens pour prémunir nos militaires du danger auquel il s'expose. Pour nous en protéger. Face au péril nous rendons aujourd'hui hommage à leur courage à leur détermination et à alors. Compétences qui n'ont jamais fait et qui ne feront jamais défaut à la nation à travers cette loi de programmation militaire, c'est aussi la nation qui leur rend hommage. Et qui leur affirment leur soutien. Nos débats revêt donc une importance singulière et ce d'autant plus qu'ils interviennent dans un contexte de grand chamboulement. Bien sûr, nous ne pouvons placer nos travaux sur ce texte fondamental sous le seul prisme de la guerre en Ukraine car bien d'autres paramètres actuels ou en devenir devront être prises en considération. Mais reconnaissons tout de même que l'agression russe est un événement majeur qui a tout changé les équilibres diplomatiques mondiaux à la donne stratégique sur notre continent. C'est du reste précisément pour cela que le président de la République a souhaité interrompre la programmation actuelle 2 ans avant son terme pour en proposer une nouvelle. Monsieur le Ministre, il est important de rappeler ce contexte car il permet de bien comprendre la démarche de notre commission. Le point de départ logique de toute LPM. C'est l'analyse des menaces. Or si nous sommes réunis aujourd'hui et pas en 2025 pour étudier ce projet de loi c'est qu'hélas les menaces se sont accrues. Dès lors, nous nous attendions à une accélération de l'effort de remontée en puissance des moyens de nos armées. Vous le savez Monsieur le Ministre, ce sera là l'un des points principaux de débat entre le gouvernement et le Sénat. Car en l'état. La trajectoire que vous nous proposez ne marque de notre point de vue, aucune différence avec celles prévues par la LPM précédente. Ce n'est pas logique. Car si les menaces sont avérées alors les besoins qui en découle aussi le sont tout autant. Notre commission ne conteste pas l'effort louable du gouvernement et elle lui rend hommage. Le gouvernement propose en effet une enveloppe de 413 milliards d'euros répartis sur 7 ans. Au total, si cette programmation va à son terme, nous aurons bien eu plus qu'un doublement de notre effort de défense entre 2019 et 2030 ayant été rapporteur des 2 LPM je peux en témoigner ici et je souhaite que ce soit bien noté. Mais notre commission après avoir salué cet effort a aussi identifié plusieurs sujets de préoccupation. Bien sûr c'est d'abord la question de l'inflation. Vous avez évalué son impact à 30 milliards d'euros, ce qui est considérable sur l'ensemble de la programmation, peut-être même une estimation assez optimiste. C'est aussi, c'est surtout la question des ressources extra-budgétaires. Comme vous le savez notre commission s'est toujours opposé dans toutes les LPM précédente au recours à ce type de financement pour boucler les besoins de programmation. Alors certes, une partie de ses recettes affectées seront très probablement au rendez vous leur affectation. Nous sommes donc assez logique et juste. Je pense par exemple aux ressources générées par l'activité du service de santé des armées, les votes les les ventes des fréquences ou les ventes immobilières Une seconde catégorie nous paraît beaucoup plus incertaine. Ces femmes 7 milliards que le Haut conseil des finances publiques a ici pudiquement qualifiés de non documenté. Tout le problème est donc là. Monsieur le Ministre. Contrairement à ce que vous nous dites. Le Sénat est une assemblée raisonnable et très attentive à l'équilibre des finances publiques et nous n'entendons pas dépassé l'enveloppe des besoins de 413 milliards d'euros. Alors peut-être avez-vous changé la méthodologie. Mais nous restons sur notre principe simplement dans une volonté de clarté. La Commission a voulu sécuriser les crédits qui ont été annoncés comme objectif par le président de la République à Mont-de-Marsan, soit 413 milliards. Or ces 413 milliards sécurisé. Nous ne les retrouvions pas dans votre texte, naturellement, si dans le futur des marges frictionnel je des je je j'explique qu'il s'agit par exemple de retards de livraison. Si ses marges frictionnel interviennent ces crédits ne seront pas dépensés.

Dans les circonstances actuelles, le but n'est pas de préparer la guerre en Ukraine dans laquelle nous ne sommes pas belligérants. Le but, c'est de nous préparer au mieux aux menaces de demain. Alors ne perdons pas de temps. Grâce à un cadencement des dépenses beaucoup plus ambitieux renforçons immédiatement l'entraînement de nos armées les soutiens qui sont indispensables à leur efficacité est la condition militaire à un moment où la question de l'attractivité du métier des armes se pose de façon brûlante 1500 postes étaient au recrutement, 700 ont été pourvus. Les réponses de notre modèle d'armée sont encore marqués, trop hélas par les dividendes de la paix, pas suffisamment de masse, pas assez de stocks des réductions temporaires de capacité des niveaux d'entraînement insuffisants face aux objectifs nous retrouvions dans le bleu, un objectif de 147 heures d'entraînement pour des pilotes de Rafale. Les normes autant sont de 220 heures. La valeur l'engagement et le professionnalisme de nos armées sont largement reconnus par nos alliés et même par nos adversaires mais ils ne peuvent compenser les effets de 25 ans des rendements dans le cadre des dividendes de la paix avec les opérations en Afghanistan en Libye en bande sahélo-saharienne nos références ont été recentrées sur un modèle de conflits asymétriques dans le cas de la projection de nos forces. Mais c'est bien d'autres, un autre type de conflit qui est revenu au 1er plan avec l'invasion de l'Ukraine, celui de la haute intensité. C'est pourquoi à l'annonce d'une nouvelle LPM. Notre commission a voulu fonder ses choix sur une analyse rétrospective de ces dernières années et ce n'était pas regarder dans le rétroviseur. Nous avons ainsi lancé cette rapport préparatoire un retour d'expérience de l'opération Barkhane et de la guerre contre le terrorisme. Un retour d'expérience de la guerre d'Ukraine dont je souligne à nouveau qu'elle doit nous éclairer sans nous aveugler et 5 rapports thématiques correspondant à chaque problème chaque programme budgétaire intéressant nos armées. À l'issue de cet important travail préparatoire nous tirons principalement de conclusion que le texte adopté par la commission traduit concrètement. Premièrement, nous devons mobiliser plus rapidement les crédits prévus sur l'ensemble de la programmation ce cadencement révisé de nos efforts doit nous permettre de mieux financer et ce dès l'année prochaine. Tout ce qui conditionne le niveau d'activité de nos forces qu'il s'agisse de leur entraînement à proprement parler de l'entretien du matériel, des stocks ou encore des capacités du service de santé des armées nous possédons à l'heure actuelle 44. Régiment de chars Leclerc et si on met bout tabou leurs heures d'utilisation. On s'aperçoit qu'ils sont à 50% seulement de leur capacité. Parallèlement, dans une moindre mesure, nous pourrions aussi améliorer très vite les étalement de quelques programmes capacitaire tels le programme Scorpion pour l'armée de terre qui était une priorité sous l'ancienne LPM et qui a été freiné les patrouilleurs hauturiers pour redonner un peu d'air à notre marine le programme de l'A400M, 400 M pour accroître les chances de maintenir la chaîne de production et ne pas compromettre ce produit qui tient maintenant toutes ses promesses. Second axe principal de nos efforts. Les moyens de contrôle du Parlement. Monsieur le Ministre, nous le redisons ici. Le Sénat n'entend pas se substituer à l'exécutif ni empiéter sur ses prérogatives. En revanche, nous en sommes absolument convaincus, nous ne pouvons pas demander aux Français de consentir dans la durée un tel effort budgétaire sans leur garantir en même temps que le Parlement exécutera pleinement sa mission de contrôle que lui confie la Constitution pour le dire franchement l'actualisation raté de 2021 a laissé ici un souvenir assez amer. Notre commission présente donc un certain nombre de modifications qui, dans leur esprit sont du reste en cohérence avec plusieurs ajouts de nos collègues de l'Assemblée nationale. Monsieur le Ministre, il s'agit de sujet sur lequel notre commission travaille depuis de nombreuses années. Nos propositions dans ce domaine nous paraissent à la fois raisonnable et plus que jamais dans les temps que nous connaissons ces propositions sont opportunes. En conclusion, et avant d'ouvrir nos débats je souhaiterais remercier tous nos collègues qui ont participé à la préparation de ce texte si important et en 1er lieu les 11 commissaires de ma commission qui monte assister dans la préparation de mon rapport. En second lieu, je voudrais saluer, remercier les rapporteurs pour avis de la commission des Lois François-Noël Buffet et la commission des finances Dominique de Lège qui ont enrichi le texte de leur accord. Et enfin bien sûr tous les auteurs d'amendements de tous les groupes qui exprime l'importance de ce texte pour notre pays et j'ai veillé à ce que chaque groupe puisse contribuer par l'acceptation de leurs amendements à la réalisation de ce texte. Monsieur le Ministre, le Sénat est ici plein de bonne volonté avec une franche volonté d'aboutir, nous comptons bien évidemment sur votre écoute. Vous en avez fait quelques ouvertures ici il y a un instant, vous pourrez compter sur notre mobilisation mais surtout sur notre ambition pour nos forces armées. Je vous remercie.

Monsieur le rapporteur. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission de la défense sert collègue cinq minutes pour 400 milliards. Difficile d'émettre un avis circonstancié aussi si je me bornerai à vous proposer 3 considération. La première, le contexte économique général. Monsieur le Ministre, vous aimez citer le général de Gaulle dont les décisions et actions ont été marquées par le souci de l'indépendance et la souveraineté de la France. L'armée sa dissuasion il contribue au 1er plan. Mais là, cela ne suffit pas. Quelle est la souveraineté, l'indépendance d'un pays qui consacrent plus d'argent à la charge de sa dette qu'à sa défense. La dette sera supérieure de près de 10 milliards d'euros au budget de la défense en 2025. Soit. Et ce qui faisait Quelle est la souveraineté, l'indépendance d'un pays dont le déficit du commerce extérieur est 3 fois supérieur au montant du budget des armées. Déficit, dont une partie est liée à ses approvisionnements alimentaires et énergétiques quand il ne s'agit pas des matières premières indispensables à notre industrie de la défense. Je vous donne bien volontiers acte que l'actuelle LPM a été respectée dans sa trajectoire budgétaire pour autant celle que vous nous sommes. Avec la multiplication de textes programmatiques qui va se trouver en concurrence avec les lois de programmation du ministère de l'intérieur de la recherche de la justice et tant d'autres annonces transition énergétique. Accès aux soins, éducation. Le tout avec l'objectif maintes fois annoncée de réduire le déficit public pour le ramener à 3% en 2027. Une gageure, comme l'a démontré le Haut conseil des finances publiques lorsque tout devient prioritaire. Il y a urgence à faire des choix. La 2ème considération porte sur la crédibilité financière. Rien ne vous obligeait à faire une nouvelle LPM dès cet été et donc à recourir à la procédure accélérée, puisque l'actuelle loi court jusqu'en 2025. Sans contester la nécessité de l'ajuster. Pour mieux intégrer le MCO qui conditionne la disponibilité effective de nos armements et la montée en puissance du suaire. J'observe que l'ambition capacitaire de 2030 est reportée à 2035, sur fond de retour de guerre sur le sol européen. Plus. Et la trajectoire proposé puisque le président de la République qui vantera les mérites de cette loi. Dès le 14 juillet prochain n'est pas celui qui aura à trouver les milliards annoncés à compter de 2028. Laisser à d'autres le soin de financer dans 5 ans les décisions prises aujourd'hui n'est pas acceptable politiquement ni démocratiquement. Sans compter qu'une telle trajectoire des crédits seraient en contradiction avec le concept d'économie de guerre qui a introduit cette LPM et que vous avez définie comme produire plus produire plus vite et moins cher au final, on risque de produire moins moins vite et plus cher. La montée en puissance doit donc débuter dès cette législature. Par ailleurs, l'on peut s'interroger sur les fameuses marges frictionnel qui consiste à anticiper des retards de livraison ou de paiement. Les reports de charges devrait approcher les 5 milliards d'euros en 2023 avec les six de que vous projetez pour la période 2024 2030, ce sont près de 11 milliards qui manquent, soit 20% d'une année de fonctionnement ou encore un porte-. Avions qu'un besoin de financement d'un besoin financier est estimé à 413 milliards d'euros, il doit être inscrit dans la loi, il doit être intégralement couverts par des crédits budgétaires, exception faite de recettes extra-budgétaires. C'est pourquoi nous proposons de porter à minima, l'enveloppe des crédits à 407. 4 sur cette période. À défaut de garanties sur ces 2 points, une révision de la trajectoire pour la rendent plus linéaire sur la période et une réévaluation du besoin de financement plus réaliste. Nous considérons que la crédibilité la sincérité de steak ne sont pas acquise. 3ème considération sur la méthode. Monsieur le Ministre. Vous êtes en quelque sorte la victime de la manière dont le gouvernement a traité le parlement tout au long de l'actuelle LPM et singulièrement de son refus d'appliquer l'article 7 qui prévoyait qu'il serait invité à débattre de son actualisation. Nous avions cru déceler jusqu'à des propos récents que vous étiez dans un autre état d'esprit et nous nous en réjouissons mais échaudé. Nous souhaitons avoir des garanties et c'est le sens de nombreux amendements qui viennent n'ont pas modifié le rôle du Parlement, mais tout simplement veiller à lui permettent de l'assumer en disposant des procédures et informations indispensables à sa mission. La situation géopolitique, économique et social, voire intérieur requis est plus que jamais lucidité et courage tout au long de la discussion, nous serons guidée par 2 objectifs un texte de vérité plutôt qu'un texte d'affichage. Un Parlement qui entend prendre toutes ses responsabilités constitutionnelles c'est-à-dire voter et contrôlé, c'est le sens des amendements de la commission des Affaires étrangères et de la défense, dont je salue la qualité du travail, c'est le sens des amendements et précisions que nous lui avons proposé et qu'elle a bien voulu retenir c'est pourquoi sous réserve de leurs adoption la commission des finances, donne un avis favorable. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant président François Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le président. Monsieur le Ministre Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des affaires étrangères de la Défense cher Christian Cambon, chers collègues. La commission des Lois s'est saisi de trois sujets au sein de ce texte les dispositions relatives aux renseignements à la sécurité des systèmes d'information et la protection contre les drone malveillants. Tout d'abord, nous devons nous féliciter que les trois services de renseignement relevant du ministre des armées DGSE DRSD et DRM voient leurs effectifs augmenter leur investissement immobilier et opérationnel financer c'est là le premier objectif de l'autre programmation. Les dispositions inscrites dans le texte gouvernement s'inscrivent dans le prolongement des textes antérieurs. La commission des lois, les a approuvé sous réserve de précisions mais le projet de loi ne comportait aucune disposition pour renforcer le contrôle des des services de renseignement et cela alors même que l'équilibre entre l'extension des pouvoirs des services et les instruments de contrôle est essentiel à la conformité de notre régime aux exigences constitutionnelles en matière de protection des libertés et à la jurisprudence européenne. La Commission comme la commission des Affaires étrangères et de la défense. Les sénateurs membres de la DPR ont souhaité que l'information de celle-ci et le contrôle exercé par la Commission nationale de contrôle des techniques et de renseignement soient renforcées. Il s'agit d'abord de garantir que lorsque les sujets d'actualité concernant une action des services de renseignement sont révélés à la presse et ont été admis par le gouvernement ceci puisse faire l'objet d'un suivi par la délégation parlementaire au renseignement. C'est un sujet qui a pu donner lieu à divergences les différentes interprétations entre la délégation et le gouvernement l'année dernière mais qui depuis a fait l'arbitrage n'a fait l'objet d'un arbitrage au plus haut niveau de l'État que nous consacrons désormais dans la loi. Les ajouts apportés au stade de la commission des affaires étrangères de la Défense permettent également de renforcer les Liens entre la DPR et la CNCTR en prévoyant la présentation à la délégation d'un bilan annuel des recommandations de la commission, ainsi que son information sur les saisine du procureur de la République dans le cadre des dispositifs de lanceurs d'alerte. Enfin le dernier amendement tend à permettre l'accès immédiat de la SNE, c'était la CNCTR aux éléments collectés par les services de renseignement lors de la mise en oeuvre des techniques les plus intrusive dont il faut souligner que nous ne contestons pas, nous Je note d'ailleurs que le gouvernement souhaite la suppression de cet article 22 quater pour des raisons de principes et de calendrier sur les principes, il est important que le développement des techniques les plus intrusif s'accompagne d'une amélioration des moyens de contrôle. Ce que nous ne souhaitons, ce que le Ministre, il est bien sûr nécessaire de prendre en compte les contraintes opérationnelles, nous pourrons donc il y revenir. Il n'est pas question de placer en difficulté nos services dans des sites qui, ce qui ne serait pas naturellement acceptable compte tenu des projets et des objectifs que nous partageons dans la même logique afin d'éviter l'émiettement du contrôle. Nous avons souhaité que la CNCTR puisse donner un avis avant la prise des décrets renforçant les pouvoirs de l'Inde. Si en effet et il faut le redire à ces tribunes l's'il n'est pas un service de renseignement. Elle n'est pas un service de renseignement ses Liens avec ceux-ci sont étroits et la nature de son intervention à peine un regard informé par la pratique de ces services. Un mot enfin. D'un sujet qui va peser dans le cadre légal du renseignement le régime encadrant les échanges d'informations entre les services français de renseignement les services étrangers. C'est un sujet extrêmement sensible à telle enseigne que nous n'avons pas souhaité et je n'ai pas voulu, il a intégré dans le texte. Le sujet par voie d'amendement, en revanche il faudra dans un délai assez rapide, que les choses puissent être réglés. La délégation parlementaire au renseignement reste je le crois. Le lieu d'échange, le plus efficace sur ce sujet. S'agissant de la sécurité des systèmes d'information. Les articles 32 à 35, renforce la capacité de lancer de détecter identifier et prévenir les attaques informatiques visant les systèmes d'information des autorités publiques des opérateurs stratégique ou de leurs sous-traitants ces dispositions vont dans le bon sens d'une meilleure défense de la France et nous ici ils vont été favorable sous réserve de quelques précisions s'agir d'un régime de lutte contre les drone malveillants. L'article 27 du projet de loi vise à doter nos services de l'État de moyen de parer sans délai à des menaces imminentes. Il a par là. Il a paru à la Commission nécessaire de renforcer les garanties en ce qui concerne notamment les droits de propriété, le droit d'informer. Un amendement a été déposé dans ce sens. Sous réserve de ces amendements qu'elle a soumis et qui ont été adoptés par la commission des lois à la commission des lois, considère que le projet de loi et puis il y a naturellement par la commission de la défense. Monsieur le Président, je m'excuse de l'avoir omis a considéré que le projet de loi comporte des mesures utiles pour les services de renseignement et pour la sécurité des systèmes d'information et a donc émis un avis favorable à l'adoption de ce texte. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer à la discussion de la motion qui tente à opposer la question préalable. Monsieur Pierre Laurent et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée numéro 37 qui tente à opposer la question préalable. Je vais donner la parole au président Pierre Laurent pour la motion. Merci, Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Avec cette question préalable le groupe CRCE souhaite poser à notre Haute assemblée une question simple et Thierry vraiment sérieux de débat dans ces conditions, d'une loi de programmation militaire d'un montant exceptionnel de 413 milliards d'euros. Son ampleur le tournant stratégique qu'elle opère son poids énorme face à tous les autres au budget de la nation pour le climat à la réindustrialisation, le logement, la santé, l'éducation. Tout appelait à ce qu'elle fasse l'objet d'un large débat avec la nation. Le terme initial de l'actuelle LPM en 2025 le permettait. Monsieur le Ministre, le 22 mai à l'Assemblée nationale vous avez vous-même déclaré que cette LPM et je cite un défi aussi important que celui qu'ont dû relever les gaullistes dans les années 60. C'est vrai, mais avec une différence de taille, le général de Gaulle installaient alors le choix de construire à l'indépendance de notre défense. Vous faites aujourd'hui, celui de l'OTAN nisation et de la guerre. Le débat démocratique sur vos joies vos sur vos choix n'ont n'était donc plus impérieux. Mais vous en avez décidé autrement. Le président a confisqué l'évaluation stratégique, préalable nécessaire à toute LPM. Il l'a réduite à l'écriture en cercle restreint. D'une revue nationale stratégique jusqu'ici sous la Ve République. Les grands tournants de la stratégie militaire française ont tous été pris suite à la publication de livres au Blanc. Je ne vous apprendrai pas que les communistes constant et cohérent attaché à une défense nationale indépendante ont souvent fait valoir des désaccords essentiels avec les orientations de ses livres au Blanc. Mais ces documents avaient au moins le mérite de permettre un débat stratégique national d'ampleur. Animé par une commission dédiée associant pendant une année entière la représentation parlementaire les grandes administrations de l'État et Les hiérarchie militaire la plus rien. Une consultation confinant à la parodie avec un questionnaire remis aux commissions parlementaires 12 jours avant le discours de Mont-de-Marsan. Voilà la tare originelle de cette LPM elle porte la marque d'un grave défaut de conception démocratique. Pour cette question préalable, je m'en tiendrai à 3 critiques majeures et je tenterai de vous convainc chers collègues de la nécessité de reprendre le débat sur d'autres bases. Car une autre politique de défense et possible pour notre pays. D'abord cette LPM nous on nous éloigne des objectifs de défense de la nation au profit du choix de la guerre et en l'occurrence de la guerre projeté hors de nos frontières. Avoir une guerre d'avance c'est votre nouveau mantra. Derrière le panache apparent de cette formule, se cache un profond défaitisme un choix dangereux pour la sécurité collective. On nous dit que la paix n'est plus une option qu'il faut prendre place dans la grande dérive militariste mondial. C'est oublier toutes les leçons du 20ème siècle la militarisation et le surarmement singulièrement en Europe ont toujours préparé la guerre et bien pire encore jamais la paix. C'est oublier toutes les leçons des 30 dernières années. Après la chute du mur, le monde n'a pas été on paie l'Occident a usé de sa puissance pour multiplier les guerres, guerre du Golfe, ex-Yougoslavie, Afghanistan, Irak, Libye Sahel pour quel résultat. Le chaos, l'insécurité, la déstabilisation durable des États et la militarisation des sociétés jamais la paix durable. C'est oublier enfin que la guerre affame les peuples et nourrit les fauteurs de guerre dans ce chaos prolifèrent, les monstres et les entrepreneurs de violence terroriste milices et société paramilitaire privée. Trafic de drogue et d'armes traite d'êtres humains nationalisme guerrier et impérialismes régionaux extrême droite et radicalisme religieux, le surarmement nourrit la guerre il ne la désarme jamais. Les arsenaux nucléaires prolifèrent à nouveau le réarmement Naval est à un niveau inédit depuis 45, les Budgets militaires Expro explose en Europe comme au Moyen-Orient et en Asie. Face à la Chine, les États-Unis veulent entraîner tous leurs alliés dans un dangereux continuum compétition économique guerre militaire. Quant à la Russie elle s'enfonce dans une guerre en Ukraine au coût humain, économique et militaire astronomiques aux conséquences imprévisibles pour l'Europe et pour elles-mêmes. Comme vient de le révéler l'incroyable épisode de la rébellion Wagner. Quand allons-nous nous réveiller quand allons-nous cesser cette insupportable banalisation de la guerre. Pour notre part, nous appelons toutes les consciences libres à Saint-Georges et contre cette folie car d'autres chemins sont possibles pour le monde. Vous allez me dire que nous sommes naïfs que la menace partout que la guerre en Ukraine dit qui est l'ennemi et qu'il faut bien re- riposter se réarmer dans tous les domaines. Oui, le monde a effectivement changé et les menaces sont nombreuses. Mais vous vous trompez sur le diagnostic, le diagnostic de ces bouleversements et les moyens de conjurer les menaces, vous vous trompez d'époque. La guerre de Poutine en Ukraine n'est pas le symptôme le symptôme du retour des blocs d'hier. C'est un signe de plus de la décivilisation du monde qu'entraîne la militarisation des relations internationales et l'affrontement de plus en plus violents, des logiques de puissance. Le chaos mondial et paradoxalement le résultat d'un monde plus interdépendants. Mais en même temps toujours plus inégale pour relever les grands défis mondiaux tout appelle le partage et les plus riches le refuse la loi du plus fort la puissance militaire ne régleront plus les problèmes, bien au contraire. Faut-il suivre alors les États-Unis ou tout autre d'ailleurs dans l'escalade militaire, faut-il les suivre quand ils cherchent à déstabiliser toute puissance émergente pour maintenir coûte, coûte que coûte leur Leadership planétaire est la voix que la France doit suivre. Je ne le crois pas et c'est la 2ème conviction je veux partager avec vous. La stratégie d'alignement, derrière les États-Unis et le bloc occidental que poursuit de facto cette LPM et dangereuse pour notre pays pour l'Europe et pour la paix mondiale. Les paradoxes apparents de la LPM souligné d'ailleurs dans les débats de la commission des affaires étrangères du Sénat n'en sont pas. Dissuasion nucléaire porte-avions espace fonds marins dans tous les modes domaine cette LPM court après la sophistication militaire au risque d'y perdre notre boussole et la mesure de nos moyens réels. Et tout cela au titre d'une haute intensité en vérité uniquement entendu comme la capacité de projection de nos armées dans des opérations militaires de l'OTAN hors de nos frontières. L'intégralité du vocabulaire du concept stratégique de l'OTAN révisé à Madrid et à Madrid. Et d'ailleurs recyclés dans la LPM. L'OTAN nisation complète de l'Europe est en cours. Elle met à bas toute velléité d'autonomie stratégique européenne. Elle finance en 1er lieu les industries américaines de l'armement. Le Bloc atlantiste n'offrent pourtant qu'une cohérence de façade. Et est incapable d'enrayer les velléités bellicistes et expansionnistes de certains de ses membres. La Turquie d'Erdogan à l'opportunisme géopolitique décomplexé en dans l'exemple le plus criant. Et que dire de nos alliés des monarchies du Golfe. Que dire en Europe même, de la Hongrie, de la Pologne de l'Italie et du poids grandissant dans ces pays d'extrême droite raciste et militariste. Pour notre part, nous vous proposons de remettre la LPM en chantier car ces objectifs se trompe de cible sur le monde à construire vous sauter comme des cabris la guerre, la guerre, la guerre. Mais vous ne voyez pas le nouveau monde qui. Qui s'avance quand accepterez-vous d'entendre qu'une majorité de peuples du monde ne veut plus avoir à s'affilier à telle ou telle superpuissance. Les peuples aspirent à maîtriser leur destin à disposer de souveraineté pleine et entière à décider librement de leurs alliances et coopération. Vous restez accrochés à vos vieux schémas hors de l'OTAN. Vous ne voyez que la main de Moscou ou celle de Pékin, quand tant de pays en réalité cherche de nouveaux partenariats plus équilibrés. Comment pouvez-vous ignorer que les insécurité sanitaire alimentaire énergétique climatique que l'absence de partage réel de la gouvernance politique de la mondialisation sont au coeur de tous les conflits et par conséquent à la racine de toutes les guerres, entendez le constat lucide du secrétaire général de l'ONU. Si nous ne nourrissons pas les gens nous nourrissons les conflits. Vous persistez à nauséabond avec des mécanismes qui ont échoué à construire la paix, 20 ans de guerre au terrorisme s'achève par le départ des troupes américaines d'Afghanistan. En proie à la famine. Ce pays est devenu un narco-État pour financer la guerre sous domination des talibans. 10 ans de Barkhane au Sahel non il éteint le djihadisme ni permis le développement de la région il est temps de changer de paradigme. L'agenda pour la paix et la sécurité collective. C'est la construction d'une sécurité humaine globale répondant aux besoins vitaux des populations leur permettant de cohabiter en paix dans la durée et autour de perspectives de développement. La France dispose encore d'une voix écoutée dans le monde. Utilisons-là pour relancer tous les processus de désarmement multilatéraux conventionnel comme nuque comme nucléaire utilisons-là pour clamer le droit à la paix ce mot que certains voudraient aujourd'hui tabou. Jamais nous ne nous rallierons à cette affirmation absurde selon laquelle est désormais dépassé le temps des dividendes de la paix. Mais non seulement la paix n'a pas de prix mais elle est et restera le seul horizon raisonnable pour l'humanité. C'est pourquoi constant et cohérent. Nous saurons tout au long de ces débats animés par une double conviction garantir à notre pays, une défense souveraine et solide et agir en même temps pour que grandisse partout des coalitions de la paix. Je vous remercie. Merci monsieur le président. Y a-t-il un orateur contre la motion. Je ne vois point. Quel est l'avis de la commission, monsieur le président. Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la Ministre, mes chers collègues. Je pense qu'il est utile de resituer cette motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de programmation militaire dans son contexte. Il y a un an à la fin du printemps 2022, le président de la République a estimé que l'agression de l'Ukraine par la Russie était un événement d'une telle ampleur géopolitique qui imposait d'arrêter prématurément la LPM 2019 2025 pour adopter une nouvelle programmation militaire chacun peut penser ce qu'il veut de cette décision. Certains disaient puisque la LPM précédente prévoit déjà des marges d'augmentation de crédits à 3 milliards, allons au bout de cette LPM et nous en ferons une nouvelle en 2025 lorsqu'on aura une vision plus claire de la situation nouvelle le projet de loi a été déposée après une revue stratégique qui n'a pas franchement convaincu ni par sa méthode ni Monsieur le Ministre par ces groupes de travail préparatoire à la LPM ni par son calendrier jugé parfois précipitées ou en tous les cas trop resserré pour permettre un travail approfondi. Ni enfin par ses conclusions succincte qui n'aborde pas la question fondamentale qui nous est posée aujourd'hui quel modèle d'armée, voulons-nous pour la France pour les années qui viennent. Ou pour dire les choses en termes plus politique et moins militaire. Quelle est notre ambition pour la France dans un monde de plus en plus instable et dangereux. Et avec quels moyens. Ces constats dressés amène le groupe CRCE à déposer une motion tendant à opposer la question préalable. La commission ne la votera pas et appelle bien évidemment le Sénat à ne pas la voter et ce pour 2 raisons. Nos concitoyens s'attendent légitimement alors que la guerre frappe de nouveau le sol européen que nous débattions sereinement des moyens mis à la disposition de nos forces armées. Nos armées attendent des adaptations nécessaires pour se préparer à la haute intensité et à l'hypothèse d'engagement majeur nos industriels ont besoin de visibilité requise par l'émergence de la notion d'économie de guerre. Ce que propose le projet de loi, nos alliés et nos partenaires mais aussi nos compétiteurs et sûrement nos adversaires sont attentifs aux signaux que nous enverrons en examinant ce projet de loi le 1er signal sera celui d'un Parlement investi ce fut le cas à l'Assemblée nationale, ce sera aussi le cas au Sénat. Je crois que nous pouvons raisonnablement dire que nous ne l'avons que nous n'aurons jamais autant préparé et aussi en amont une LPM. Nous avons certes écarté la méthode proposée par le gouvernement mais le bureau de la commission avait choisi de lancer. Pas moins de 7 rapports d'information. Je l'ai évoqué il y a un instant sur la guerre d'Ukraine Barkhane et chacun des programmes concernés et je souhaite ici à nouveau rendre hommage à toutes celles toutes celles et ceux d'entre vous qui a enrichi la réflexion de la Commission par ses rapports très riche, très fouillée et important. Comme président de la commission. Je suis évidemment fier des conditions dans lesquelles a été menée ce travail colossal. Je suis tout aussi fier de l'esprit dans lesquels ces travaux ont été menés, fait du respect de chacun et d'esprit républicain qui associés tous les groupes, je dis bien tous les gros. Je pense que cet esprit de responsabilité. Ce consensus républicain autour d'un socle de valeurs partagées au-delà de nos sensibilités politiques légitimes. C'est la marque de fabrique du Sénat et elle contribue au rayonnement de notre assemblée. Nous sommes donc prêts et nous avons débuté en commission le travail d'examen du projet de LPM le 14 juin dernier de commission, celle des lois et des finances se sont saisis pour avis. Nous avons adopté 171 amendement pour établir le texte de la commission dont d'ailleurs 11 amendements du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. C'est donc un texte déjà largement améliorée par les commissions par les groupes politiques, dont nous allons sereinement débattre et que nos armées attendent, elles en ont besoin ne différent ne différons donc pas le débat et le travail parlementaire sur ce texte essentiel dans un contexte géopolitique si différents et si dangereux par rapport à ce qu'il était en 2018 lorsque nous avons voté la précédente LPM je conclus donc bien évidemment au rejet de cette question préalable déposée par le groupe CRCE je vous remercie. Merci. L'avis du gouvernement. Féministes. Oui, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président Laurent pour le gouvernement c'est un. Un avis évidemment défavorable et une demande que le Sénat rejette cette cette question préalable. Tout simplement parce qu'elle n'aurait qu'un seul effet c'est de ne pas permettre le débat. Et si j'en crois ce qui a été dit à de nombreuses reprises en commission dont vous êtes membre d'ailleurs par ailleurs ce qui est dit ici ou là dans la presse à l'Assemblée nationale, c'est que la démocratie représentative précisément elle a besoin de s'emparer de ce sujet de cette question du modèle de sécurité collective que nous voulons défendre. que nous ne soyons pas d'accord sur la dissuasion nucléaire, que nous soyons pas d'accord sur nos alliances qu'une fois, il n'a pas d'accord sur les coopérations industrielles que ne soyons pas d'accord sur le modèle économique de nos industrie ça sera le temps du débat mais adopté cette question préalable c'est tout simplement. Mettre. Quelque part au au classeur cylindrique pardonnez-moi cette expression. Cette loi de programmation militaire dont malheureusement nous ne pourrons pas opposer une question préalable aux menaces qui pèsent sur la nation française et elles sont d'actualité. Ça a été dit par le président Cambon. Il y a une accélération stratégique parfois pour remettre au goût du jour. Malheureusement des problèmes sécuritaires que nous connaissions jadis du temps de la guerre froide ou des questions qui sont posées autour de la prolifération nucléaire parfois certaines menaces continuent malheureusement de se faire sous nos yeux et plus personne n'en parle suffisamment et je le redis, merci pour le débat qui a été demandé par le groupe socialiste sur l'Afrique parce que la question de terroristes doit continuer à nous mobiliser et il faudra bien qu'on y apporte des réponses et qu'on continue d'y apporter des réponses que nous avons pardon mais des sauts technologiques. C'est pas une affaire de choix politique. C'est tout simplement que ces sauts technologiques s'impose à nous la militarisation du cyber, on ne peut pas d'un côté déploré les attaques que les différents hôpitaux français ont pu connaître sur un terrain plutôt. Cybercriminalité et ne pas voir que demain le cyber à une utilisation est évidemment une traduction en matière militaire. On ne peut pas ne pas voir la militarisation de l'espace que l'on peut regretter sur le terrain des valeurs mais qui néanmoins va s'imposer à nous, y compris sur l'ensemble de nos infrastructures civiles. La question des fonds sous-marins, la guerre des mines. Bref, autant de sujets dont il était peu question dans cet hémicycle en 2018 et pour cause puisque les technologies nous ont rattrapés et c'est ce qui explique aussi ce pourquoi nous nous retrouvons avant même le terme la loi de programmation militaire actuel puisque au-delà même de la guerre en Ukraine, un certain nombre d'éléments nous conduisent à de nouveau sollicité la représentation nationale, et pas que pour une trajectoire budgétaire et pas que pour des aspect normatif mais aussi pour soumettre des orientations politiques nouvelles qui pivote en quelque sorte. Aussi pour notre modèle d'armée. J'ajouterais aussi pardon mais que ce texte comprend des mesures qu'on pourrait qualifier de social pour la troupe. Revalorisation des grilles indiciaires indemnitaire je vois mal comment le gouvernement aurait pu les mettre en oeuvre en loi de finances sans repasser par une mise à jour, à minima, la la programmation militaire et mieux une nouvelle loi de programmation militaire. C'est ce que nous faisons donc demande de, de Roger et d'opposer justement à cette question préalable le fait de pouvoir conduire un débat sur lesquelles on pourra examiner l'ensemble des amendements y compris les vôtres et qui permettra de mieux redessiner des modèles de sécurité qui certes ne seront peut-être pas les mêmes. Je le dis moi moi même j'ai pris les devants à la tribune mais qui au moins viendront s'nourrir la méthodologie qui a été la nôtre. Merci au président quand d'avoir dit que jamais une LPM n'a été. Autant. Préparée certes pas comme d'habitude on y reviendra, mais au moins, pour le coup il y a un foisonnement de contribution les rapports parlementaires ont tous été intégré aussi dans la réflexion globale. Et moi je saurai défendre les choix militaires qui ont été retenus, proposée par les états majors au président de la République est telle que vous voulez retrouver dans notre programmation tels que vous est soumis demande de Roger. Merci. Explications de vote. Je rappelle qu'il y a une explication de vote par groupe monsieur et. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la Ministre, Monsieur le président de commission. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Notre groupe voudrait mettre en exergue un certain nombre d'éléments qui permettent de s'opposer à cette motion. Tendant à opposer la question préalable. Lorsqu'on parle de d'immaturité du texte. Je voudrais rappeler que ce texte il a été élaboré sous l'autorité déjà du président de la République, chef des armées dans la concertation en étroite relation avec les militaires. La direction générale de l'armement avec les directions de nombreux ministères en raison de sa transversalité, mais aussi très en amont et je tiens ici à saluer votre démarche. Monsieur le Ministre, avec nos deux chambres du Parlement et les acteurs du monde de la défense en général. Ce texte il cherche également à répondre à un enjeu fort de sécurité de souveraineté et à traduire une conviction simple à celle des menaces qui pèsent sur la nation et qui n'ont jamais été aussi protéiforme qu'elles ne le sont actuellement. À bien des égards, elle place la France face à des défis majeurs qui oblige à anticiper et à prévoir ces lois de programmation militaire nous oblige à bien des égards mais je retiendrai personnellement de points qui me semble particulièrement important de souligner tout d'abord il s'agit d'une loi de programmation qui comme son nom l'indique va se mettre en place de manière cohérente. Posé sur un certain nombre d'années la programmation et le geste stratégique par excellence, nous indiquait dernièrement le président à Mont-de-Marsan. Je crois qu'aucune politique sérieuse ne peut se passer de vision à long terme, il faut voir loin et les enjeux et défis d'aujourd'hui justifie amplement les efforts qu'il nous faut mener demain. Elle nous oblige également au regard des sommes engagées, 413 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et si ce chiffre peut parfois être critiqué discuter tiraillée tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agit pas de dépenses passives. Il faut rééquiper et moderniser nos armées, leur donner les capacités de se défendre et d'agir dans des champs hybride espace fonds marins cyber en incluant les fonds international pour tous c'est pour toutes ces différentes raisons à ces différents éléments. Notre groupe s'opposera à la motion tendant à s'opposer à la question préalable. Je vais dormir. Pas d'autres demandes d'explications de vote. Je vais consulter le Sénat sur la motion tendant. À opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte, en discussion.

Dans la suite de notre discussion générale je vais donner la parole. Notre collègue Rachid Temal. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Messieurs les rapporteurs. Mes chers collègues. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour évoquer la loi de programmation militaire pour les années 2024 2030. Permettez-moi tout d'abord à cette occasion de saluer l'engagement le professionnalisme des femmes et des hommes qui composent nos forces armées. Qui parfois malheureusement connaissent la mort et pour défendre à la fois je l'ai dit, notre pays et nos intérêts vitaux. Je vais essayer de résume mon propos en 3 points. D'abord le contexte de cette loi de programmation militaire. Ensuite, bien évidemment, son contenu et ensuite j'ai envie de dire le travail du Sénat puisque nous reviendrons sur effectivement ce que nous avons porté collectivement. Monsieur, vous évoquiez tout à l'heure le fait d'une loi de programmation militaire c'est effectivement à la fois un temps long. On sait quand on lance des programmes c'est parfois pour 30 40, 50 ans et en même temps des temps relativement courts. Et d'ailleurs nous sommes en secret de voilà tout ce que parfois. D'une prise en fait à une autre, il faut revoir cette loi de programmation militaire parfois une effectivement de la revoir de la reconstruire de l'image un nouveau. Et pour cela, permettez-moi de revenir sur quelques dates pour dire comment le monde peut changer en 30 ans. Et se dire comment se fait la projection. D'abord effectivement beaucoup de gens, elle évoque qui voulaient bloquer le ce midi sur. Les disons de la paix aussi le monsieur le rapporteur. Mais là aussi je crois que c'était une réalité pour tout le monde, pour tous les bancs de tous les hémicycles quand le mur est tombé le 9 novembre 1989. Je crois que chacun. Légitimement a pu penser que, d'ailleurs c'était même touristes sur la fin de l'histoire que un nouveau temps pouvait s'ouvrir et ce ton-là, c'était celui de la démocratie en tout cas sur le continent africain et la capacité à à être dans une autre logique. Chacun a pu voir depuis la suite. Autres dates sur lequel je veux m'arrêter un instant s'également sur le 11 septembre 2001. Effectivement c'est un temps qui vient, gravement perturbé, on le voit, vous l'avez dit tout à l'heure la question du terrorisme. D'abord dans une forme que nous avons vu, je l'ai dit le 11 septembre des attentats aussi en Europe et dans le monde occidental. J'ai envie dire mais également d'études terroristes qui continuent à perturber encore et encore on voit sur la question de l'Afrique, vous l'avez évoqué, on l'évoquera tout à l'heure sur la question de Barkhane sur la question de la présence encore la France en Afrique sur la question du redéploiement de nos bases. Et puis aussi le 15 août 2021. Le départ des troupes d'attente américaine du de Kaboul. Parce que là aussi c'est un sujet aussi important. Je crois qu'on a, on peut passer sous sous les radars. C'est la question de l'implantation et la conviction. De cette force que sont les États-Unis d'être ou non dans une logique, à la fois d'être et c'est toujours leur leur leur réflexion être dans le monde ou être dans leurs frontières et ça c'est un élément aussi que nous devons garder l'esprit au-delà de simplement d'une élection préenseigne note avec élection présidentielle mais ça veut dire que leur volonté. Autre date. Le 24 février 2022. Je l'évoquerai tout à l'heure bien sûr. C'est la question. Déclenchement de la guerre en Ukraine, avec pour la première fois une force dotée de l'arme nucléaire qui décide sur le africain de passer ses frontières de semer le doute ou le chaos. Avec les conséquences que nous connaissons et puis une date peut être pour l'avenir. J'ai envie de parler de du de l'année 2049. 2049 c'est le centenaire de la République populaire de Chine. Mais c'est également la question. De son rapport à Taïwan. Et donc ça nous renvoie la question d'entre aujourd'hui et 2049. Sur la position de la Chine. Chacun a pu entend des déclarations du président, 1er secrétaire du Parti communiste chinois par ailleurs responsable des forces armées mais son annonce très clair.

Qu'il faille revoir notre loi de programmation militaire. Et donc chacun peut imaginer effectivement je crois qu'il y a un travail pédagogique doit être fait. J'en dirai un mot telle heure sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Et là je ne parle encore que quelques dates, on y ajoute bien évidemment la question des États désemplir contrarier la Chine, la Russie. Je vous rappelle que. Depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, les rencontres entre les deux dirigeants sont massives régulière, on le voit d'ailleurs maintenant ce qui se passe sur la guerre en Ukraine sur les Liens entre les 2 pays. y a pas cela c'est vrai qu'il nous faut réfléchir cette façon-là donc les empires contrarier je voudrais j'bien sûr la Turquie. On voit bien d'ailleurs qui aujourd'hui, avec la réélection. Malheureusement de son président, cette volonté de pousser les pions, on le voit notamment sur le continent africain qui soit en Libye ou ailleurs. En Ukraine, c'est vrai que la donne a beaucoup changé. Puisqu'on le voit, je l'ai dit, un pays doté de l'arme nucléaire décide d'envahir. Qui parfois fait pour le le président Poutine fait du chantage à la dissuasion nucléaire à l'armement nucléaire. Nous avons aussi une réflexion sur les conflits d'haute intensité sur également nos armes diverses et variées qui sont aussi positionnés. J'ajoute l'indopacifique. Nous avons quand même plusieurs questions sur ce volet-là. D'abord nous avons une question de même de présence française. Quand je revois les résultats électoraux en Nouvelle-Calédonie et dans la pacifique. Également, je l'ai dit la volonté chinoise de pousser les pions. Nous sommes aujourd'hui sur des niveaux de construction. Par exemple la flotte chinoise fait seulement la moitié seulement de la flotte, la flotte américaine, on voit les progressions sur les dans les mers sur sur l'avenir de la volonté chinoise et donc se pose la question, la France, qui je le rappelle, est la seule puissance européenne soit un continent offrir indopacifique se pose la question de son rôle de sa présence de non pas de sa capacité à porter le fer, le cas échéant au niveau de la Chine. Ben dis donc mais en tout cas, de protéger ses territoires et sa zone économique spéciale qui la plus vaste du monde. Je crois que vraiment qu'il faut apporter et 7 la volonté que nous avons c'est cette loi de programmation militaire, il répond. J'ajoute un mot sur le continent africain. Bien souvent oubliés. Qui pour le coup est bien souvent le lieu de la sous-traitance d'ailleurs j'ai envie de dire là avec la présence, je l'ai dit forte des Chinois. Des Russes. Nous avons, je crois que Monsieur mise à évoquer ou je sais plus qu'interlocuteur a évoqué la question de Wagner des derniers jours. Je rappelle, se pose la question de la suite de la Miss Wagner dans un non certain nombre de pays africains. pays où ils viennent à la fois spolier les populations parfois martyriser les populations mais également surtout capter les le le sous-sol éliminerait et donc là aussi se pose la question. Notre propre présence. Vous l'avez évoqué, c'est la première LPM depuis la fin de l'opération Barkhane. Ce n'est pas neutre. Depuis l'annonce qui a été faite de redéployer nos bases et c'est vrai que, à ce stade, nous allons parler d'une peine. Nous n'avons pas trancher cette question là, je crois que ces éléments qui me semble important. Et puis pour ne pas être trop long, je pourrais évoquer bien sûr la prolifération nucléaire et cetera mais je voudrais dire un mot aussi sur la question du Sud global. Puisque c'est la première LPM aussi. Où pour la première fois et on l'a vu à l'occasion d'ailleurs du vote des différents votes aux Nations unies sur la question de l'Ukraine. Pour la première fois ce qu'on appelle le Sud global a décidé de ne pas suivre et ne pas voter, ne pas condamner l'invasion de la Russie en Ukraine. Qui décide ce ce global. De changer les normes en disant que les règles occidentales sont trop importantes, ce Sud global qui décide dorénavant d'avoir sa propre monnaie et on voit bien que la question de la puissance occidentale aussi militaire maintenant est largement posée. Alors une fois que j'ai dit ça sur ce contexte là, quelques mots sur la loi de programmation. Vous l'avez dit, monsieur le Ministre, c'est la 15ème. Alors vous citez souvent le général de Gaulle et comme je vous le dis à chaque fois on peut parfois. Comment. Tout à fait mais vous savez souvent général de Gaulle et je vous le dis à chaque fois on pouvait à la fois gaullien sur cette gaulliste. Et donc c'est vrai qu'on peut se satisfaire effectivement du choix. J'ai voulu d'ailleurs la LPM du général De Gaulle, convenons-en, c'était d'un autre niveau que celle que nous avons aujourd'hui devant nous Ce n'est pas un sou séances là mais comme vous le savez aussi. Ce qui a fait que la LPM Les LPM et la logique notamment dissuasion nucléaire et d'armes conventionnelles a aussi pu être poursuivi sélections de 1980 puisque là aussi, François Mitterrand a fait le choix lui aussi. Deux totalement porter ce concept là d'ailleurs en allant jusqu'au bout de la dissuasion nucléaire en expliquant que ce qui faisait la force de son nucléaire, c'était le président de la République. Le reste était de choses n'était que matière inerte et donc je le dis comme ça parce que je sais souvent que vous citez le général Gaulle permettra de rappeler que ma famille politique. François Hollande. L'an dernier, juste avant Lionel Jospin. Et encore, François Mitterrand ont été aussi les artisans fortement important d'une dissuasion nucléaire d'une armée à la hauteur des des enjeux et de la défense de notre territoire. Je crois que c'est important de le rappeler mais pour ne pas être trop long sur ces questions là. Comme l'ont dit certains de mes collègues le souci avec cette LPM. C'est que le Sénat est aujourd'hui un peu. Inquiets interrogatifs parfois chagriné parce que nous avons l'instance de l'actuelle loi de 3 hommes. La programmation militaire. D'abord parce que oh, certains l'ont dit, nous avons souhaité une remise à jour. Elle nous a été refusé. Il faut le dire. Nous avons souhaité dans la construire de la nouvelle que le Parlement puisse j'ai tout son rôle. Ça nous a pas été possible puisque encore une fois il n'y a pas eu de livre blanc. Il y a eu une revue nationale stratégique fait en chambre sans le Parlement et c'est vrai que le Parlement bien sûr fait la loi, mais aussi à la question du contrôle du gouvernement et sur l'évaluation des politiques publiques. Une fois je vous dis ça je pourrais évoquer la question financière. Alors je pourrais vous parler de pour 100. Je pourrais vous parler des 7 milliards, je pourrais parler 13 milliards chacun. Mais je vais dire un mot quand même sur le montage financier. Parce que si on prend les 413 milliards. Mettons de côté les 13 milliards. Il nous reste 400 milliards de crédits budgétaires. Convenez avec moi que l'année 24 25. Qui devait être ceux qui ceux qui sont dans l'PMC grosso modo 97 milliards. Qu'on compte quasiment deux fois. S'y ajoute à ça les 30 milliards. D'inflation. Je mets de côté à ce stade. Les 100 milliards de reports de charges que vous venez avec moi, que les besoins de financement sous quand même réelle devant nous et j'ajouterai pourrait pas faire trop long que nous aurons Nexon présidentielle en 2010 et en 2027 et force est à parier parce que la condition est ainsi rédigé, même si je crois que certains pas changer. Je ne crois pas que ce sera le cas nous aurons un nouveau, une nouvelle prison public qui est aussi fera une nouvelle programmation militaire et par ailleurs pour pas être trop long sur ce sujet. Cet aspect-là des choses, vous savez bien que quand on y ajoutera le fait que. la facture sera payé par la la suivante majorité tout, vous voyez que ça va être un peu plus complexe. Mais moi ce qui me choque ce qui ne pose pas la sauce stade. Je crois qu'il faut être honnête. Une autre majorité aurait également une armée complète. C'est ce que nous souhaitons. Dissuasion conventionnelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Chacun est tenu par les finances publiques. Donc nous serions à peu près dans l'épure et donc se pose la question. Certains diront une armée complète et miniature un bonzaï chacun y mettra les mots qu'il souhaite donc la question à partir de là, c'est notre capacité à agir seuls ou j'en j'en veux dire accompagné et je trouve et c'est là d'ailleurs que j'ai le regret sur le Livre blanc c'est que nous ne pourrons pas voir dans ce cadre là, le vrai débat, à mon sens c'est que doit faire la France pour maintenir sa capacité de défense et d'armement. Quel rapport effectivement le ton et on le voit ces derniers jours. Moi je suis pour une grande part avec mon groupe favorable, elle est beaucoup plus loin dans le temps et je le dis être dans le temps, ce n'est pas redire son indépendance ce n'est pas réduire sa capacité à agir, ce n'est pas réduire sa capacité à décider, ce n'est pas mettre en partage. La dissuasion nucléaire, bien au contraire. Mais quand je vois les Allemands qui ces derniers jours ont été pilote pour la question de la protection sur le j'veux dire le le la protection missile voyez bien c'est ce que devrait faire la France et c'est dommage qu'on puisse pas le faire dans un texte législatif, c'est-à-dire comment on, soit on soit leader dans l'OTAN. La ensemble de grandes questions que on peut avoir, a reçu le débat sur la question européenne. J'y reviendrai, mais sur la question de l'OTAN. Je crois que c'est un manque. Monsieur le Ministre, dans nos débats. Il n'est pas possible parce que c'est un texte de loi, il aurait été possible si nous avions une vraie hein devrait Livre blanc sur la question européenne. Je crois qu'il faut aussi l'assumer. Il ne faut pas il faut une politique urbaine des forces beaucoup plus importante. Là aussi, cette impression. Ce texte sur les questions de recherche développement. Sur les questions notamment de commande commune ou de projets communs d'armements et je crois que là-dessus il faut porter les choses pour ne pas être trop long, je vous dire un mot également sur contrôle parlementaire. Beaucoup de choses. Oui, nous avons souhaité renforcer cela avec la Commission, nous avons travaillé parfaitement avec le président Cambon et l'ensemble des commissaires et je les remercie de ceux-là c'est vrai contrôle parlementaire nous est important pour nous. Alors c'est vrai que nous avons fait adopter un amendement notamment sur la question d'un nouveau livre blanc.

Alors. Parce que le temps maintenant on peut et s'est réduit pour terminer mais on aura l'occasion de débattre encore dans, dans nos débats. Vous dire que la position des socialistes. Pour notre groupe, on l'a dit depuis le début, la question c'est de bonifier la LPM. Et je crois je parle sous contrôle du président Cambon que par nos amendements en commission, nous avons su bonifier ce texte. L'article premier, beaucoup d'autres textes, je vous le dis sur ensemble de questions sur hé on reviendra dessus sur le SNU sur la question du contrôle, j'ai envie de l'armement survient des la question aussi la question sociale pour pour pour les militaires. Vous voyez que nous avons et seulement progressé et et et et aussi sur la question de la puissance d'équilibre ou. Ou la question d'influence voilà beaucoup d'éléments sur lequel nous avons fait progresser ce texte nous souhaitons nous l'avons lu ce matin à l'interview dans Le Figaro. Monsieur le Ministre, oui, nous avons fait beaucoup d'amendements et ce n'est pas parce que nous n'avons pas. C'était pas décider comme cela, c'est parce que nous souhaitons qu'on qu'on sera avec vous. La question la défense nationale parce que il y aura une nouvelle majorité en 2027. Espérons en être pour pouvoir avoir aussi d'autres visions sur la question militaire, mais donc nous attendons maintenant beaucoup effectivement de la sagesse. Voir le soutien du gouvernement selon bon nombre d'amendements, vous verrez qu'ils ne font que bonifier cet axe-là et je crois que c'est la demande de l'ensemble des bancs du Sénat bonifiant ce texte là améliorons notre texte faisant en sorte que notre pays puisse avoir son armée à son niveau et que nos hommes et nos femmes qui la composent soient fiers de porter notre uniforme et porter nos couleurs, je vous remercie. Je vais appeler. Madame, Michelle Gréaume. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'enjeu de ce projet de loi définissant la trajectoire budgétaire de nos armées pour les 7 prochaines années est immense. Malheureusement cette loi fut décidé à la hâte 2 ans avant la fin de l'actuelle LPM et ne dispose d'aucune orientation stratégique précise juste celle d'une obligatoire, augmentation des dépenses militaires. Dans un contexte marqué par des logiques de puissance et parfois de remise en cause des principes du droit international. Le sujet dont traite ce projet de loi aurait dû associer bien plus largement la représentation nationale mais une fois de plus, elles furent décidées par un seul homme. Il est assis à côté de maintenir et moderniser nos 2 composantes de dissuasion nucléaire, sans que ses choix n'ait été préalablement réévalué. Outre l'opacité totale sur les programmes précis des 53 7 milliards consacrés aux armes à destruction massive soit 13% du budget de la LPM vous refuser tout débat sur la pertinence stratégique du match d'une telle stratégie de dissuasion. Moderniser de tels systèmes d'armes, c'est engager la France dans une stratégie pour des décennies qui pourrait devenir obsolètes en une. Monsieur le Ministre, ce pari est beaucoup trop lourd de conséquences pour être décidée sans concertation avec la représentation nationale ne balayez pas nos interrogations en faisant croire à nos concitoyens qu'en matière de dissuasion nucléaires nous serions face à un choix binaire entre le tout et de rien. Ce choix de la dissuasion pour assurer la sanctuarisation de notre territoire. Lui, un autre choix très discutable privilégier l'équipement de nos forces conventionnelles vers des stratégies de projection extérieure, il serait sans doute temps de cesser de voir la défense de notre pays partout ailleurs qu'en France ce modèle de projection au détriment de la défense de nos territoires a des implications stratégiques concrète et de lourds coûts budgétaires d'une part stratégique puisque malgré les éléments de langage creux du type la cohérence sur la masse, en réalité, ce que je vois ce sont des capacitaire qui perdure et une logique échantillonnaires qui reste reine. La place excessive accordée à la dissuasion nucléaire conduit à opérer des coupes claires dans nos défenses. Hors de quel conflit souhaitez-vous nous prémunir avec 200 chars Leclerc. Lorsque l'on sait que la Russie, on a perdu plus de 2000 depuis son conflit en Ukraine. Quel territoire maritime sur les 11 millions de kilomètres carrés que compte la France pour nous surveiller ou défendre avec une dizaine de bâtiments de 1er rang. Le paradoxe, c'est que votre logique présente des coups au budgétaires colossaux. Par exemple nous allons dépenser plus de 10 milliards d'euros dans un porte-avions faire valoir depuis ce bâtiment ne sera en aucun cas utile en cas de guerre du fait de sa trop grande une vulnérabilité il mobilisera davantage son groupe aéronaval pour sa défense que pour celle de la nation vous justifié ce choix par le besoin de puissance et par celui de pérenniser la filière industrielle de nos chaudières nucléaires à usage militaire. D'autres choix sont possibles et à quoi sert de se doter aujourd'hui d'un nouvelle d'un nouveau porte-avions, si ce n'est caresser dans le sens du poil, l'imaginaire collectif du symbole de la souveraineté. En réalité, il s'agit de pouvoir intégrer une task force task force américaine et avoir l'illusion de la commander pendant quelques jours sous l'étroite tutelle d'un commandement américain. Alors oui, nombreux sont ceux qui pointent les pays qui qui ayant une ambition navals construisent des porte-avions mes chers collègues, en faire de même. Est-ce pour autant répondent avec pertinence et réalisme au défi de sécurité qui sont et seront les nôtres. Privé de réflexion stratégique souveraine. Vous ne faites que Mimi. Celle des autres, vous vous alignez sur une course mondiale à l'armement qui atteint les 2240 milliards de dollars l'année dernière non instruit manifestement de cette stratégie qui vise pour garantir son hégémonie a imprimé un rythme que les autres ne pourront pas suivre. Vous vous alignez sur les injonctions de l'OTAN de monter le budget de défense à 2% du PIB et tant pis si cet indicateur n'a aucune signification militaire pour la défense de notre nation puisque l'objectif absolu c'est de pouvoir se gargariser d'être l'élève modèle En réalité, ce déficit de visée stratégique menace directement notre sécurité et notre souveraineté. D'abord nous pensons que la défense de la patrie passe d'abord et avant tout par la promotion de la paix, une paix durable, une paix qui s'inscrivent en écho aux désastres des guerres. Or en s'alignant sur des intérêts qui ne sont ni les siens Nice participant à la sécurité humaine, la France se détourne de son engagement indéfectible pour la paix et le libre développement de tous les peuples 3ème réseau diplomatique au monde notre nation doit s'inscrire dans une visée stratégique global visant à prévenir les conflits a multiplié les accords multilatéraux de désarmement nucléaire et de démilitarisation des espaces communs. La revue nationale stratégique accrue la diplomatie dans le Champ de l'affluence. Hé bien Swat oeuvrons avec toutes les nations qui le souhaitent à travers l'ONU à travers des coopération. Viviers à lutter contres les insécurités global et notamment l'une des plus menaçante. La sécurité environnementale qui elle et nous en avons la certitude renouera des plans entiers de notre territoire et sera une catastrophe systémique pour l'humanité. Ensuite je voudrais évoquer les lacunes de la politique cyber qui témoignent des avancées stratégiques flagrante de cette LPM plusieurs types de lutte informatique saut assuré. Mais quid des couches intermédiaires du numérique dans la production des logiciels des systèmes d'exploitation. Quid de la production des matériels des routeurs au micro processeur ou même des infrastructures réseau. La commission de la Défense du Sénat des États-Unis avait déjà établi en 2012 que des millions de composants électroniques contrefaits ou compromis avait pénétré les systèmes d'armes de leur pays au regard des ruptures technologiques à l'oeuvre aujourd'hui qui ont tous pour pour base commune une hyper technologie Satio et par là même une demande croissante à la matière de composants électroniques. De se résigner à ne pas maîtriser souverainement les soucis de conception et de production du numérique c'est se résigner à perdre notre taux notre autonomie stratégique. Alors que le gouvernement s'apprête à faire 10 milliards d'euros du coup de rabot dans les crédits budgétaires cette loi en hausse de 40% par rapport à la précédente ne répond pas à l'unique objectif qui devrait préoccuper nos armées, celle de la stricte défense de nos territoires. nous continuerons à nous éparpiller dans toutes les régions du globe afin d'assouvir des intérêts étrangers à la France est contraire aux enjeux de sécurité globale qui préoccupe l'humanité pour toutes ces raisons, notre groupe votre raconte ce but. Ce projet de loi et à travers une quarantaine d'amendements, nous vous donnerons détailleront nos propositions afin d'exprimer clairement notre vision d'une France souveraine capable de se défendre et promouvant la paix merci. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Olivier Cigolotti pour l'Union centriste. Monsieur le président. Madame, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. 413 milliards c'est bien l'effort budgétaire que prévoit cette loi de programmation militaire pour la période 2024 2030. Depuis plusieurs décennies dans un contexte post-guerre froide bénéficiant des dividendes de la paix. Nos forces se sont vu imposer une érosion des moyens budgétaires et une diminution drastique des effectifs. Cette augmentation de la part du budget de la nation consacrée à nos armées est la bienvenue. Elle poursuit le mouvement engagé dès 2019 avec la précédente LPM qui avait déjà pour objectif de porter la part des dépenses militaires à 2% du PIB en 2025 et de créer 6000 emplois. Cette trajectoire budgétaire de croissance visait déjà à régénérer le capital opérationnel des armées pour constituer une première étape vers un modèle d'armée complet et équilibré. En février 2022. L'agression de l'Ukraine par la Russie a constitué un glissement stratégique. La guerre était de retour sur le flanc oriental de l'Europe et il apparaissait nécessaire de revoir notre ambition face à un regain de tension dans toutes les zones du monde. Ainsi les risques, les menaces sont plus importants que jamais et pourrait aller jusqu'à un engagement de très haute intensité. Les travaux de cette nouvelle loi de programmation militaire ont été engagés depuis de nombreux mois et malheureusement, l'exécutif a préféré faire l'économie d'un livre blanc au profit d'une revue nationale stratégique à laquelle les parlementaires n'ont été que peu pour ne pas dire pas associé. Ce que nous regrettons. Cette revue nationale stratégique se limite malheureusement à un inventaire des défis sécuritaires futur sans les hiérarchiser, alors que nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe, marquée par de nouveaux c'est. Passe de conflictualité mais aussi par la persistance de certains réflexes comparables à ceux des derniers conflits mondiaux. Nous nous sommes étonnés en commission de constater que, malgré une hausse. Considérable du budget des armées octroyée par cette loi de programmation militaire certains objectifs. Sont bien plus étalés qu'initialement prévu. Et nous regrettons également certain certains décalage de programme et même parfois des révisions à la baisse. Nous nous félicitons cependant des avancées majeures désormais introduit dans ce texte et des crédits fléchés. Sur des programmes à effet majeur comme sur des cibles ô combien importante. Nous nous réjouissons bien évidemment de langage. Du programme dédié au porte-. Avions de nouvelle génération qui constituera un élément de crédibilité de souveraineté et des 5 milliards d'ores et déjà fléchés dans cette LPM. Même si l'inflation hein. Il y aura cette trajectoire budgétaire. Nous ne pouvons que saluer les efforts réalisés pour nos services de renseignement et la lutte contre l'ingérence pour nos forces spéciales afin de leur permettre d'améliorer encore leur capacité leur polyvalence pour notre capacité de dissuasion, aérienne ou océanique qui bénéficieront également de crédits de modernisation pour la consolidation du socle d'entraînement grâce. Nos capacités de simulation. Pour l'effort en faveur des munitions qui permettra aux armées de consolider, de recompléter les stocks de munitions pour favoriser également une transition nécessaire vers les futures capacités feu dans la profondeur ou encore munitions télé-opérées. Pour les crédits accordés à l'innovation, oh combien vitaux pour affirmer supériorité technologique et garantir la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité enfin pour notre modèle RH et pour l'attention portée à nos services de soutien. Dans ce contexte, notre groupe soutient le lissage et la consolidation de la trajectoire budgétaire ainsi que les amendements venant sécuriser le budget du ministère. a également répondu à un appel des industriels de la défense et de leurs prestataires rencontrant encore souvent et trop souvent des difficultés de financement en créant le livret souveraineté. En tant que rapporteur pour avis du programme 178 lors de l'examen du budget. Je ne peux m'empêcher d'évoquer quelques points. L'effort consenti en faveur des crédits de paiement dans le cadre de cette LPM est conséquent. 3 chiffre marque une progression très nette. 69 milliards d'euros bénéficieront à l'entraînement et à l'activité des forces, soit un effort supplémentaire par rapport à la précédente LPM de 20 milliards. 49 milliards sont alloués à l'entretien programmé du matériel, soit 14 milliards de plus et enfin 18 milliards pour les services de soutien, ce sont 4 milliards supplémentaires. Les forêts là il était indispensable tant le programme 178 et dit mentionnant pour répondre à l'hypothèse d'engranger d'engagement majeur comme à la haute intensité. Mais les résultats en matière de préparation opérationnelle et de disponibilité technique représente de fortes préoccupations pour notre commission en 2023, les indicateurs en la matière. Sont parfois particulièrement décevant. La situation s'est dégradée. Sans que nous n'ayons aucune visibilité sur le décrochage qui s'est opéré pendant les 4 premières années de la LPM faute d'application de l'article 7 qui devait fixer des objectifs annuels dans ces domaines. Nous nous assurerons également que les indicateurs de l'armée de terre qui n'atteignent aujourd'hui que 70% de la norme l'entraînement ne soit pas sous-estimer. La consommation de ces crédits ne devra pas donc être repoussée à la deuxième moitié ou au dernier tiers de cette LPM et nous ne pouvons pas accepter cette fois encore, de ne pas avoir les jalons tout au long de l'exécution d'LPM nous aurons très certainement le débat en séance. Nous devons collectivement. Veuillez au capital technique de nos armées. Nous ne pouvons pas comme certains de nos alliés, nous retrouver avec une armée qui présente bien mais qui s'effrite lors d'un examen détaillé. Le groupe Union centriste portera avec conviction plusieurs amendements sur le service de santé des armées, afin que le ministère des Armées s'engage à préserver leur savoir-faire parfois unique au monde, ou sur les grands fonds marins qui constituent un nouvel espace de conflictualité. Il y a un an, le Sénat a rendu un rapport sur cette problématique des grands fonds marins où il indiquait qu'à ce jour-là. Marine ne disposait d'aucun équipement propre capable d'atteindre 6000 mètres de profondeur. Il est nécessaire que l'objet. Type d'acquisition d'équipements spécifiques pour mieux connaître surveiller et agir jusqu'à des profondeurs importantes soient poursuivis et atteint cela permettrait de couvrir près de 97% des fonds marins du globe. Pour la France dans la superficie maritime représente 17 fois la superficie terrestre grâce à ses outre-mer. Il s'agit de préserver son rôle historique de grande puissance militaire et scientifique au niveau mondial. Nous avons également déposé de nombreux amendements sur l'importance de la filière stratégique des drone enfin nous soutiendrons les amendements visant à consolider notre BITD. Mon collègue Philippe Folliot insistera pour sa part dans quelques instants sur tous les enjeux liés à nos outre-mer et porté par le groupe Union centriste. Enfin pour conclure, j'aimerais avoir une pensée pour les soldats tombés pour notre drapeau ou qui ont été blessés sur les différents théâtres d'opérations. Extérieures, et particulièrement pour les 58 soldats qui ont perdu la vie durant l'opération Barkhane. Monsieur le Ministre durant l'examen de ce texte structurant pour nos forces, nous avons le devoir ensemble de déterminer le modèle d'armée que nous souhaitons pour faire face aux enjeux de souveraineté auxquels la France doit répondre à l'heure où les compétiteurs et les États puissance ne cachent plus leurs ambitions. Merci cher collègue. La parole est à présent à monsieur Jean-Noël Guérini pour le Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues permettez-moi tout d'abord de dresser un constat qui sonne comme un regret. Monsieur le Ministre. Il a fallu attendre le retour de la guerre sur le sol européen aux portes de l'Union pour réaliser surtout. Assumer officiellement que l'outil de défense dont nous disposons est a minima, adaptés aux seul temps de paix. Pourtant déjà avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons connu de sérieuses alertes en 2021. 2 exercices interarmées de simulation de conflits internationaux. Organisés avec les Américains et des Britanniques avaient permis de constater les limites capacitaires des forces françaises. La commission de la défense nationale des forces armées avait alors appelé en février 2002 je la cite.

Il est manifeste que l'aviation de chasse française pourrait être réduite à néant un séjour. À qui la faute, me direz-vous. Avant le à tout le monde et à personne à la fois ne voyait pas en cette formule. Une manière d'excuser une responsabilité à la noyant dans une MP Roesti collective. Nous avons tous autant que nous sommes pêcher par naïveté, persuadé que la construction européenne suffirait à nous préserver. Bercer par cette douce illusion de paix la nation a laissé filer le budget de la défense le réduisant en variable d'ajustement. Pourtant, selon les derniers classements publiés en mai dernier, la France dispose de la 9ème armée au monde et la première dans dans l'Union. Quel paradoxe. Après et vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre une LPM 2019 2024 à hauteur de 295 milliards qui entendaient combler les retards dans tous les domaines. Des équipements en passant par la préparation opérationnelle le renseignement ou encore la condition de la vie militaire, le temps des vaches maigres semble révolue néanmoins. Si nous nous accordons tous à dire que l'enveloppe de 413 milliards d'euros à partir de 2024 sur 7 ans et substantielle des incertitudes demeurent sur sa soutenabilité comme l'a rappelé notre président de la commission. Ainsi. L'étalement des cibles de matériel et la question de l'inflation. Dont le coût serait d'ores et déjà estimée à 30 milliards d'euros incite à la prudence mais félicitons-nous d'avoir en commission réorganiser la variation des crédits dans le temps sans pour autant modifier le budget global. Ils progresseront de façon rythmée et régulière de 47 milliards d'euros en 2024 pour atteindre 69 milliards en 2030. Avec ce montant prêcher hein ten la nation doit pouvoir garantir la crédibilité dans la durée de notre dissuasion nucléaire transformer nos armées, aux fins de conforter notre supériorité opérationnelle renforcer la cohérence, la préparation et la réactivité de nos forces armées Poursuivre l'attractivité et la fidélisation des militaires c'est des civils. Je ne vais pas détailler les différentes enveloppes dit les nombreuses dispositions qu'elle soient relatives aux autres avec la mise en place de la solidarité interministérielle où les garde-fous entourant le service national universel mais je me félicite qu'au-delà de la prévision de 136 milliards d'euros pour la préparation de l'emploi des forces l'entretien programmé du matériel et des soutiens. Les services de renseignement du 1er cercle bénéficieront de CM 4 milliards d'euros. De même que 15 milliards d'euros seront sont consacrés uniquement à l'innovation et à. Et à la rue nisation des forces. Nos forces armées, quant à elles bénéficieront de cibles de matériel de nous pourrions élevé l'influence au rang de fonction stratégique. L'effort est notable. Pour la marine nationale avec les commandes de sept patrouilleurs de haute mer et trois ensemble de chasseurs aux mines et la perspective d'un porte-. Avions de nouvelle génération, à l'horizon 2037, de même problème. L'armée de l'air avec 137 Rafale d'ici 2030. J'espère que les engagements seront tenus sur les dates et l'achat de 6. Système d'drone tout comme l'armée de terre qui renforce de 2 milliards son budget munitions il est apparu nécessaire de créer un régime d'apprentissage militaire et de promouvoir le lien nation-armée pour atteindre des objectifs. Quant à l'acide de réserve fixé au plus tard en 2035 et c'est aussi dans le cas de la promotion de lien de ce lien fort nation-armée que la commission a créé un livret d'épargne souveraineté destiné au financement de l'industrie de défense en complément de l'effort budgétaire en tant que représentant de la nation. Nous nous félicitons des dispositions qui permettront de sacraliser le rôle du Parlement. À cet égard la Commission a renforcé là les garanties de l'actualisation dans étang et par un vote. Quoi de plus logique la LPM n'est pas seulement un test égrenant une farandole de chiffres dont l'accumulation peut rendre perplexe le commun des mortels. Elle appelle des ajustements, des évolutions qui ne peuvent être l'otage d'orientation budgétaire, il appartient à la représentation nationale de veiller au respect des engagements. Pris pour la défense ensemble. Mes chers collègues, nous devons la construire la consolider et donc la défendre C'est donc avec bienveillance, que le groupe RDSE abordera l'examen de ce test. Je vous remercie. Merci cher collègue. Et je donne la parole à Monsieur Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Le 24 février 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a brutalement refermé la parenthèse géopolitique ouverte il y a 30 ans avec la chute de l'URSS et la fin de la Guerre froide. Balayant les dernières illusions hérité de cette période de confort stratégique. L'agression de Moscou a forcé les Européens à sortir de l'indolence et à regarder en face la nouvelle ère dans laquelle ils sont entrés. Une aire placé sous le signe de l'incertitude de la polarisation et de la confrontation. Une aire où les mouvements tectoniques, de l'ordre international qui agissait jusqu'à présent à bas bruit apparaissent désormais en pleine lumière. Veille des impérialismes affirmations des puissances régionales multilatéralisme en délitement recours au fait accompli et à la force. Diversification des menaces. Contestation de l'influence occidentale. La guerre en Ukraine fait partie de ces événements historiques qui éclaire la bascule du monde autant qu'il accélère. Face à ce séisme géopolitique dont nous avons encore ce week-end ressenti une réplique la sécurité de notre continent et de notre pays n'apparaît plus comme une évidence, mais comme un bien à protéger. Cette réalité nous amène aujourd'hui à examiner ce projet de loi de programmation militaire. Pour la France comme d'ailleurs pour les autres États d'Europe. Le constat est implacable, après 30 ans de désinvestissement massif dans leur outil de défense c'est largement démunie pour ne pas dire désarmer qu'ils abordent le nouveau paradigme stratégique qui s'imposent à eux. Depuis plus d'un an, tous ou presque ont affirmé leur volonté de renforcer leur budget militaire. Avec 400 milliards, plus 13, 3 milliards d'euros reprogrammer pour les 7 prochaines années. La France s'inscrit pleinement dans ce mouvement global de réinvestissement. Nous vous donnons acte monsieur le Ministre, et vous vous êtes battu pour ça. L'enveloppe est conséquente et ce d'autant qu'elle intervient à la suite de réels efforts financiers entrepris depuis 2019 pour restaurer le potentiel militaire de notre pays pour autant. Sera-t-elle suffisante pour permettre à nos armées, de se hisser rapidement au niveau des enjeux et des défis posés par la guerre à l'Est de l'Europe. Sans doute pas. Et c'est bien là le grand paradoxe de la LPM que vous nous proposez aujourd'hui un paradoxe entre des crédits qui augmentent fortement et des dotations en équipement majeur qui ne progresse pas. Pour certains programmes. La situation va même se dégrader puisque les cibles fixées hier pour 2030 ne seront finalement atteinte qu'à l'horizon 2035. Nous devons cette vérité aux Français qui financeront l'effort de défense de la nation. Ce n'est pas tant une affaire de nombre de véhicules parqués dans les hangars. Monsieur le Ministre, que de remplacement de nos matériels consommer ou envoyer à nos alliés. Il n'y aura pas davantage d'hommes et de femmes sous les drapeaux. Le format des armées restera lui aussi identique à celui qui est visé à la porte de la programmation militaire en cours. Pour compenser cette atonie du. Le gouvernement table sur une augmentation spectaculaire des effectifs de la réserve opérationnelle qui serait doublé en 7 ans et nous souscrivons bien entendu à cet objectif. Mais suivant en cela l'analyse du Conseil d'État, il me semble bien difficile de ne pas être sceptique quant à sa réalisation. Et pour cause. La lecture de la LPM ne nous permet pas de comprendre comment le gouvernement entend financer cette montée en puissance, ni comment il compte former, équiper et employer les les réservistes supplémentaires. Naturellement ce projet de loi de programmation militaire préserve à horizon 2030 des acquis fondamentaux auxquels nous adhérons en particulier notre modèle d'armée complet. Restera complet évidemment est capable d'agir dans quasiment tous les domaines, il demeurera sous-tendu par une dissuasion nucléaire indépendante renouvelée et modernisée. Malgré, là encore, nous devons tenir un langage de vérité. Malgré leurs qualités unanimement reconnues. Malgré les efforts portés sur leur cohérence nous armée resteront y compris au sein d'une coalition sous-dimensionné pour faire face à l'exigence d'un engagement majeur nécessairement long et coûteux en vies et en matériel. Bien sûr nous comprenons qu'il ne soit pas possible d'effacer en quelques années, des décennies de désarmement. Nous comprenons que tous ne puissent pas être financé, a fortiori dans un dans une période où l'inflation fait peser des incertitudes budgétaires inédites. Permettez-moi, à ce titre de souligner à quel point l'estimation retenue par le gouvernement, environ 30 milliards d'euros sur la période me semble optimiste. Les coûts des grands équipements militaires n'évoluent pas de la même manière que le panier de la ménagère. C'est près du double, soit, au bas mot, l'équivalent d'une année de programmation qui pourrait au final être effacées par l'érosion monétaire. Nous comprenons enfin qu'une LPM soit contrainte de faire des choix. Mais précisément, ce que nous ne comprenons moins c'est l'absence de choix stratégiques fort sur l'orientation de notre modèle d'armée sur les segments à privilégier. Face aux menaces les plus prégnante. Le texte qui nous est soumis donne davantage l'impression de proroger l'existant jusqu'à la prochaine élection présidentielle que de prendre acte des immenses bouleversements stratégiques à devenu ces derniers mois. C'est me semble-t-il, l'une des grandes occasions manquées de la LPM. Ce que nous comprenons moins ensuite, c'est le choix d'affecter au financement de nos armées certaines ressources femmes frappées d'une si grande incertitude. Monsieur le Ministre, la fable de la vente des fréquences hertziennes est encore dans toutes les mémoires. Vous comprendrez donc après avoir pris connaissance de l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Le parlement fasse preuve d'une certaine méfiance sur le sujet. Nous vous proposerons donc sans alourdir la dette et en respectant le budget défini par le président de la République de sanctuariser véritablement ces 413 3 milliards d'euros et rien que ces 413,3 milliards d'euros sur lesquels vous avez tant communiquer. Ce que nous comprenons moins enfin c'est le choix de précipiter l'élaboration d'une nouvelle LPM, tout en conservant pour les premières années des efforts budgétaires identique à ce qui avait été décidé avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire 3 milliards d'euros par an. Car le texte qui nous est soumis en somme laisse au prochain président de la République le soin d'accélérer la cadence, alors que c'est maintenant que la guerre fait rage en Europe. que nos armées doivent remonter en puissance. Maintenant que nos industriels ont besoin de visibilité et donc de commandes pour donner un tant soit peu corps à la notion d'économie de guerre si cher au président de la République. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous entrerons dans la discussion de ce texte avant tout animé d'un esprit de responsabilité. Tant vis-à-vis de nos concitoyens que vis-à-vis de nos soldats de nos marins et de nos aviateurs. Qui acceptent de faire de leur vie. Notre ultime rempart face aux menaces. Nous n'avons donc pas l'intention d'ajouter des milliards aux milliards. Nous sommes trop conscient de la situation financière déplorable de notre pays pour nous permettre une quelconque désinvolture en la matière. Notre commission conduite par notre excellent président et rapporteur Christian Cambon défendra néanmoins quelques idées simples. D'une part, ne pas laisser subsister le moindre doute sur le fait que les ressources, les ressources promises à nos armées seront bel et bien au rendez-vous. D'autre part, veiller à ce que le rythme auquel elles seront mises à leur disposition soit crédible et surtout compatible avec l'évolution des dangers qui pèsent sur la France et l'Europe. Je ne sais pas si une courbe budgétaire permet de protéger notre nation. Monsieur le Ministre, mais devant les menaces. Nous ne croyons pas à la stratégie d'une défense en pente douce. Car en définitive cette courbe défini tout le reste, à commencer par la crédibilité la sincérité et l'efficacité de la programmation à venir, je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent Joël Guerriau pour le groupe les indépendants République et Territoires.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Seul pays de l'Union à disposer d'un modèle d'armée complet. La France est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre les groupes terroristes, que ce soit en Afrique au le vent ou en Asie centrale. Jusqu'au coeur de nos partenaires, nous connaissons le prix de la souveraineté et celui du sang. Je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont donné de leur vie pour la France à ceux qui ont été blessés ainsi qu'à l'ensemble de nos forces. Leur engagement et leur professionnalisme nous permettre d'être libre. La guerre est de retour sur notre continent autant que nous le pouvons, nous devons continuer à de soutenir l'Ukraine qui se bat pour survivre, pour l'Europe et pour la liberté. Ce soutien ne doit cependant pas obérer la montée en puissance de nos capacités. La commission sous la conduite notre président a veillé à maintenir ce chemin de crête. Il était trois mais il est incontournable jusqu'en 2030. Les besoins de nos armées s'élève à plus de 400 milliards d'euros. La Commission a fait le choix de laisser davantage l'augmentation du budget de la défense afin de crédibiliser cette hausse. Un fonds européens destinés à l'industrie de la recherche dans le domaine militaire a vu le jour, d'un montant de 7 milliards d'euros pour la période 2021 2027. Ce fonds européens. La prise de conscience unanime de la nécessité d'agir solidairement pour la défense de notre continent, nous devons pouvoir faire face au réarmement qui est non seulement français mais aussi européen et international. Nous aux entreprises doivent être à la hauteur de ces enjeux et prête à répondre à la demande. Dans mon département ça là va des petites entreprises. Comme par exemple M2 à Ancenis, une très des très rares entreprises spécialisées dans les emballages d'obus qui fait face actuellement à une demande exponentielle en raison de la guerre en Ukraine. C'est un chiffre absolument faramineux qui est la demande qui leur a été faite, ce qui montre la gravité de la situation aux grandes entreprises comme Naval Group que les chantiers de l'Atlantique qui seront chargés de construire d'ici 2038 un porte-avions à Saint-Nazaire pour un budget supérieur à 5 milliards d'euros. À sujet j'attire votre attention. Monsieur le Ministre, un véritable défi doit être relevé une part significative des travaux à Saint-Nazaire et réalisé par des sous-traitants étrangers pour un court salariales moins élevées. Ce qui bien sûr nous interpelle. Nous devons d'ores et déjà à former du personnel qualifié, capable d'assumer la construction du futur porte-avions. L'État doit être au rendez-vous sur le plan éducatif, sur le plan de la formation professionnelle mais également pour accompagner les petites et les moyennes entreprises, qui devront investir pour absorber une demande la visibilité pour les programmes à venir est essentiel pour ces entreprises. Si nous voulons des acteurs français capable de répondre à des besoins complexes et variées en matière de défense, leur contribution à la sécurité nationale, européenne et internationale est un est inestimable. Notre engagement, de la défense et la sécurité non seulement un impératif stratégique, mais c'est aussi une opportunité de renforcer notre industrie de créer des emplois et de stimuler l'innovation. Nos entreprises sont un atout pour l'économie de nos territoires. Elle constitue une source d'expertise technologique de 1er plan mais également de développement qui contribue non seulement à notre sécurité, mais aussi à notre prospérité. La dissuasion nucléaire doit rester la clé de voûte de notre stratégie de défense. Il nous faut absolument préserver cet héritage du général De Gaulle qui a permis à la France d'être libre pour demeurer crédible. Nous devons veiller à l'entretien au développement de nos vecteurs ceux-ci présente bien sûr un coup il est très élevé ce mais c'est c'est aussi celui de notre liberté. Il est donc pas négociable. Nos forces conventionnelles doivent également être préparés à être engagés dans des conflits de haute intensité. Contrairement à Poutine. Nous ne voulions pas, nous ne voulons pas que ne soient que nos soldats ne soit que de la Chair à canon. Ce n'est pas notre conception nous les considérons comme des techniciens très efficace qui doivent pouvoir servir en bénéficiant la LPM prévoit donc pour les années à venir. Une montée en gamme. La France s'apprête à moderniser ses équipements en privilégiant la qualité. Sur la quantité. Les dernières technologies sont certes plus onéreuse mais elle permet une précision et une discrétion qui peut faire la différence. Aujourd'hui comme hier, la patrie a besoin de femmes et d'hommes pour la défendre. Les effectifs de nos armées devront être porté à 275.000 ETP en 2030 pour les appuyer, mais aussi pour faire vivre le lien armée-nation. La laine, la LPM prévoit d'accroître le nombre de réservistes à 80.000 à à l'horizon 2030 et nous approuvons cette orientation afin de parvenir à nos objectifs, nous avons également besoin de renforcer notre base industrielle et technologique de défense que j'évoquais tout à l'heure le texte simplifie la passation de marchés et adapte les enquêtes de coups. Plusieurs dispositions également pour objet de permettre à la France de disposer de matériel nécessaire à une confrontation la création d'un livret d'épargne souveraineté est à cet égard pertinente. Mes chers collègues. L'invasion de l'Ukraine par la Russie marque le début d'une nouvelle ère d'autres conflit de haute intensité pourrait éclater à l'avenir impliquant la France ou ses alliés. La guerre est est toujours une tragédie. Il est de notre devoir de préparer au mieux notre pays à cette triste éventualité. Clémenceau disait qu'il faut savoir ce que l'on veut quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire et quand tu le dis, il faut avoir le courage de le faire, nous avons dit ce que nous voulons, à nous d'avoir le courage de le faire. Merci. Mes chers collègues. Merci, cher collègue, la parole est ensuite au président Guillaume Gontard, pour le groupe écologiste solidarité et territoires.

Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Je voudrais d'abord. Souligner l'engagement des femmes et des hommes au sein de notre armée et souvent au péril de leur vie. Nous examinons cette loi de programmation militaire dans le contexte que chacun connaît et après le nouveau rebondissement de ce week-end, permettez-moi en préambule de rappeler notre plein et entier soutien au peuple ukrainien et à ses dirigeants dans la reconquête de leur souveraineté. L'invasion russe en Ukraine a justifié aux yeux du gouvernement à la nécessité d'accélérer le processus d'élaboration d'élaboration et d'adoption de la présente loi de programmation militaire. Les termes économie de guerre, ce sont même invités hâtivement dans le propos présidentiel. Monsieur le Ministre, malgré vos explications répéter. Nous ne comprenons pas l'urgence qui guide le gouvernement. Nous ne voyons pas de rupture telle avec les deux dernières LPM que justifieraient pourtant la nouvelle donne géostratégique européenne et mondiale. Nous voyons une la LPM dans la continuité des deux précédentes mais élaboré avec un déficit de concertation parlementaire et démocratique. Cela est dommageable. Car vous demander un effort important à la nation, avec une augmentation du budget des armées de près de 50% d'ici à 2030 et un effort global de plus de 118 milliards d'euros sur le reste de la décennie 17 milliards par an en moyenne 100 financement spécifique. Vous étiez plus regardants pour trouver 13 milliards pour nos caisses de retraite, quitte à mettre le pays dans un état d'extrême tension et piétiner la démocratie parlementaire. Votre gouvernement, enfermé dans son dogmatisme refuse de faire contribuer les plus aisés à l'effort national et promet un retour du déficit public sous les 3% d'ici la fin du quinquennat. Comment dans ces conditions, allez vous financer cette les cette LPM vos prévisions de croissance sont à l'heure ce débat nécessite que nous connaissions les perdants. Ça ne sera pas à l'intérieur et la justice désormais dotés de leur propre programmation budgétaire alors qu'il la transition écologique, l'éducation nationale, la culture aucun et aucune de ces solutions n'est acceptable. Et c'est pour nous une ligne rouge. Si nous comprenons l'effort de rattrapage budgétaire du ministère si nous avons bien en tête que cette crédit correspondent souvent au au paiement de programmes déjà engagés. Si nous n'ignorons pas l'explosion du coût des matériels qu'induit le saut technologique et les nouveaux espaces de conflictualité. Il n'en reste pas moins que vous demandez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas défini l'urgence de la menace et le besoin pour la France d'y faire face seul ou presque. À vous entendre et c'est aussi une faiblesse de cette LPM. On a parfois le sentiment que la France est seule, seule au monde qu'elle doit être en capacité de faire face à une guerre de haute intensité sur son sol et sans aide de ses voisins. Or ce que ce nouveau contexte géostratégique nous rappelle c'est l'immense dépendance des Européens aux États-Unis pour assurer la sécurité de notre continent. Malgré cette froide réalité. La France et ce projet en est l'illustration cultive son rêve d'autonomie et de puissance d'équilibre. Nous ne partageons pas ce récit. La France est une puissance Blin plus moyenne qu'elle veut le croire et continuer à promouvoir un modèle d'armée complète c'est prendre le risque du saupoudrage de l'échantillonnage et cette LPM n'échappe pas à ce constat, chacun en conviendra. Résultat des courses pour renouveler la dissuasion nucléaire au coût exorbitant pour dégager des marges pour investir de nouveaux espaces de conflictualité nous n'investissons pas comme nous le devrions pour notre armée de terre pour son équipement et pour le confort de vie des soldats et de leurs familles. Cette fameuse armée à hauteur d'homme, cher à votre prédécesseur. Les écologistes, pour leur part, considère que notre effort ne peut être qu'européen. Nos besoins en hommes en équipement en stock stratégique en munitions ne peuvent se mesurer que dans le cadre d'une coalition européenne la revue nationale stratégique était d'une grande faiblesse en la matière et le rapport annexé de la présente LPM améliorée par l'Assemblée nationale et le Sénat demeure insuffisant quelle coordination de notre effort avec ceux de nos voisins et notamment avec l'effort sans précédent opérer outre-Rhin quelle impulsion pour une base industrielle et technologique de défense résolument européenne, une nécessité, tant pour harmoniser nos équipements que pour diminuer nos coûts de production. Quels nouveaux efforts pour construire politiquement la réponse européenne au défi stratégique du XXIe siècles dont la guerre en Ukraine vient de nouveau rappeler l'absolue nécessité cet effort peut-il à court et moyen terme raisonnablement s'inscrire en dehors du cadre otaniens sur toutes ces questions la LPM et soit muette soit vague soit ambiguë. Il est certain que pour renforcer la dimension européenne de notre effort militaire. Il faudrait commencer par respecter les règles communes de l'Union et je pense en 1er chef au code de conduite sur les exportations d'armes de 1998 qui sans l'opposition de la France en particulier, pourrait devenir juridiquement contraignant. Monsieur le Ministre, la création d'une délégation parlementaire au contrôle des exportations d'armes ou l'extension en ce sens les prérogatives de la délégation au rationnement adopté en commission est un impératif. J'en profite au passage pour saluer les efforts de notre commission pour renforcer le contrôle parlementaire sur tous les volets de l'action de l'exécutif en matière de défense, il faut mettre un terme à ce domaine réservé indigne d'une république démocratique. J'insiste pour conclure sur le renforcement des efforts de transition écologique et énergétique de l'armée qui reste à ce stade, largement incantatoires. Je pense en 1er chef à la rénovation du bâti. Bien sûr la solution nos armées est à part. Mais en tant que 1er poste ministériel en termes de consommation d'énergies fossiles. Un effort tant écologique que financier doit être produit. Avec les 6 petites minutes qui mettait un parti ce propos est davantage un préambule qu'un tableau général et je profiterai bien évidemment des jours de débats qui s'ouvrent pour être plus complet. Merci. Merci cher président. Et à présent, la parole est à Nicole Duranton pour le groupe Rassemblement. Démocrates, progressistes et indépendants. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la Ministre, mes chers collègues. Avant d'entrer dans le vif de ce texte fondateur qui marquera notre politique de défense pour les prochaines années. J'aimerais m'adresser directement à nos soldats. Vous êtes des femmes et des hommes d'exception engagées en France et aux 4 coins du monde. Votre combativité est inégalable votre abnégation est un modèle pour tous. Je veux dire au nom de notre groupe RDPI combien nous sommes fiers de nos militaires. Combien nous vous en sommes reconnaissants. Je crois qu'au fond dans cet hémicycle, nous défendons un objectif commun. Celui de protéger notre population et notre souveraineté. Et celui d'accorder à nos armées les moyens d'atteindre cet objectif. Nous vision des choses et nos manières d'y arriver sont multiples mais jusqu'à présent nous avons toujours su avancer ensemble. Je forme le voeu que les débats de ces prochains jours se déroule sereinement et qu'il soit constructif. J'espère que nos discussions nous permettront d'y voir plus clair en particulier. Aux moyens budgétaires de cette programmation militaire. Si finalement il y a lieu d'augmenter l'enveloppe budgétaire. Nous en débattrons. Elle prévoit en effet des moyens financiers progressif est suffisamment conséquent pour permettre à notre armée de rattraper le retard d'investissement pris depuis 30 ans. Sans pour autant déséquilibrer le budget de la nation ou venir impacter d'autres postes de dépenses qui sont nécessaires aux Français. Si en revanche, il y a lieu de maintenir la même enveloppe globale. Ce débat sera l'occasion de comprendre où les coupes budgétaires doivent se faire pour compenser les nouvelles dépenses intégré. En ce qui concerne notre groupe, nous faisons le choix de faire confiance en notre État-Major et notre Ministre des Armées. État-Major avec qui cette loi de programmation militaire a été minutieusement pensé et élaboré. Nous faisons également le choix de ne pas rigidifier le travail de l'État-Major. De lui laisser l'attitude nécessaire pour s'adapter à tous les défis. Au cours de ces prochains jours notre groupe vous proposera plusieurs amendements sur des sujets qui nous tiennent à coeur. Par exemple pour compléter les missions de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre l'ONAC VG afin de le conforter dans son rôle de relais territorial de l'action mémorial du ministère. J'en profite pour saluer le travail incessant de madame la ministre en charge des anciens combattants et de la mémoire pleinement engagée aux côtés des anciens combattants et des blessés de guerre. Par exemple avec le remarquable plan blessés 2023 2027 présentée le 10 mai dernier. Ou encore un amendement pour stopper une inégalité de traitement entre étudiants en supprimant le paiement de droits d'inscription des élèves des lycées de défense qui viendraient à être exonérés de droits d'inscription sur des critères sociaux. Dès 2017, le président de la République a engagé une politique de rupture avec ses prédécesseurs afin de mettre un terme à plusieurs décennies de diminution de nos capacités militaires. Dans le cadre de cette loi de programmation militaire pour 2024 2030. Il est essentiel que la France continue de renforcer ses moyens garantir son autonomie stratégique assurer ses engagements en tant qu'alliés de l'OTAN et membres de l'Union européenne. Être une puissance d'équilibre. Avec cette nouvelle LPM on passe une première loi de réparation. 2019 2025 à une loi de transformation de nos capacités de défense pour être plus efficace et performant. Outre le renouvellement des capacités opérationnelles. Le ministère des Armées a entrepris un effort de modernisation. Cette modernisation participe de la réforme de l'État et vise notamment à dégager des marges de manoeuvre budgétaires pour adopter les capacités militaires notamment. Les équipements garantir les normes d'activité et d'entraînement et poursuivent l'amélioration de la condition du personnel civil et militaire. Le ministère des Armées travaille avec 10 grands groupes, 4000 PME et ETI et 200.000 personnes. Près de 27.000 entreprises sont partenaires du ministère des Armées. Mes chers collègues. Sur ces 413 milliards d'euros qui sont nécessaires pour garantir notre sécurité 268 milliards vont principalement profiter à nos industries soutenir l'emploi dans les territoires, préserver et développer les compétences. On sait que pour un million d'euros d'investissements. On génère sept emplois Directs et indirects. Aussi au cours des décennies, la France a fondé sa politique de défense et de sécurité entre autres sur la dissuasion nucléaire et la notion d'autonomie stratégique élaboré vis-à-vis de l'OTAN. Les menaces identifiées dans le livre blanc de 2008 se sont amplifiées terrorisme cybermenaces prolifération nucléaire pandémie. Dans un tel contexte, l'objectif d'une souveraineté maîtriser concernent les domaines critiques de la dissuasion. L'accès à l'espace, la capacité d'entrer en premier mais aussi le renseignement. La dégradation du contexte géostratégique a entraîné l'émergence d'une idée d'autonomie stratégique européenne et doit conduire à prendre en compte le retour de la notion de guerre à haute intensité comme en Ukraine. En effet, cette guerre a rappelé la nécessité de disposer de solides systèmes de défense antimissile et anti-aérien en cas de conflit avec une puissance étrangère 5 milliards sont programmés dans le rapport annexé sur la période pour la défense surface R le cyber 4 milliards les drônes et robots 5 milliards les stocks de munitions 16 milliards la fabrication d'un porte-avion nouvelle génération 10 milliards ces éléments figurent parmi les priorités stratégiques de développement pour les armées françaises. Cette programmation militaire ne se résume pas aux soldes d'investissements matériel elle comprend aussi un volet humain très important avec un doublement de la réserve opérationnelle et plus de 6400 créations de postes. Avec 700 nouveaux postes ouverts dès 2024 et 2025. Un objectif qui si il est réalisé dépasserait les augmentations de postes réalisées par la précédente LPM, selon les chiffres de la Cour des comptes. Cette programmation militaire comprend aussi un plan famille de 750 millions d'euros pour compenser les absences et les contraintes opérationnelles. Et une politique RH modernisé avec une gestion des carrières rénové. Dans l'indopacifique, face à une Chine qui ne cesse de multiplier cette démonstration de puissance cette programmation militaire permet à la France de tenir son rang, grâce à son armée et grâce à ses territoires d'outre-mer. Un effort particulier sera fait sur les infrastructures en outre-mer la part outre-mer de la LPM sera 13 milliards d'euros sur la période. Nos forces de souveraineté bénéficieront d'un effort généralisé sur le plan capacitaire Corvette avions de transport drone Jenny Dual et constitueront un premier échelon renforcer immédiatement disponible, afin de décourager toute tentative de stabilise de déstabilisation ou de prédation. Elles disposeront par ailleurs de capacités de surveillance qui amélioreront la couverture de nos territoires outre-mer et leurs zones économiques exclusives, les capacités de commandement seront durcis de manière ciblée en fonction des enjeux régionaux des réformes et une loi de programmation qui envoie le signal que la France peut compter sur une armée moderne et totalement connecté à son époque pour atteinte d'ici 2030, un modèle d'armée complet et équilibré apte à répondre à l'ensemble des menaces. Je vous remercie. Et la parole est à monsieur Philippe Folliot. Pour le groupe Union centriste. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la Commission. Mes chers collègues. Tous ces milliards que nous nous apprêtons à voter tous ses moyens. Tous ces matériels qui vont entrer dans le cadre de cette loi de programmation militaire ne serait rien sans celles et ceux qui les Serbes je voudrais rendre un hommage particulier à nos soldats, nos aviateurs nos marins. À l'ensemble des personnels des services de renseignement. Ceux qui s'occupe de cyber ceux qui s'occupe aussi de soutien. Les personnes les civils les ingénieurs. J'ai de l'armement en fait toutes celles et ceux. Réservistes compris qui contribuent à cet effort de défense. C'est un élément particulièrement. Important et essentiel. Monsieur le Ministre, c'est la 5ème. Loi de programmation militaire à laquelle j'assiste dans le cadre des débats parlementaires.

volonté donc de doubler le budget de notre défense et c'est un élément important et un élément est essentiel et est fondamental. Je voudrais. Dans ce cadre-là. Dire combien il est important aussi de ne pas rester focalisés sur des enjeux d'actualité ce qui se passe en Europe de l'Est est un élément important et essentiel et nous devons continuer à appuyer soutenir nos amis ukrainienne dans leur combat pour les valeurs pour la liberté pour leur souveraineté pour leur indépendance. Mais au-delà de ces éléments, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux particulièrement. Particulièrement important. Je voudrais en citer quelques-uns. Monsieur le Ministre. Cette loi de programmation militaire. Malheureusement pour moi à certains égards, elle manque d'audace. Si vous me permettez l'expression, nous sommes encore dans ce qu'on pourrait, ce que je me permettrai de qualifier de Global riquiqui, c'est-à-dire donc une posture globale, nous avons tous de la dissuasion jusqu'aux. Sur le terrain mais nous avons tous un très petit et il est dommage de ne pas avoir eu cette capacité à pouvoir prioriser un certain nombre de choses j'insisterai de, d'une part, la capacité de projection parce que ce qui fait la force de nos forces de nos armées, c'est cette capacité à pouvoir rentrer un théâtre et puis le 2ème point. Ce sont les forces de souveraineté. Les forces de souveraineté, c'est quelque chose d'important 15.000 effectifs il y a 30 ans, 8700. Il y a 10 ans, moins de 7000 aujourd'hui un enjeu, un enjeu important et majeur parce que. Oh de l'un, du fait, comme vous l'avez dit. De la nécessité de tenir compte des enjeux régionaux derrière cela se joue quelque chose qui est encore plus essentiel c'est la capacité de notre pays a donné de la crédibilité à sa stratégie à sa stratégie indopacifique. Alors certes nous sommes aussi protégé par l'article 5 de l'OTAN et nous sommes dans un système d'alliances je regrette du reste que l'article 42 7 de l'Union européenne ne revêt pas peut être une importance plus importante de pour nombre de d'autres. Acteurs mais il faut poursuivre les efforts de réarmement en vue de nos forces de de souveraineté il faut Monsieur le Ministre. Sortir de cette logique qui fait que sur les 26 base aérienne aucune de plein exercice aucune dans les Outre-mer. Il faut sortir de la logique des 2 moitiés, Brest, Toulon, pour aller pour notre Marine nationale vers une logique des 4 quarts, Brest, Toulon. Toulon. Saint-Denis de La Réunion Nouméa ou Papeete pour le le le Pacifique. Il faut sortir de cette logique d'avoir uniquement des régiments de tournant pour l'armée de terre à voir des des régiments prépositionnés pour avoir une capacité de projection à partir des outre-mer ce sont tous ces enjeux qu'il faut relever par rapport à tout cela. Un objectif, une ambition collective que nous devons avoir, nous défendrons un certain nombres d'amendements pour permettre, ceci pour essayer de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir cette lisibilité, cette stratégie qui fasse ce que la France finalement. Ne soit ne ne se considère pas telle qu'elle croit être c'est-à-dire continentale européenne mais qu'elle le agissent en fonction de ce qu'elle, elle est aussi au-delà du fait d'être continentale européenne c'est d'être mondiale et maritime. Je vous remercie. La parole est à présent hein monsieur Pascal Alizart pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président et rapporteur, chers collègues. La défense, c'est la première raison d'être de l'état, il n'y peut manquer sans se détruire lui-même. Telle était la conception du général De Gaulle. La loi de programmation militaire et donc déterminantes pour notre avenir dans le contexte actuel et en effet depuis la dernière. Le monde connaît un regain de tension inquiétant. L'Europe est confrontée à un conflit majeur causé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie Russie puissance dotée et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU de l'OSCE ceci en dit long sur l'état de l'ordre international nous redécouvrons à nos dépens que la paix ne va pas de soi. Combien de programmes militaires. De coupes budgétaires et de réduction d'effectifs ont été justifié en Europe par les dividendes de la paix. La France n'a pas échappé à cette tendance même si elle a su conserver avec peine un modèle complet d'armée et une BITD performante. Mais aujourd'hui un nouvel ordre mondial se mettent en place entre le camp occidental. Le reste du monde et le pôle eau russo-chinois. L'Europe pourrait se trouver cornérisé. Une Russie au pouvoir contesté par des mercenaires nationaliste cerné par l'OTAN est dépendante de la Chine est en fait une menace sérieuse pour la sécurité. Rien ne me paraît plus dangereux qu'un pays acculé au seuil de la guerre civile. Surtout lorsqu'il s'agit d'une puissance nucléaire aux multiples capacités militaires ces évolutions ne sont pas sans conséquences sur nos intérêts et en Afrique. La pression des compétiteurs stratégique ça trois y compris sur l'espace francophone. Leur stratégie de soft power s'déploie en même temps que d'autres moyens hybride. Ce sont là les outils du jeu des puissances auquel nous devons être préparés. L'opération Barkhane, à montrer le savoir-faire de nos armées mais aussi les limites du pôle du modèle expéditionnaire français grâce à leur capacité d'adaptation. Nos forces ont obtenu des succès incontestable au prix néanmoins d'une usure des personnels des matériels, mais aussi de pertes humaines notable. En indopacifique. Nos forces sont présentes, en particulier la marine et agissent avec nos alliés de la région face notamment à la Chine qui avance ses pions à marche forcée et avec habileté. Autour de nos outre-mer l'immensité des zones sous souveraineté française à surveiller à protéger restera un défi. Les drone et le traitement de masse des données par Intelligence artificielle ne pourront pas tous. Être et durer. Telle est la problématique posée aux chefs militaires. Qu'en sera-t-il demain dans la perspective d'un conflit complexe de haute intensité, mêlant tous les champs de la conflictualité et entraînant une forte attrition des moyens. Que ce rapide de l'exercice Orion 23 fermé Trade savoir où la France en est dans ce domaine et d'envisager des ajustements. Qu'en sera-t-il dans la perspective de conflit larvé, mais plus hybride. L'action combinée de quelques centaines de mercenaires Wagner sur le terrain africain et d'opérations de propagande désinformation a permis de prendre le contrôle de fait de certains États conduisant à l'éviction de la mission Barkhane. Les cyber attaques contre nos hôpitaux font aussi des dégâts dangereux et coûteux. Prenons-nous pleinement la mesure de la force de ces déstabilisation réalisé à moins de recours. Je n'en suis pas convaincu. Pour préserver la paix les capacités actuelles ne sont plus suffisantes. Il faut des moyens adaptés dimensionnées capable d'évoluer rapidement. Vous portez, Monsieur le Ministre cette LPM avec des ambitions fortes des moyens forts annoncés et aussi une certaine communication. Le sénat examine ce texte avec sérieux. Voulue par le président Cambon les différents groupes de travail ont conduit des dizaines d'auditions sur plusieurs moi c'est mon cas, avec mes collègues des groupes sur le renseignement et la prospective et sur le bilan de l'opération Barkhane. Les amendements adoptés en commission témoigne d'une volonté d'aider les armées sans esprit de polémique, il est souhaitable que leur contenu demeure dans le texte final. Je ne m'étendrai pas sur le montage financier de cette LPM. Nous faisons, vous faites des hypothèses notamment sur l'inflation. Vous tablez. Nous tablons sur des ressources additionnelles certaines plus incertaine que d'autres si je puis dire ainsi que sur des ajustements de dépenses au fil de l'eau. Avec le poids de la dette. Néanmoins les mauvaises surprises sont sans doute à venir. La défense, ce sont aussi des industries que seraient nos forces dans une BIT des fortes et indépendantes. La concurrence d'entreprises étrangères aux contraintes limitée et fortement soutenus par leurs États se durcit. Les financements sont cruciaux pour la survie d'un des derniers écosystèmes industriels français. Il s'agit d'une filière d'excellence non délocalisables qui représentent un vivier d'emplois dans les territoires. Malgré les efforts de l'État trop d'entreprises sont passées ces dernières années sous pavillon étranger, notamment pour y trouver les financements nécessaires à leur croissance. D'autres craignent de devoir être absorbé par de grands groupes d'y perdre leur liberté et leur capacité à innover. Quant aux grands groupes, ils redoutent eux la défaillance d'un de leurs fournisseurs critique. Les soutiens publics sont importants, les financements privés le sont tout autant. Il faut créer un environnement favorable pour les banques et les investisseurs. Le passage à une économie de guerre ne pourra pas se faire sans eux. Par ailleurs, un plus grand activisme français s'impose sur les projets de texte européens qui impacteront l'industrie de défense la veille ne suffit plus. Car derrière ces textes à vocation écologique et sociale. Il y a souvent des lobbies qui poursuivent en fait des politiques économiques contraires à nos intérêts. N'ajoutons pas des contraintes. Qui fausseraient ainsi encore un peu plus la concurrence aussi, j'ai fait adopter en commission de nombreux amendements pour conforter notre BITD, la pérennité de ces industries requiert une visibilité de commande, elle leur permet de pouvoir réaliser les investissements souvent lourds les stocks les machines-outils. Les robots de maintenir les compétences et de pouvoir embaucher pour répondre aux besoins des armées, en particulier dans le contexte économique guère les Stop and Go empêcheront de produire vite et mieux la continuité industrielle est indispensable car les capacités et les compétences. Ce père de vite mais se rattrape lentement. Le paradigme des coopérations européennes atteint aussi ses limites avec nos partenaires allemands. Enfin il y a est simple, ni sur le SCAF ni sur le MGCS. Il y a aussi beaucoup de vigilance à voir sur ces points. Alors Monsieur le Ministre. Avec la guerre en Ukraine, les autorités russes sont partis du postulat selon lequel les démocraties sont faibles, sont malades. Elles ont d'ailleurs tout fait pour les diviser et mieux les affaiblir face aux instincts belliqueux porté par la convergence des autoritarisme. Nous devons nous les démocraties afficher une détermination sans faille le droit et les valeurs sont des instruments nécessaires mais insuffisants pour défendre nos sociétés démocratiques. Donnons-nous ensemble réellement les moyens à la hauteur de nos ambitions et des menaces nouvelles, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'examen de la loi de programmation militaire par notre haute assemblée constitue toujours un de ces moments graves ces solennel où nous réalisons que ce qui se joue n'est ni plus ni moins que la sécurité de notre pays et de nos compatriotes et donc de leur avenir. C'est une lourde responsabilité qui nous incombe, alors dans ce monde où plus personne ne le niera désormais les enjeux de sécurité et de défense n'ont jamais été aussi cruciaux investit au sein de la commission Affaires étrangères défend ses forces armées du Sénat depuis mon entrée au Sénat en 2004, j'ai parfois eu l'impression que ces enjeux de défense et de sécurité n'avait pas toujours été prise en compte à leur juste valeur et je me réjouis donc d'autant plus que la prise de conscience collective, aussi bien dans l'opinion que par les décideurs publics de leur importance primordiale. À l'heure où l'Ukraine se bat avec un courage Il est indispensable d'afficher clairement dans cette LPM nos ambitions en matière de sécurité collective et notre ferme volonté de tenir notre rang en tant que première année armé de l'Union européenne et de maillon essentiel essentiel de l'OTAN. Cette alliance euro-Atlantique qui n'a jamais failli et qui est la meilleure garante aujourd'hui de notre sécurité de notre défense collective. L'enrichissement substantiel de ce texte que nous avons proposé en commission démontre une nouvelle fois la qualité du travail de notre assemblée et contribuera très très nettement à mettre cette LPM au niveau que nos armées à qui je veux rendre ici moi aussi un hommage appuyé, sont en droit d'attendre et à la mesure des engagements qui sont les nôtres vis-à-vis de nos concitoyens et de nos alliés et partenaires. L'adoption de cette LPM permettre ainsi à la France au sommet prochain de l'OTAN, les 11 et 12 juillet à Vilnius d'apparaître aussi crédible et fiable qu'elle se doit de l'être. Je rappellerai que les 274 membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN que j'ai l'honneur de présider, et dont je porterai la voix auprès des 31 chefs d'État et de gouvernement lors de ce sommet sommet de Vilnius. Appel à l'unanimité à renforcer le soutien politique et militaire à l'Ukraine et à renforcer notre politique de défense et de dissuasion en consacrant plus de moyens à l'accroissement à l'accroissement de nos capacités collectives. N'ayant que 5 minutes et arrivant en toute fin de discussion et ne voulons pas répéter tout ce qui a été dit et ex-et le excellemment dit par plusieurs de mes collègues je me contenterai de m'arrêter sur 2 autres sujets. Tout d'abord la désinformation. La guerre informationnelle qui est mené quotidiennement par la Russie notamment et d'une grande violence et ses conséquences pourraient être des plus désastreuse et destructif triste pour notre pays, nos sociétés, nos démocraties. Si nous ne la prenons pas collectivement on compte mettant moi même penché sur cette nouvelle forme de guerre dans un rapport que j'ai présenté à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je voudrais insister sur la nécessité de se préparer, de se former et donc de s'armer et ce dès le plus jeune âge comme se lâcher dans plusieurs États scandinaves. Face à ces attaques qui visent à saper les fondements même de nos sociétés démocratiques. Ensuite découlant de ces nouvelles mesures. Il me semble tout aussi essentiel de développer nos outils d'influence et de rang mais le lien armée nation et ce tout particulièrement auprès de nos jeunes, Français établis à l'étranger de plus en plus nombreux. Les Journée défense et citoyenneté représente à ce titre une excellente opportunité pour acquérir les premières connaissances indispensables à la compréhension des grands enjeux de défense qui touche notre pays. Mais ces journées ne sont à mon grand regret que rarement organisé alors même que les jeunes Français résidant à l'étranger sont déjà exclus du SNU. Et je défendrai des amendements en ce sens. Ne perdons pas de vue que les Français établis hors de France demeure la vitrine de notre pays à l'international. Un de nos meilleurs outils d'influence, un relais essentiel chez nos partenaires alliés et parfois admis les Français établis hors de France sur des Français à part entière des citoyens engagés qui ne demandent qu'à servir leur pays que ce soit par la promotion de nos intérêts économiques par une vague géostratégique. Par une cyber défense adapté ou encore par une lutte contre la désinformation, c'est un devoir et une responsabilité de les soutenir, et donc de leur donner dans ce texte, les moyens de mieux servir notre pays nos armées et nos valeurs ne les décevrons pas. Merci de votre attention.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre Mesdames les Ministres, Monsieur le Président chaque Christian Cambon, mesdames, messieurs, cette loi de programmation militaire est essentiel. Pour plusieurs raisons, d'abord. Le contexte géopolitique internationale. Nous avons tous en tête. La guerre en Ukraine, c'est le fait générateur. Mais il y a d'autres événements évidemment à suivre et. Première pensée pour l'Afrique, nous avons eu le débat il y a quelques jours et c'est vrai qu'il y a une dégradation incontestable de la situation en Afrique avec le développement d'un sentiment anti-français. Je pense au Mali. Je pense ouais Centrafrique. Malheureusement au Burkina Faso et puis. Au Maghreb, ça été évoqué la semaine dernière ici même. Par nos outre-mer, nous avons une responsabilité. Sur l'ensemble du globe. C'est à la fois un atout mais c'est aussi pour nous évidemment une une obligation et je salue l'ensemble de mes collègues ultramarins présent. Ça veut dire que ça va nécessiter des moyens maritimes dont tu nous reparlerons, monsieur le ministre. Et puis il y a d'autres théâtres d'opérations potentiel, je pense à l'Iran, l'Afghanistan, la Corée du Nord. Toute cette accumulation de menace sur tous les continents vient obligés effectivement en moyens nouveaux et c'est ce qui fait que nécessitait d'actualiser la loi de programmation militaire. Et puis les guerres sont multiples, c'est l'autre grande raison. C'est le grand changement du XXIe siècle. Il y a les vieilles guerres les guerres brutal. Les images que nous voyons en Ukraine rappelle celle de nos livres d'histoire sur la première guerre mondiale. Une époque où chaque était un couloir de la mort. Et puis il y a des nouvelles guerres pernicieuse. Il y a effectivement ces gardes technologique. Où on a une montée en puissance. De l'informatique, du numérique, du quantique au cyber ou les drônes sont partout et demain l'Intelligence artificielle. Et puis. Il y a ces guerres aussi. Lié au terrorisme tout à l'heure notre collègue. Qui intervenait Amal avaient mis en date comme ça. Tournant le 11 septembre. Bien sûr, nous avons tous en tête le 11 septembre 2001. Monsieur le ministre, j'ai une pensée parce que j'espère que vous en ferez la commémoration dans quelques semaines pour le Drakkar au Liban. Octobre 1983 où déjà le terrorisme était venu. Voilà se mêler à à la guerre. Et l'ensemble de de ces données vient justifier des moyens nouveaux. Indispensable face. Aux menaces. Et a diversification des menaces. C'est un, un effort indispensable face à la conflictualité de demain avec nécessité. De transformer nos armées. d'anticiper et bien évidemment d'associer la nation parce que ces risques nouveaux font qu'il y a une Exposition civils. Alors une fois qu'on a posé le cadre évidemment il y a la question des moyens et des ressources humaines, les moyens Monsieur le Ministre, ils sont essentiels. Vous en avez. Longuement évoqué tout à l'heure avec le rapporteur Christian Cambon mais plusieurs veut me vient en tête la la tête de pont. La tête de chapitre, c'est évidemment la dissuasion nucléaire et nous devons la rappeler. Nous devons réaffirmer cette dissuasion nucléaire et puis derrière il y a les moyens maritimes. Où en sommes nous ne sous-marin où en sommes-nous d'un prochain porte-avions et nous portons ce projet cher mais essentiel. Il y a la question des des stocks stratégiques, pardon. Et il faut évidemment donner un signal fort par cette loi de programmation militaire avec nos équipementiers et puis y a toutes les questions des livraisons qui sont d'actualité Rafale scorpion Griffon Jaguar. Nous devons avoir par ce débat. Et parce. Ce qui ressortira ici du Sénat Monsieur le Ministre, un message fort pour l'industrie de guerre. Un mot sur les ressources parce qu'effectivement vous faites des réserves. Une des pierres angulaires des mobilisations possible alors. Les questions qui viendront et que nous nous posons légitimement dans cette assemblée sont évidemment. Quel calendrier. Quelles formations, quels équipements. Et donc. Nous sommes là sur le, ce débat maintenant, du budget. Monsieur le Ministre et je crois que face. À ce qui se présente, nous ne pouvons pas trop attendent et tout à l'heure le président Cambon a parlé de cadencement. Je crois que c'est le terme exact, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une montée sans doute plus linéaire des questions budgétaires pour soutenir notre armée évidemment je sais combien le Sénat ici dos s'adresse à l'ensemble des forces armées militaires et de gendarmerie, un message de soutien en tout cas il est là aussi en tant que. Questions de défense nationale. Plus de question de perte de temps, le temps perdu ne se rattrape le plus donc ce débat et et capital avec un message de soutien à nos armées, je vous remercie. La discussion générale est Close et nous allons passer la discussion du texte de la commission. Eh bien nous commençons par l'article 1er sur lequel il n'y a pas d'amendement et je le mets donc aux voix. Qui est pour l'article 1er. Qui est contre. Y a-t-il des abstentions il est adopté. Nous arrivons à l'article 1er bis et nous commençons par l'amendement 54 rectifié que présente Monsieur Guillaume qui a la parole.

les grands objectifs de la défense nationale qui sont protéger la population du territoire national outre-mer compris lutter contre les menaces actuelles et à venir concourir à la sécurité collective et la défense de la paix dans le cadre de nos alliances et partenariats, d'une part et du multilatéralisme. D'autre part. Et enfin, renforcer le lien entre la nation et ces armées. Cet amendement vise à compléter ses objectifs en rendant explicite la protection des Français à l'étranger. En effet le nombres des ressortissants français, voyageant ou résidant à l'étranger, ne cesse d'augmenter leur sécurité peut être menacée lorsqu'ils se trouvent dans des espaces mal contrôlée qu'il s'agisse de pays aux structures étatiques défaillante ou de zones maritimes en proie à la clinique Si depuis une quinzaine d'années, les attaques visant collectivement une communauté française expatriée ont été rares. Le risque d'enlèvement perdure. Par ailleurs, nos compatriotes peuvent régulièrement au pris dans des situations exceptionnelles qui nécessite une action d'urgence, que ce soit des coups d'État. Une guerre civile ou une catastrophe naturelle comme vous le savez en avril dernier, l'armée française a procédé à l'évacuation rapide et un toute sécurité de citoyens français du Soudan. Pays en proie à un conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires. J'en profite pour saluer l'effet que l'efficacité de nos armées qui dans des situations sont très réactive et à la hauteur des enjeux. Aussi il me semble utile de rappeler cette fonction de protection des Français résidant hors de France que les militaires sont régulièrement amenés à mettre à l'heure, je vous remercie. J'ai le président c'est un excellent amendement que la commission soutient et nous nous associons à l'hommage qui a été rendu à nos forces françaises. Qui dans l'opération sagittaire ont réussi un exploit exceptionnel. Avis favorable, Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Oui, monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, sur la finalité de l'amendement, il y a pas de doute et sagittaire est venu montrer effectivement comment les forces armées ont mené à bien cette mission d'évacuation d'ailleurs si on se compare avec d'autres nations européennes on a su le faire vite en réactivité seul faisant jouer à la fois nos capacités articuler forces spéciales j'en dis pas plus. Aviation de transport mais aussi nos accords de défense avec Djibouti. Et c'est un cas pratique intéressant d'ailleurs sur les, les types de d'évacuation que nous pourrions être amenés à accomplir dans les années qui viennent, même si je ne veux pas douché l'enthousiasme de la presse sur le sujet, on était quand même sur un nombre de ressortissants français limitée et que dans d'autres pays d'Afrique. On est évidemment sur des communautés qui sont beaucoup plus importantes et qui nécessiterait évidemment une planification peut être un peu différente, c'est pas pour amoindrir évidemment le travail des forces armées, c'est juste pour nous inviter collectivement à réfléchir. Alors après c'est c'est un. La position du gouvernement au fond sur cet amendement et. Va aussi au fond dépendent de manière globale de ce qu'on attend du texte. Si on y rigoureux. Si on n'adopte l'amendement si vous adoptez, pardonnez-moi l'amendement que vous proposez. On encadre et on restreint la capacité à protéger puisque ça laisse à penser au fond que la protection de nos ressortissants à l'étranger ne sont que sur le terrain sécuritaire et militaire. Or comme vous le savez d'autres ministères évidemment procèdent à des évacuations et des protections sanitaires. Non mais on est dans la partie normative. On n'est pas dans le rapport annexé. C'est pour ça que je. Dans la partie rapport annexé, on pourra peut-être se permettent des des signalements politique sur un certain nombre de sujets sur la partie normative sur la partie légale en tant que législateur vous produisez du droit donc je je je le dis, il est évident que les évacuations se sont dans le domaine des compétences. Quand vous êtes sur des évacuations sanitaires. Individuels ou même collectives ou semi-collective on n'est pas forcément dans le domaine des armées. Donc moi je suis plutôt réservé en fait sur la fidélité, je comprends très bien l'amendement mais si on est un peu rigoureux dans le le le normatif que l'on produit on vient en fait un peu restreinte, les choses donc demande de retrait, le cas échéant, Monsieur Guillaume de la loi de programmation militaire qu'on envoie et que quand tu les Français et notamment leur militaires font des des actions exceptionnelles de qualité, il est important de renvoyer l'ascenseur. Messieurs Cadic demande a expliqué son vote.

aussi bien tous les ressortissants européens et on ne peut en témoigner. À chaque fois et y compris étrangers on sait. Avec quelle humanité nos forces interviennent quand il faut secourir des étrangers. Quand il y a un problème. On l'a vu par le passé. S'il y a effectivement des sujets améliorer, c'est tout ce qui est. Plan de sécurité nos élus des Français de l'étranger le rappel souffrent souvent qui qui soit mieux associés lorsqu'il y a un problème, merci. Mon cher collègue, d'avoir noté ce point évidemment je vous soutiendrai et. Et et sincèrement, encore une fois c'est pas du tout pour mettre en doute parce que vraiment à chaque fois qu'on a eu des interventions de nos forces armées pour nous protéger quand il y avait. Un des. Comment dire. Un défi sécuritaire à l'étranger, ils ont toujours été au rendez-vous donc pour nous et pour tous les Européens. Merci. pour d'abord pour plus largement sur sur l'article qui est proposé et puis sur le moment que nous souhaitons, c'est vrai que il nous semblait. Parce que nous sommes à l'origine de cet article là il me semblait nécessaire de, de mettre un chapeau parce que F. si effectivement il y a des éléments dans le rapport annexé chacun connaît aussi. Le destin qui je crois est proposé au rapport annexé nous semble important pour vu. Je vous rappelle. La loi sur l'aide publique au développement. La différence entre la partie normative et le rapport annexé, nous pourrions parler des heures évidemment. Donc il me semble important de mettre un chapeau et c'est vrai, d'essayer de préciser le sens de cette loi de programmation militaire d'essayer d'avoir quatre objectifs qui soit totalement clair avec notamment la question la protection des Français. Donc c'est pour ça que le considérons que cet amendement qui est proposé, on va dire ajoute et c'est une bonne chose ou alors une précision pour dire ça. Je crois que c'est une bonne chose et nous sommes favorables bien sûr à l'amendement qui est proposé. Monsieur le Ministre vous souhaitiez de nouveau exprimé votre avis. pour le préciser donc sagesse. Qui m'amène de commentaires hein sur l'ensemble du chapeau. Je pense qu'il va dans le bon sens et c'est pour ça que le gouvernement d'ailleurs n'apporte aucun n'amendement et je pense que il. Il fait bien la synthèse au fond des grands attendu politico-militaire mais aussi diplomatique telle qu'il a été introduit par la commission et comme je vois qu'il y a pas eu d'autres amendements en particulier dessus je je crois qu'il est, il est en tout cas consensuels comme je l'ai dit tout à l'heure à à la tribune. En tout cas pour les sensibilités politiques telles qu'elles sont représentées ici en grande partie au Sénat après c'est une autre affaire et 2ème des choses moi je voulais juste éclairé le, le Sénat pour la mémoire des débats. Ce que je veux juste évidemment d'où la vie de sagesse et non pas un avis purement favorable. Ça veut dire que cette mission de protection des ressortissants ne repose pas que sur le seul ministère des Armées. Mais l'éclairage du Parlement est en fait ça. Je mets aux voix l'amendement 54 rectifié avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse. Du gouvernement qui est pour cet amendement. Ah mon. Abstention, pardon, donc il est adopté, je mets aux voix l'article 1er bis.

Comme ça ne vous a pas échappé, l'article 2 est réservé jusqu'à la fin de l'examen du texte. Nous passons l'article 3 sur lequel le président Retailleau a demandé la parole. Merci monsieur le président. L'article 3. Monsieur le Ministre, c'est la clé de voûte de la LPM. Et si j'ai souhaité prendre la parole, c'est à la fois pour vous répondre. Répondre à l'article de ce matin qu'on a tous lu répondre à vos propos tout à l'heure, mais aussi pour préciser notre pensée. Pour la préciser, pour aujourd'hui et pour demain, pour la commission mixte permanente. Je ne reviens pas sur le fait et nous le pensons tous ici, sur ces bancs, quelles que soient les bancs sur lesquels nous sommes assis que 413 milliards d'euros. Ça n'est pas rien, c'est un vrai effort simplement nous voulons. Dans cet article lever un doute, un doute qu'est lié à une incertitude. Un doute qui est liée aussi à une facilité. L'incertitude ce sont les crédits qui ne sont pas budgétées. Ça n'est pas nous qui l'avons pointé c'est le Haut conseil aux finances publiques et notre trajectoire a un mérite c'est que. Il matérialise cette voir matérialise concrétise les 7, 4 milliards. Qui ne le sont pas. Et le doute lié. Évidemment au reste, c'est-à-dire à la facilité, c'est que l'essentiel. De l'effort est reportée après 2027 et nous on veut que ça soit une progression qui soit linéaire. Parce que sinon c'est le même effort les mêmes marche que la LPM actuelle. Parce que c'est maintenant la guerre c'est maintenant qu'on doit faire un effort. Parce que c'est maintenant l'inflation que l'euro d'aujourd'hui n'a pas la même valeur il vaut plus que l'euro de demain. Voilà ce que je voulais vous dire et on veut s'assurer dans un monde chaotique et nous ne sommes pas du tout d'accord avec les 420 milliards. Que vous avez cité ces 413 milliards. Et d'ailleurs. Nous l'avons vérifié aussi avec notre commission des finances. C'est notre façon de compter l'argent public. nous avons Lyon si nous avions voulu. Sortir de l'enveloppe. Alors dans le premier alinéa de l'article 3, nous n'aurions pas inscrit 413 milliards. Mais 420, donc mes collègues, mes chers collègues, on modifie le cadencement mais on reste dans l'enveloppe décrite défini à Mont-de-Marsan par le président de la République, je tenais à le dire solennellement. Sur cet article 3, nous avons quatre amendements en discussion commune le 1er 66 qui est présenté par notre collègue Todeschini qui est la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre Mesdames des des ministres ce le président de la commission. commission. Ce ministre par cet amendement. Nous voulons simplement vous avez fait une large communication sur les efforts. Jamais réalisée sur des lois de programmation militaire. Nous voulons simplement ramenée à sa juste proportion. Cet effort budgétaire. Le chevauchement calendaire des de loi de programmation militaire permet au gouvernement de budgétiser sur les et les exercices 2024 et 2025 dans les 2 lois de programmation militaire. Dans la LPM 2019 2025. On estime à 97 milliards, ce qui était prévu pour les Budgets 2024 et 2025. Ils n'ont jamais été budgétisé. Parce que d'abord le il y a eu une absence de véritables. Réactualisation en 2021 mais ça c'était. Un autre ministre, pas vous et puis les cours autrement de l'actuelle loi de programmation. Mais Amène à cela les crédits 2019 2025 il devait être de 295 milliards. Ils seront tout simplement pour 2019 2023 de 198 milliards. La loi de programmation militaire 2024 2030 réaffecte ainsi les 97 milliards que j'ai cité l'effort réel serait donc de 303 milliards auxquels il faudra un jour soustraire l'inflation d'un peu près 30 milliards que vos services et que le gouvernement ont estimé. Merci cher collègue ensuite l'amendement 282 du gouvernement. D'en faire un amendement d'appel je suis sans illusions sur son issue. Mais ce qui permet aussi d'avoir le, la grande clarifications et précisions car au regard de ce que vient dire le président Retailleau en fait je crois que politiquement ça peut converger mais que dans l'écriture du texte on ne partage pas la même lecture de technique. Alors il y a 3 sujets devant nous hein sur lequel je n'y reviens pas Monsieur le Ministre Todeschini c'est les 30 milliards ne sont pas à soustraire puisqu'ils sont déjà dans la copie. Je le redis, je l'ai dit à plusieurs reprises en en audition. Je l'ai dit au sénateur de Lège. Dans ses fonctions de deux rapporteurs et d'ailleurs il je m'étais engagé auprès de lui à lui communiquer par l'écrit, les modalités de calcul de cette inflation. Je l'ai fait par écrit, donc je pourrais répondre à vos questions. Une nouvelle fois sur ce sujet mais c'est pas à 413 ou 420 ou 400. Ce que vous voulez moins 30 milliards. Ça c'est pour le débat sur l'inflation, c'est déjà dans la copie et d'ailleurs le principe d'une programmation des années 60 à nos jours, c'est évidemment d'intégrer un aléa dont nul ne sait aussi ce qu'il deviendra est ce que, au fond, les facteurs macro-macroéconomiques se retourne, auquel cas ça sera une bonne nouvelle puisque les. les. Projections sont plutôt prudentes dans les critères que nous avons retenus ou est-ce qu'auquel cas ça s'aggrave et je vais vous dire une chose, mesdames, messieurs les sénateurs. Si ça s'aggrave ça s'aggravera. Pour l'ensemble du budget de l'État et pour d'autres programmes et on aura l'occasion de toute façon d'y revenir et au regard. Monsieur le Président encore bon des engagements que nous avons pris de documenter l'inflation, année par année en loi de finances des de toute façon les documents budgétaires annuelles, vous verrez les impacts sur l'inflation et vous constaterait d'ailleurs sur ce qu'on appelle le physique, c'est-à-dire en clair, de voir des décalages de commande. Ce que vous n'avez pas constaté jusqu'alors première familles de sujet l'inflation on est revenu de nombreux soins en commission. Mais je voulais le refaire devant. 2ème, sujet qui est la deuxième partie du propos du président Retailleau. C'est la dynamique où le rythme en quelque sorte. De de l'effort budgétaire. Alors il y a, j'ai envie de dire, il y a là il y a la politique au sens noble du terme ou évidemment quand vous dites que l'essentiel de l'effort est après 2027 comme moi je regarde depuis 2017 je vois quand même 2 tiers d'efforts entre 2017 et 2027. Mais je reviendrai dans un instant. Et donc je considère que cette trajectoire là, évidemment, elle n'est pas la même marge, comme on dit puisque dans un escalier si vous montez sur la même marche globalement au fait du surplace et qu'on est bien sûr 3 milliards qui s'ajoutent à chaque fois. Après il y a la dynamique de cette de ces marches sur lequel on pourrait revenir et il y a un 3ème sujet je les découpe en morceaux pour. Ils se rencontrent, mais ne ce ne sont pas complètement joint c'est la la somme globale

ma difficulté d'où peut être aussi cet article cette interview de ce matin, c'est que nous, dans notre manière de non. Monsieur le président. Quand. Certains membres de votre groupe tweet quelques minutes après le discours du président de la République à Mont-de-Marsan. C'est le sénateur Perrin. Je ne m'en offusque pas lorsque le Sénat et c'est de bonne guerre trouvent que le texte manque d'ambition. Je ne m'en offusque pas, c'est aussi le jeu démocratique. Vous avez une lecture et un avis sur le projet de loi portée par le gouvernement, le gouvernement peut avoir un avis sur le texte tel qu'il sort de la commission. Ça me semble sain au contraire que c'est lieux. Ça a eu lieu en commission par 3 fois sous l'autorité du président Cambon et j'en informe aussi de nos concitoyens. Il y a pas d'agressivité, vous le savez très bien, non. En revanche, techniquement je je je veux quand même vous partagez la manière dont on lit le chiffre près. On verra ça peut être à d'autres débats plus politique dans un autre cadre, mais je pense utile de. De redécaler, la copie du gouvernement. Ce que j'ai fait par courrier en date du 2 juin dernier que j'ai adressé un certain nombre d'entre vous pour expliquer comment l'affaire était monté, vous avez 400 milliards d'euros de crédits budgétaires pour 413,3 milliards d'euros de besoins militaires. Cette distinction, elle se documente par 13,3 milliards d'euros que l'on. Découpe de la manière suivante, 5,9 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires dont on estime désormais qu'elles sont sécurisées. Il a eu de nombreux débats sur le sujet et ça on est d'accord mais on les retrouvera tout à l'heure. Ensuite, nous avons 1,2 milliards d'euros, qui est une départ du financement de l'Ukraine, hein, vous avez en tête, qui a trois modalités de financement différent de l'Ukraine, là on est sur les prélèvements du parc des armées qui donne lieu à une, un recomplètement par du matériel neuf. En clair, quand on sort un AMX 10 RC, ou lorsqu'on sort un crotale c'est remplacé par un jaguar dans le 1er cas et par un VL Mica. Dans l'autre cas, on a donc touché au format des armées, lesquels matériel, même s'ils sont anciens étaient encore dans la cible capacitaire pour au moins 2030 voire 2035 et donc c'est là où on a provisionné se 1,2 milliards d'euros pour l'Ukraine et puis ensuite on a 6,2 milliards d'euros de 2 outils différents d'ailleurs, hein, qui est un outil qu'est le report de charges. On nous a suffisamment reproché de ne pas. Suffisamment bien gérer l'inflation pour désormais balayé d'un revers de main l'outil qui de tout temps permet de gérer l'inflation et la 2ème des choses et frictionnel qui sont au fond les retards qui sont déjà intégrées dans la copie des 413 milliards. Alors, avec du recul. Bien m'en a pris de de de faire ce distinguo puisqu'en fait il se trouve et là même si j'y suis pour rien, je le soufflé à l'oreille de mon voisin, il se trouve que dans les programmations militaires précédentes. Ça a toujours été construit comme ça sauf que ça n'était jamais montrées au Parlement. Pour des raisons je vous laisse deviner. Et si je vais vous donner un exemple très concret que est la loi de programmation militaire actuelle, celle dans laquelle nous sommes encore sous l'empire, vous aviez voté 295 milliards d'euros de ressources budgétaires. C'était donc une LPM à 295 milliards d'euros. Sauf que nous étions à 304 milliards d'euros de besoins militaires et ce trois, quatre n'avait pas été montré au Parlement et donc ce que j'ai souhaité au regard des sommes importantes qui sont en jeu désormais dans ses programmations et aussi parce que c'est la modification. On en a suffisamment discuté avec les uns et les autres dans le tableau capacitaire c'est pas tant les commandes qui nous intéresse, mais réellement ce qui est livré aux forces armées c'est de repartir du besoin militaire et en face, ils mettent les ressources budgétaires qu'elle soit extra budgétaires ou sur le budget de la nation. Ce qui nous amène à la lecture de ce qui a été modifié en commission. Je ne parle pas des marches du rythme hein je je sors les marchés et le rythme de nos, de nos conversations le le temps d'un instant. La copie du Sénat en tout cas telle qu'elle existe au moment où je vous parle, c'est 407 4 milliards d'euros de crédits budgétaires. Auxquels s'ajoutent toujours les 5,9 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires. Et auxquels s'ajoutent toujours les 7,4 milliards de reports de charges parce qu'ils sont dans la programmation. Donc en fait mais si ils sont dans la programmation. Ou alors ça revient à les compter 2 fois. Donc vous les compter 2 fois. Mais non on les compte qu'une seule fois puisqu'ils sont dans les 413. Mais non ils sont, par définition, on a déjà des indications sur des retards. Alors très bien, Monsieur le Président, Retailleau allez je prends le problème par l'autre bout. Si vous ne partageait pas cette lecture là je vais dans l'autre sens. Vous avez déjà 413 milliards d'euros dans le tableau capacitaire. Il se trouve que la commission a déjà rajouté un milliard d'euros pour l'entraînement, 200 millions d'euros pour les ressources humaines et des amendements à venir tablent sur 2 milliards d'euros de plus du capacitaire, ça veut dire que déjà même si vous ne partagez pas ma lecture sur les marges frictionnel. Nous sommes déjà à 3,2 millards d'euros en plus des 413. Alors là vous allez me dire non, on reste à 413, là c'est le moment de la vérité parce que si vous restez à 413 avec plus de MCO, plus de moyens capacitaires et plus d'entraînement. Ça veut dire qu'il y a des renoncements quelque part. Et donc là pour le coup. Je, je vous le dis, si vous êtes à 416. De ma lecture est à 420 mais si vous ne la partageais pas je l'abandonne l'espace d'un instant, et si on reste sur 416,2. Ça veut donc dire que ces 3,2 milliards. Faut bien les trouver quelque part donc, soit vous êtes tout de suite 413. Soit il a des renoncements sur d'autres postes. Mais il y a pas il y a pas d'argent magique comme dirait quelqu'un que je connais bien, qui m'a nommé et donc je, je le dis, non mais. Comprenait bien mon état d'esprit n'est pas à la polémique, je le dis sincèrement, je dis juste que c'est compliqué sur une programmation comme celle-ci de ne pas s'accorder techniquement sur la lecture des chiffres donc. Je l'ai écrit, je l'ai répété, c'est pas nouveau. Monsieur le Président Retailleau quand le ministre Longuet qui est mort membre de votre groupe était ministre de la Défense les marges frictionnel existait déjà quand Alain Richard pardonnez-moi madame la présidente, je pensais qu'il présidait toujours la séance était ministre de la Défense, les les les marges frictionnel existait déjà quand Jean-Pierre Raffarin présidé la commission et qu'il était 1er ministre les marges frictionnel existait déjà, donc je n'ai fait que montrer. Une méthodologie qui est vieille comme Hérode mais au delà même de la méthodologie vieille comme Hérode. Il y a une réalité c'est que vous avez décidé. Mais vous êtes parlementaire est complètement souverain dans cette manière de faire hein je je le je le respecte mais on est au-delà des 413. Et ça pour le coup, je le dis, je ne suis pas 1er ministre ou ministre du Budget. Mais évidemment, ça pose des questions pour la soutenabilité budgétaire globale donc. Ça c'est c'est un point important parce que il y a l'inflation. Il y a les marches. Et il y a l'enveloppe globale et sur l'enveloppe globale. Soit il y a une lecture on est à 416 de c'est factuel. La la la la colonne des dépenses et augmenter en commission. Ça je veux bien tout ce qu'on veut mais c'est et de l'autre côté au-delà de même de cela. Par définition, on a une lecture sur les marges frictionnel qui n'ont pas disparu parce qu'il ne s'agit pas de les budgétés pour qu'elle disparaisse. Donc moi je suis prêt évidemment, s'il faut même suspendre pour avoir une, une réunion sur le sujet, je l'aurais bien volontiers de nouveau parce que je veux vraiment montrer la bonne foi du gouvernement dans cette manière de faire, je pense que l'exécution à l'euro près. De la LPM désormais nous oblige justement à être rigoureux, sur sur le sujet en tout cas moi je reste à la disposition de du Sénat pour nous entendre sur ce sujet dont nous ne faisons pas un préalable, politiques ou politiciens mais bel et bien un élément de clarification important si on reste à 413 milliards. C'est donc à 113 milliards de dépenses, or là au moment où je vous parle on est déjà au moins à 416,2 si ce n'est qu'elle s'en va donc l'amendement est défendu. Sur le contenu, il remet les marches la trajectoire telle qu'elle était présenté à l'Assemblée. Mais enfin vous l'avez compris, c'est pas tant que la trajectoire et les marches aussi l'amendement d'appel pour avoir cette conversation et cette discussion et ce débat noble sur les 3 aspects inflation marche. Mais surtout enveloppe globale désormais puisque là il y a un enjeu de soutenabilité qui m'inquiète beaucoup. Merci, monsieur le Ministre. Non monsieur Perrin. L'amendement numéro 6. Monsieur de Lège au nom de la commission des finances. Merci madame la présidente. Ai effectivement souhaité. À nouveau présenté cet amendement de la commission des finances. Pour plusieurs raisons, d'abord pour soutenir. La commission de la Défense sur le chiffre de 407 milliards, c'est notre analyse aussi à la commission des finances, je tiens le dire. 2ème raison c'est que nous considérons que on ne peut pas reporter l'effort au prochain quinquennat. Mais à cela s'ajoutent d'autres arguments. Monsieur le Ministre. C'est que j'entends bien toutes les arguties de Bercy, on a même vu un haut gradé. Faire le tour des sénateurs pour nous donner des leçons de. Calcul budgétaire, on s'en serait bien dispensée. Mais je dois dire que votre explication ne nous a pas plus convaincu parce que ça reviendrait à dire que au fond on finance une partie de l'objectif capacitaire. En espérant qu'on ne va pas l'atteindre ou pire qu'on va tout faire pour digérer soit les paiements soient les livraisons et il s'ensuit forcément il a un moment ou un autre. Il y aura une conséquence sur la loi de programmation des finances publiques qui d'elles-mêmes se trouvera frappé de la même insincérité et si vous ne souhaitez pas le mot insincérité disons du même doute. Je voudrais profiter. Monsieur le Ministre de cet amendement pour vous poser de questions. La première, dans quelles conditions nous allons rentrer dans la nouvelle loi de programmation militaire par rapport au report de charges parce que ceci n'est pas tout à fait neutre, sauf erreur de ma part, c'est 5 milliards. Ça veut donc dire qu'il y a a 5 milliards de cavalerie qui s'ajoutent aux sept que vous voulez nous expliquer. Qu'il n'existerait pas et puis j'ai souvenir que en avril. Dans un interview vous avez déclaré que, en 2013 2023, le budget de la défense serait abondé d'un milliard 5 il faut concrétiser nous en dire un petit peu plus sur ce milliard cinq, je vous remercie.

et de permettre que les montants. Soit effectivement ceux qui seront perçus par nos armées. Vous avez évalué, j'ai dit tout à l'heure à 30 milliards. Les sommes qui seront consacrés à l'inflation pour 2024 à 2030. La seule solution trouvée. Elle a été cité déjà c'est d'utiliser le report de charges pour neutraliser ses effets d'un de l'inflation et donc. Le respect à l'égard de nos armées, de ce qui était prévu. La sincérité de cette loi de programmation militaire serait totale si elle était exprimée en euros constants. Merci alors l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président. Sur ces quatre amendements. Merci madame la présidente. Alors sur le 66. Cet amendement était satisfait puisque je rappelle que en commission, nous avons adopté une nouvelle trajectoire. Donc il est satisfait. Et je propose que les auteurs que l'auteur de l'amendement 66 puisse le retirer. Car nous aurions dans ce cas-là une trajectoire différente de celle que nous avons adopté.

Je reprends votre répartition 413 milliards annoncé par le président de la République à Mont-de-Marsan, repris par tous les orateurs, tout le monde a en tête l'idée selon laquelle la le la nouvelle LPM porte sur 413 milliards. 400 milliards sont budgétés 5 5 milliards neuf font l'objet de ressources qui sont bien identifiés. Je les rappelle et bandes de fréquences. Le produit de. Le produit des des soins. Dispensés par les hôpitaux militaires, la vente de l'immobilier. On les accès reste ces fameuses 7 milliards. Je veux dire c'est une étrange méthode qui consiste à dire, ces 7 milliards ne font pas l'objet de budget mais de de ressources extra-budgétaires, mais c'est quoi les ressources extra-budgétaires de 2 choses l'une,

pour évoquer ce sujet. Nous ce que nous voulons c'est sécuriser être assuré que 413 milliards vont être dépensés. Pour le renforcement de nos forces armées et pour nous les reports de charges, c'est un sujet que nous aborderons que nous détestons car nous savons très bien ce qui se passe, on l'a vu dans la précédente LPM et quand on a demandé une actualisation, on s'est aperçu qu'il manquait 10 milliards parce qu'on n'arrêtait pas de reporter déjà alors de 2 choses l'une, ou on a 413 milliards à dépenser où on les a pas, c'est ça que ces ces difficultés où cet arrangement. Oratoire qui laisse à croire que le Sénat veut dépenser plus, nous maintenons l'idée sur laquelle et je suis prêt, nous sommes prêts à en discuter avec vous, nous nous je pense ici qu'il y a le sentiment unanime qui consiste à dire que on veut rester dans l'enveloppe de 413 milliards on n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dire il y a des il y a 400 milliards qui sont budgétés et puis il y a 7 milliards qui sont des ressources extra-budgétaires. Alors vous nous parlez des marges frictionnel. Vous nous parlez des. Des programmes qui sont en retard. ne sont pas. Et qu'ils ne sont pas exécutées bah dans les lois budgétaires qui se succéderont vous reprendrez ces chiffres. J'ai repris la comparaison que j'ai dit dans mon intervention si vous commentez des des A400M et qui ne vous sont pas livrés à vous les payez pas et donc vous avez cet argent qui est disponible. C'est ça que nous n'arrivons pas à saisir par quel subterfuge. Vous avez présenté cette affaire, il eut mieux fallu dire la LPM, ces 400 milliards ou 405 milliards, c'était clair, tout le monde aurait compris. Je pense qu'on on ne se serait pas livré depuis des semaines et des mois à des débats et des exégèses sur le fait de savoir où sont les justificatifs futur des 7 milliards et demi donc c'est pour cela que évidemment nous maintenons notre amendement dans le. Nous on nous maintenons notre position et nous nous Nous émettons un avis défavorable. À l'amendement du gouvernement parce que nous souhaitons qu'il y ait des éclaircissements complémentaires et que l'on puisse évidemment en discuter. Sur l'amendement numéro 6 de notre collègue de Lège donc qui propose une trajectoire dont les deux premières annuités sont les mêmes que celles qui sont proposées par le gouvernement, avec un effort complémentaire là je sollicite notre collègue pour que au nom de la commission, cet amendement puisse être retiré puisque nous avons adopté en commission, une autre trajectoire qui a rassemblé. La majorité de notre commission c'est une accélération de surcroît qu'est souhaitable, je le redis, c'est en ce moment que nous sommes non pas en guerre mais en situation excessivement grave étendue par rapport à l'Ukraine. C'est en ce moment que nous livrons des armes les armes que nous livrons, nous ne les avons plus et si jamais il y avait un conflit de haute intensité. Nous n'aurions plus les AMX nous n'aurions pu les armements c'est les. Ce n'est pas le moment de baisser la garde et c'est ce pourquoi cette accélération est possible. Par ailleurs, vous avez quand même prévu entre 30 et 60 milliards. D'effet d'inflation tout ce qui est dépensé maintenant ne sera pas sujet. À l'érosion de l'inflation, donc c'est ce pourquoi. Nous proposons que cet amendement six puisse faire l'objet. D'un retrait sinon l'avis sera défavorable. l'amendement 67 relatifs à la d'option d'une trajectoire en euros constants là c'est évidemment un avis défavorable car pour le coup ceci entraînerait. Une hausse de 30 à 60 milliards d'euros courant supplémentaire là nous ne pouvons pas rentrer dans cette logique, même si nous comprenons encore une fois, le sens de l'amendement et que comme vous l'avez dit, chaque année lors des Budgets, on aura une idée précise du dérapage de l'inflation, donc avis défavorable sur le 67. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, mesdames messieurs les signataires. Alors si je reprends les amendements le 66 du groupe socialiste présenté par le ministre, est On peut prendre les chiffre par tous les bouts. Si on ne prend pas sur l'ensemble de la programmation avec les chevauchements d'années mais on avait déjà eu le débat avec le sénateur es mal en commission on prend le budget annuel de la défense en 2017. On prend le budget annuel telle qu'on le propose en 2030 et on voit qu'il a doublé. oui mais le tel qu'est rédigé l'amendement on, on voit bien quand même qu'on cherche à tourner autour du pot. Bon non mais je le dis parce que. Allez je je dis j'ai déjà répondu plusieurs fois j'ai reviens pas sur l'amendement. Du gouvernement. Je crois que j'ai dit ce qu'il avait à dire mais je pourrais revenir à la faveur de l'amendement de monsieur Bon déjà. Monsieur le sénateur Joe. Je vois que vous essayez de faire en sorte que les deux premières annuités correspondent aux 2 premières annuités de la programmation des finances publiques que vous avez voté. C'est un argument que je manie avec précaution puisque ce que le Parlement a fait le Parlement peut très bien l'adapter mais enfin je salue quand même la cohérence ou en tant que commissaire aux finances. Vous essayez évidemment de de de vous assurer la soutenabilité. C'est cette affaire et donc vous proposer au fond dans les années, dans lequel la LPFP n'a pas encore inscrit une somme si je comprends bien d'accélérer au moment où justement cette trajectoire n'a pas encore été adoptée par le Parlement. Si j'ai bien compris l'esprit de votre amendement. j'ai émis un avis défavorable mais je vois ce qu'intellectuellement vous vous voulez faire et qui pose la bonne question de la soutenabilité pour nos finances publiques sur le report des charges. Globalement, nous sommes à 4 milliards d'euros au moment où nous parlons. Alors quand le président comme on dit, on a horreur des reports de charges. Moi non, parce qu'en fait ça nous permet de traiter l'inflation et s'est entendu avec les industriels et en plus les industriels bénéficient d'intérêt dans cette affaire, c'est-à-dire que on est sur de tels programmes d'une telle masse que le report de charges nous permet aussi de déclencher la facture en accord avec l'industriel au moment où les critères macro-économiques sont les plus satisfaisant pour le contribuable. et je je comprend pas l'acharnement sur le report de charges. Les autres ministères se pardonnez-moi cette expression se roulerait par terre pour avoir les mêmes outils de gestion de l'inflexion que le ministère des Armées. Mieux que ça, ce sont souvent des outils qui ont été suggérés par les parlementaires dans des lois de programmation, il y a 10, 15 ou 20 ans, considérant que les lois de programme était-elle. On va revenir à au recours, en euros constants, qu'il fallait permettre à l'ordonnateur des dépenses pourvu qu'il le montre dans la loi de finances, ce que nous faisons. Quel était le mécanisme de reports de charges

je veux bien qu'on s'en prenne à cette à ce mécanisme-là c'est un mécanisme qui est bénéfique pour les armées. Voilà, ne pas dire mieux. Interrompt le ministre Richard le le ministre Longuet pour ceux de mes prédécesseurs qui siège encore ici, moi je le dis, je défends pour le coup, ce mécanisme-là quand Gérald Darmanin et votre tu ne vous fait voter pardonnez-moi vous propose une lotte mis il y a pas de mécanisme pour absorber l'inflation sur la construction des commissariats. Voilà nos élus locaux nos mères et nos présidents de départements, s'ils avaient un mécanisme de de reports de charges pour déclencher le paiement sur leur gymnase ou leur piscine. De la même manière, le ministère des Armées, croyez-moi, il serait content. Donc moi je, je le redis, là je pense qu'il y a un contresens à à s'en prendre aux mécanismes des reports de charges, il est bon pour le ministère, si le Parlement veulent supprimer très bien mais je j'expliquerai. Donc on a supprimé quelque chose qui était bon pour les finances du ministère les retards. Monsieur le sénateur, de Lège. Les retards, on ne les souhaite pas monsieur. Monsieur le sénateur, de l'âge, les retards, on ne les souhaite pas mais le charme d'une programmation sur 7 ans. C'est que si on intègre pas déjà les retards. On fera un insincérité par rapport à la copie. Pourquoi ces marges frictionnel existe tout simplement parce que depuis 1960 on a suffisamment de recul sur les différentes programmations. Et donc. J'ai pas envie de prendre cet exemple parce qu'il est malheureux mais s'il peut permettre de nous de nous de nous comprendre. C'est un peu le principe du surbooking, vu la masse des grands programmes, il est évident qu'à chaque. Des fois il y a un coefficient mais à chaque fois il est constaté. Mais pourquoi affaiblir la programmation. Annualité budgétaire, c'est la force de la programmation, c'est comme pour les reports de charges alors privons-nous d'un d'un d'un outil supplémentaire qui est utile pour le ministère des Armées. Mais je suis désolé. Je le ferai pas. Dans Le Figaro à la prochaine fois promis mais je je je je dirais non mais je prends, vous savez quand ça me connaît depuis le temps, mais sur le fond, vous êtes en train de. Non mais sur le fond

pour l'être. À l'alinéa 1 de fait vous n'avez pas modifiée mais alors si Jean, je le dis pour la suite des amendements qui viendront et peut-être aussi pour faire des amendements de correction en séance. Quoi qu'il arrive, même si vous ne partageait pas ma lecture marche frictionnel reports de charges. Le Sénat déjà alourdi la facture avec d'ailleurs des mesures qui sont bonnes mais qu'on ne sait pas payer les 3 milliards de que je parlais tout à l'heure donc. Là je je moi je ne veux plus je disposition, y compris dans un cadre plus informel pour refaire le contour de tout cela. Mais il est clair qu'on est plus à 413 au moment où on se parle, ça je peux vous le signez dès demain et et et pas dans le Figaro et avec beaucoup de bonne foi et et de manière sincère bon quant aux dernières amendement sur au recours, en euros constants. Non. Monsieur le Ministre. euros constants alors c'est c'est c'est c'est très contradictoire en plus avec ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur l'inflation, c'est en clair. On passe d'un schéma ou vous contestez nos hypothèses peut pas contesté mais en tout cas vous émettez un doute une crainte, une crainte sur nos hypothèses en matière d'inflation et en faisant la transaction courant constant vous écarter toute forme d'hypothèses sur l'inflation. Et alors je ne veux pas remuer deuxième fois le couteau dans la pluie, puisque le président Retailleau va définitivement m'en vouloir, mais jadis et vous savez d'où je viens, c'est comme ça que le budget des armées a été diminuée. C'est en faisant euros courant constant comme ça l'inflation venaient grignoter c'est comme ça que le budget global diminue donc le présent Cambon a raison de mettre un avis défavorable à cet amendement parce qu'en fait il vient quoi qu'on en dise cap et l'ensemble. Des efforts c'est pas qu'on rajoute 30.000 en plus c'est tout simplement évacue toute existence de l'inflation dans notre affaire, et là évidemment on on se prend l'ensemble du mur de l'inflation en pleine donc avis défavorable pour cette. Merci, monsieur le Ministre, alors j'ai des explications de vote. J'ai tout d'abord monsieur Perrin.

à l'issue duquel effectivement, j'ai fait un tweet en expliquant qu'à moins de 420 milliards d'euros pour moi et c'est 430 mais je vais me mais c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. À moins de 430 milliards d'euros effectivement pour moi on pouvait pas un modèle d'armée complet j'assume, je l'ai dit, je l'ai écrit et aujourd'hui on a parfaitement conscience que compte tenu de l'état de nos finances publiques, il faut faire des efforts et on veut maintenir ce budget à 413 milliards. Je rappelle que l'origine de tout ça c'est quand même une discussion qui part de 460 milliards d'euros dont on estime que c'est la somme nécessaire pour arriver à un modèle d'armée complet. Bercy voulait 375 milliards. Le président de la République. 400 milliards et vous vous êtes battu, monsieur le ministre, et je le sais pour obtenir le plus possible et vous avez obtenu qu'on est 400. depuis le départ, vous communiquez, vous l'avez fait à à grands frais à grand. Renfort de communication auprès de de l'ensemble des médias sur 413,3 milliards d'euros. si c'est vraiment 413 milliards de. 3 milliards d'euros. Alors il faut les inscrire dans le marbre. Nous ce que l'on veut aujourd'hui, c'est qu'un minimum, on respecte la trajectoire budgétaire. La trajectoire est la cible capacitaire définis dans la loi de programmation militaire de votre prédécesseur madame Parly et on oublie quelque chose d'important dans cette discussion depuis le départ c'est quand même la courbe parce que évidemment on parle de 413 milliards, mais là l'essentiel pour nous, c'est la courbe, c'est-à-dire la capacité qu'on aura dans les années qui viennent à investir 600 millions d'euros de plus que ce que vous avez prévu, c'est-à-dire les 3 milliards et ces trois, ces 600 milliards d'euros nous souhaiterions voir investi ils ont pour objectif de justement d'atteindre cette cible que nous avons voté ici au Sénat à 98% en 2018. Qui consistait à atteindre une cible capacitaire en 2025 et que compte tenu de ce que vous nous annoncez aujourd'hui malgré une augmentation de 40% du budget, on ne risque d'atteindre qu'en 2035. Donc moi je suis évidemment complètement favorable à ce que nous votions cet amendement pour Evo il essentiellement aussi modifier cette trajectoire budgétaire qui je le rappelle fera qu'un euro 2023 n'étant pas un euro 2030 nous pourrons acquérir beaucoup plus de matériel. Merci. Merci Madame Conway Mouret. Oui merci madame la présidente. Madame et. Et Monsieur le le ministre. Moi je ne veux pas du tout entrer dans dans le débat sur le détail du du budget n'y revenir d'ailleurs sur le la démonstration très complexe,

d'utiliser le terme d'économie de guerre. C'est un terme qui est plutôt fort et en même temps vous proposer un effort budgétaire pour plus tard, alors que les besoins en équipement sont maintenant. Donc. Nous comprenons bien évidemment le dilemme de Bercy aujourd'hui qui cherche à faire des économies puisque le ministre. Le maire a annoncé des économies de près de 5% pour l'ensemble des ministères. Mais pour aller dans le sens de l'annonce présidentielle avec une opinion publique aujourd'hui, qui est prête à accepter cet effort assez substantiel en matière de défense. Eh bien nous pensons en effet que il faut voter enfin il faut dépenser cet argent maintenant pour des équipements dont nous avons besoin dans cet effort de guerre. Merci, monsieur le Ministre défini. Vous qui était rentré dans le débat avec 413 milliards. Vous en avez fait une large communication tout le gouvernement et c'était pour discuter de sous la souligné tout cela que l'amendement 66 et 67. Étaient déposés naturellement je vais aller retirer mais ça a permis le débat ça permet en tout cas d'essayer de comprendre, mais je crois que vous parlez. Vous-même de dépassement avec des propositions du Sénat des 413 milliards je pense le quelques amendements que vous avez déposé au nom du gouvernement vont aussi aggraver un peu la facture, mais on y reviendra en cours de, de débats, voilà donc les deux amendements sont retirés. Merci Monsieur Delage. le prof de surbooking, c'est que tout le monde ne rentre pas dans l'avion à la fin ça veut donc bien dire qu'à un moment donné on n'aura pas la totalité de ce que vous avez affiché en terme de capacité à atteindre donc la marge frictionnel. C'est une définition élégante de crédit qui n'existe pas. J'en profite pour retirer. Mon amendement parce que j'ai été plus convaincu par les arguments de Monsieur Cambon que par les votes ne m'en voulez pas. Merci monsieur le président, Laurent. Oui merci madame la présidente, nous nous ne voterons, enfin je ne sais pas combien il en restera l'arrivée nous ne voterons qu'un de ces amendements. Ce que nous n'avons pas envie d'arbitrer ce débat qui est quand même hein. Le bal des hypocrites. Nous avons en vérité, je pense qu'il y a un grand consensus sur la cible de 413 milliards. Mais le gouvernement a du mal à assumer ce choix. Dans le budget. Parce que il y a des arbitrages budgétaires. Compliquées. Qui sont la reconnaissance du fait que il y a un arbitrage politique à faire avec la nation sur la part des richesses disponible que nous sommes capables de consacré. Aux dépenses militaires et le gouvernement a du mal à assumer ce choix. Il y a eu des arbitrages contradictoires, on le sait dans le gouvernement parce que la charge est lourde et elle va peser très lourde, très lourdement. Donc le gouvernement a trouvé un affichage des 413 milliards qui lui permet de passer la rampe dans ces compromis budgétaire et de l'autre côté nous avons une majorité sénatoriale qui s'acharne à sécuriser qui va le faire tout au long du débat. Cette trajectoire. Au nom du fait qu'il ne faut qu'il faut être dans la sincérité et j'en passe et des meilleures. Les même. De la majorité sénatoriale qui dès que nous allons entamer le débat budgétaire redeviendront. Les champions de l'orthodoxie budgétaire et de la lutte contre la dette publique. Et donc qui massacrent auront tous les autres, budget. Après avoir sécurisé, celui-là, hé bien nous sommes en train de passer à côté d'un débat qui mériterait quand même je pense un grand débat politique avec la nation, c'est quelle est la part. des richesses réelles du pays que nous voulons consacrer à ces choix-là mais en même temps que nous voulons consacrer à d'autres priorités nationales tout aussi stratégique, y compris en matière de souveraineté par exemple de souveraineté industrielle par exemple de transition climatique et de souveraineté énergétique. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples mais nous n'avons pas ce panorama noblesse mais donc tout ça en fait en débat, je le répète qu'est quand même un peu le bal des hypocrites nous trancheront pas ce débat. juste pour revenir sur les 413 effectivement le le mais on l'a évoqué des gens en commission le souci du gouvernement, c'est que tout s'est. Organisé.

Bon, une fois qu'on s'est dit ça je rappelle juste. Que en 2017 sur une élection présidentielle. Donc en plus on parle à juste de de 2002 2027 en 2027. Chacun aura corrigé et que de toute façon la loi de programmation des finances publiques aujourd'hui à 17 en 2027. Donc on voit bien que le le sujet qui est devant nous va avant poser problème et c'est vrai que c'est d'ailleurs ce que prédisaient le président du Haut Conseil. Des finances publiques, c'est que tout ça tient jusqu'en 2027, mai 22. 27 à 30, nous rentrons dans une, dans un tunnel sans que personne ne sache exactement ce qu'. Ce sera la trajectoire des finances publiques. Donc j'ai envie dire à Jojo monsieur, le monsieur le ministre, d'autres soucis, nous c'est, il vaut mieux dépenser maintenant pour les programmes. Parce que c'est sécurisé. Il faut dépenser maintenant puisqu'il y a la question de l'inflation et puis il faut dépenser maintenant parce que personne ne connaît réellement et sincèrement la très cher à des finances publiques post-2027. C'est pour ça que, encore une fois nous souhaitons maintenir à ce stade la trajectoire. Et puis il y aura le débat des 7 milliards, mais je crois comme il y aura un débat qui aura essaie de. d'être menée avant la commission mixte paritaire. Je crois qu'on y participera nous aussi avec d'autres groupes et là je crois qu'on arrivera à les uns les autres, a gardé l'essentiel et puis l'accessoire sera mis de côté. Merci Monsieur le Président, Retailleau. on est sur un point dur parce que on on est parti des quatre des 413 milliards, c'est le discours de Mont-de-Marsan du président de la République et le problème c'est les 13 milliards sur les 13 milliards il y en a 5,9 qui ont été sécurisés. Le président Cambon l'très bien dit et on bute sur. 7 4 milliards, c'est que l'autre milliard Monsieur le Ministre, c'est pas pour mettre du matériel neuf dans des hangars rouillés. C'est d'abord pour accroître l'activité opérationnelle de nos armées. Première chose 2ème chose si j'essaie parce que le raisonnement était pas simple, parce qu'il était pas clair. Mais si j'essaie de rentrer dans votre raisonnement reports de charges. Et en même temps marche frictionnel un report de charges. Chers collègues, c'est une dépense différer. Une marge frictionnel. Je me trompe pas c'est un crédit qui ne sera pas consommer. Nous sommes d'accord. Le problème c'est que vous, Monsieur le Ministre, vous comptez aussi bien le report de charges, donc la dépense différé et la marche frictionnel donc le crédit non consommé comme des ressources. Et donc par conséquent le compte ne peut pas y être. Nous ne sommes pas 400 très nous sommes sans doute un peu plus de 400, mais certainement pas quatre très chers collègues et et j'invite. À à ce que le Sénat tienne bon sur cette base là, de l'avenir de nos soldats de nos armées de leur fidélisation et comme le disait à l'instant Dominique Delage. L'image du surbooking. Comme un aveu. Vous avez un avion de 400 places ou surbooké à 413 places. Ah vous n'en ferait rentrer de toute façon que 400 point final donc. Notre point de vue, hé bien le bon j'ajoute encore une fois, Monsieur le Ministre, vraiment, croyez-moi je suis sincère. D'ailleurs vous le savez, je ne vous prends pas en traître. Ces discussions, nous l'avons eu ensemble bien donc. Je, j'essaie d'être dans la vie publique et privée. Voilà, droit. Donc ce que je veux dire par là c'est que les choses pour nous. Nous les avons inscrite à l'annuler à a dit à un de artiste de 3 du restons dans l'enveloppe de 413 milliards. Voilà. Merci. Monsieur le Président Cambon. de la présentation certes excessivement communiquant des 413 milliards. Prenons le problème à l'envers, vous auriez dit 400 milliards budgétés, plus 5 milliards 6 de recettes extra-budgétaires, mais qui sont bien identifiés les sénatrices et les sénateurs sont des gens raisonnables, ils peuvent imaginer que des ressources extra-budgétaires bien identifié. Même si on peut évoquer. Telle ou telle incertitude ou telle ou telle. Prévision un peu généreuse en tous les cas ça nous paraissait il lui fallut dire 405 milliards. Très bien, au moins 405 milliards c'était déjà un effort considérable, c'était plus de 100 milliards par rapport à la précédente LPM et ce sont ces 7 milliards qui dès le premier jour dans les commentaires de la presse dans les commentaires que longtemps ici ou là, créer des suspicions. Alors vous nous parlez des reports de charges moi je vais citer l'exemple de 2008, votre prédécesseur madame Alliot Marie. En 2008, il y a 28% de reports de charges, la nuit l'annuité budgétaire défense va exploser les les industriels dont vous nous dites qu'ils tirent des bénéfices de cette affaire, il était au bord de la dépression se disant. Mais quand va-t-on être payé parce que c'est facile de dire vous serez payé à l'année prochaine et ouvert sera des intérêts mais ce que veut un industriel, c'est généralement quand il livrent matériel c'est de recevoir le paiement qui correspond et donc je pense que le report de charges. On peut l'imaginer, mais pas dans un pour un tel niveau. 7 milliards c'est énorme, et les marges frictionnel tout autant il fallait dans ce cas ne pas en parler et dire la loi de programmation militaire c'est 400 milliards, plus 5 milliards de recettes identifié à ce moment-là. Bon alors. Cédric Perrin aurait dit peut-être plus d'auteurs et dit peut-être moins après chacun se fait son avis mais tout le monde aurait dit il y a un effort vraiment substantiel de plus de 100 milliards et ce serait très bien passé et toute la polémique qui dure. Et liée à ces recettes extra-budgétaires si vous êtes dans enfin ici il y a des gens qui ont été des maires, des conseillers départementaux. Vous l'avez dans le. Lot votre argent, vous l'avez dans le budget, vous l'avez pas si vous l'avez pas, vous pouvez dire effectivement il va m'arriver, j'ai gagné à la loterie, puis je mets cet argent pour le dépenser. Mais elle n'est pas le sens, me semble-t-il d'une loi de programmation militaire qui doit justement justement bien identifié la possibilité de faire ses dépenses parce que, comme ça vient d'être rappelé. C'est pas pour faire c'est pas pour demander des recettes en plus pour le plaisir de vous met en difficulté, c'est parce que le diagnostic de la commission mais il peut être partagé par l'ensemble de cette assemblée, c'est que c'est maintenant qu'il faut de l'entraînement quand des pilotes arrive même pas à faire 160 heures de d'entraînement alors que les normes c'est 220 heures autant que. Et du coup une fiche le camp, et ils vont s'engager chez Transavia. C'est ça le sujet c'est-à-dire il faut fidéliser. Non mais vous voyez je prends exprès des exemples qui permettent de de bien identifier les choses, ne veut plus d'entraînement plus d'entraînement pour notre armée de terre notamment hein on a cité l'exemple des des régiments le des, des. Des, des, de nos blindés Leclerc et cetera donc je crois que il y a un véritable problème dont nous sommes prêts à discuter puisqu'on a jusqu'à la CMP mais je pense qu'il faut que le sénat reste sur cette position s'il n'y a pas une prévision budgétaire stricte ou en tous les cas bien comprise. Il n'y a pas de possibilité de dire qu'on dépensera 413 milliards et ça reste de la communication. Si Monsieur le Ministre.

Après au global, j'ai parfois le sentiment quand même que donner le point au président de la République de l'augmentation des crédits militaires et parfois quelque chose qui est difficile et donc on se cherche à à moins à dire à l'effort, je ne parle pas de vous mais c'est arrivé dans un autre. Mais je je pensais un un hémicycle que j'ai quitté il y a peu de temps sur la même loi mais je, je le dis, Oui. 5 choses. Avec la même bonne foi. Et. Je veux vraiment que ça soit compris hein vous examiner un projet de loi dans lequel dans le rapport annexé. Vous avez 413 milliards d'euros de besoins militaires. Je vais me reprendre d'ailleurs j'y reviendrai ça sera mon point 4. Ce n'est plus vrai où nous sommes en train d'examiner un texte dans lequel nous avons un besoin militaire désormais de 416,2 milliards d'euros puisque la copie a été alourdie, personne n'y est revenu sur ce point mais c'est une réalité qu'il va falloir peut peut être corrigé à moment donné ou alors ça veut dire que le Sénat propose des évictions. Et des renoncements sur certaines autres cibles que vous n'avez pas. je le dis parce que sinon l'ensemble de la cohérence tombe. Ah oui, 3,2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires depuis le début de de de de de l'adoption des amendements en commission. 2ème des choses. Ne tombait pas sur le mot surbooking comme pour emballer rapidement le le le le débat. Monsieur le sénateur, de neige, il y a toujours eu des marges frictionnel dans toute la loi de programmation militaire mal m'en a pris, j'ai voulu par transparence les montrer au Parlement, je dois bien vous avouer que je le regrette un peu, néanmoins je pense quand même que c'est une bonne chose que de le montrer. Et qu'est-ce qui se passe, il y a 2 manières de faire dans cette programmation et c'est pas qu'on espère les retards mais sur 7 ans, il est inévitable que vous aurez un certain nombre de retard et donc ils sont intégrés des gens dans la copie, c'est pour ça que lorsque vous passez de 400 407 ça ne vient pas les écraser, mais ça les additionne. Et dans cette marge frictionnel soit vous l'un intégré en disant je prends 103 pour avoir 100. Ce que d'ailleurs les sénateurs ou le sénateur de votre groupe, ancien ministre de la Défense a pu faire et je revendique cette méthode, c'est une bonne méthode. Soit c'est ce que vous proposez une fine et en disant pour avoir 97 je prends sans. je ne vois pas en quoi le ministère des Armées gagnant dans cette affaire. Donc je revendique de nouveau là c'est c'est de marge sectionnaient elles sont bonnes pour le fonctionnement du ministère sur les reports de charges. La différence avec Michèle Alliot-Marie, en 2008 pardon, d'être cruelle de revenir à 2008 c'est que du report de charges sur des crédits en euros constants avec une diminution forte du format des armées, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour les industriels. Quand vous avez des reports de charges sur beaucoup de commandes pour nos propres besoins mais aussi malheureusement, hélas pour l'Ukraine forcément vous êtes dans un niveau de de de perspectives pour la base industrielle et technologique de défense dans lequel des reports de charges trouvent un intérêt différent d'ailleurs pour avoir suivi de près vos débats jamais les industriels ne se plaignent des reports de charges pour être très clair aujourd'hui, et pour cause. et pour cause, si je veux dire c'est contraire. Je veux dire, c'est bien un sujet qui ne pose pas de problème pour eux, c'est bien ça d'ailleurs au passage si j'étais sénateur dans mon opposition comme dirait l'autre, je dirais quels sont les coûts des reports de charges le caser. Bon et ben je vous réponds aussi puisque je ne suis pas mon propre proposant mais comme l'inflation est forte et ben au fond les gains que vous donne ce report de charges sont bien supérieurs au coût des de de de de ces reports de charges vis-à-vis des industriels et ça je voulais écrit, je l'ai écrit au sénateur de lait, j'en ai fait la démonstration s'ils ne pourront pas se déjuger ont fini par écraser des dispositifs qui sont bons pour le ministère des Armées. Je le regretterai. Mais promis, je ne le ferai plus. Dans Le Figaro 4ème chose. Je reviens quand même. J'ai 3,2 milliards d'euros de dépassement. On se parle. Et cela, puisque vous êtes attentif. À. Dernier point quand même sur les marges frictionnel parce que c'est le président Laurent a raison quand même de de de pointer ça si vous n'intégrait pas les marges frictionnel dans votre programmation vous entraîner en plus des risques d'éviction, soit sur d'autres politiques publiques dans l'état, c'est ce que vous avez dit monsieur le président, dans un autre argumentaire mais néanmoins techniquement c'est pas faux soit évidemment au sein même des éléments de programme pour le ministère des Armées. Je voulais aussi rajouter cet argument-là qui me semble important aussi dans la logique où vous allez regarder la LPFP Non, là on a 3,2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Je je je le redis qui sont non documentés pour le coup par le Sénat qui fait que on est pas à 400, 407 ou 413 de toute façon on est à 416 2. Et que pour le coup, puisque j'ai entendu le président Retailleau au nom de sa majorité. Dire

de c'est facile à comprendre pour le coup, le raisonnement est implacable. Si vous rajoutez du MCO, ce qui n'est pas le même débat que les marches et marche était de dire, Monsieur le Ministre conversation que nous avons eu tous les deux. Il y a des choses ça nous semble urgent de le faire dès maintenant des 24 est pas attends de 27 28 mais c'était dans les 413 ou dans les 400 comme vous voulez, d'ailleurs. Là c'est autre chose. Vous rajoutez des cibles nouvelles et des choses nouvelles, vous les glissez pas de 27 30 vert. 24 27. Sur 24 30, vous rajoutez des choses et ça pour le coup c'est pas documenté ce pas financé et si vous restez dans l'enveloppe globale. Ça veut donc dire qu'il y a des renoncements. À 3,2 milliards d'euros c'est beaucoup d'argent et donc ça veut dire qu'il y a des renoncements quelque part en tout cas moi je. Merci pour l'échange et de débat parce que ce que j'ai entendu surtout c'est que personne ne veut aller au-delà des 413 milliards d'euros. Ça je pense que c'est la clarté du débat et l'honnêteté me commande de le dire, ça veut dire que je renvoie à d'autres à d'autres cadres et d'autres formats, le fait de pouvoir nous accorder. Merci. Alors je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement numéro 100 282 avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contraint qui s'abstient. Il n'est pas adopté. L'amendement 148. Monsieur le président, Laurent. Oui merci madame la présidente. C'est un amendement qui vise à supprimer le membre de phrase qui a été rajouté. Dont le travail parlementaire visant à à dire que les chiffres que nous qui sont maintenant sécurisée par la nouvelle trajectoire adopté s'entendent comme un minimum. d'abord. Les chiffres sont sécurisés. Par par le nouveau tableau. Ces chiffres en plus si on veut vraiment avoir une idée de l'ensemble de nos dépenses militaires ils sont supérieurs puisque on sait qu'il y a une série de dépenses notamment les dépenses pour l'Ukraine et d'autres. Je ne refait pas la liste qui a fait le ministre lui-même tout à l'heure, qui ne rentre pas dans cette enveloppe, donc on est au-delà de 413 milliards de dépenses militaires et on rajoute cette phrase alors que déjà on sécurise tout. Je pense que cette phrase introduit une ambiguïté. Alors je sais que certains la en disant. Ben on continue de sécuriser au minimum mais on peut la lire autrement c'est de dire que c'est un minimum donc qui est appelé à augmenter encore au-delà de, de ces chiffres. nous nous sommes pour supprimer cette ambiguïté et supprimer cette phrase qui n'ajoutant rien en fait. Une fois que les chiffres sont sécurisés par le tableau. Nouvellement adoptés. que la ligne A que cet amendement propose de supprimer, avait été en fait introduit par le rapporteur de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Il s'agit de dire que la la trajectoire de ressources budgétaires est un minimum. C'est le ministre avait affirmé à plusieurs fois devant les commissions que les marches proposé était démarche plancher et non des marges plafond et compte tenu de, de nos finances, ces dispositions n'est peut-être pas très opérante mais étant donné à la fois les incertitudes et le jeu de l'inflation sur la situation géostratégique la précision qui a été introduite nous semble opportune. Donc c'est un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement. C'est le nouveau oui madame la présidente, même raisonnement donc même avis défavorable. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement 148 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est donc pas adoptée le 191 monsieur le président Gontard. madame la madame la présidente. Cet amendement un amendement qui vise à garantir le financement de la LPM par le recours à des nouvelles recettes. Les écologistes sont favorables aux projections budgétaires des quatre lois de programmation examiné par le Parlement. Ces 2 dernières années, l'aide publique au développement, le ministère de l'Intérieur, ministère de la justice qui permettent de renforcer les moyens des pouvoirs publics de donner de la visibilité de programmer des investissements pluriannuels et d'une manière générale, nous sommes favorables au renforcement des moyens de la puissance publique. En d'autres circonstances, les écologistes profondément pacifiste pacifiste n'aurait sans doute pas approuver une augmentation aussi massive des moyens de la défense. Mais la démocratie est plus que jamais menacée à l'Est de l'Europe et le soutien indéfectible à l'Ukraine justifie à nos yeux les efforts militaires auxquels la nation consent toutefois avec cet amendement, nous voulons nous assurer que les dépenses financières conséquentes prévues par la loi de programmation militaire n'empiète pas sur celle des autres missions du budget général tels que l'éducation par exemple la santé, le risque est en effet que la conjugaison des programmations budgétaires ambitieuses s'agissant notamment des missions régaliennes de l'État. Également du dogmatisme de votre gouvernement qui refuse de faire contribuer les plus aisés à l'effort collectif ainsi que votre promesse irréaliste et discutable de rétablir le déficit budgétaire sous les 3% entraîne mécaniquement le risque de faire peser l'effort financier proposé par la LPM sur les autres missions du budget de l'État. Je l'ai dit l'éducation nationale, la santé, la transition et le la culture vous nous le préciserez peut être en tout cas ce n'est pas acceptable donc le présent amendement vise donc à garantir hein. Finissement de la LPM assurée par de nouvelles recettes et non des transferts de crédits, susceptible d'affaiblir des services publics déjà amoindri ou d'amputer nos ambitions en matière de transition écologique. Merci. Si l'avis de la commission, monsieur le président. Madame la présidente. C'est c'est un raisonnement que l'on ne peut pas reprendre à notre compte puisqu'il tend à opposer. Les forces de défense aux autres missions du budget de l'État. Je rappelle que l'effort de défense et moins de 2% du budget, les dépenses sociales, c'est plus de 30%, donc bien évidemment c'est un, un, un raisonnement qui ne correspond pas à notre approche de ces sujets. Par ailleurs l'effort de défense est un formidable accélérateur. Économique un euro investi. Dans l'industrie de défense rapporte 2 fois plus à l'économie au bout de 10 ans, donc bien évidemment, c'est un avis défavorable.

comme parfois sur les réseaux sociaux. Ça se dit. Je pense qu'opposer les les différents pans du budget de l'État. Les uns aux autres, sont toujours très délicat et très difficile. Donc je pense que ça a ses limites de ça pose la question plus globale de la soutenabilité je pas revenir à la LPFP et cetera mais il est évident que la trajectoire initiale que nous proposons. Elle ne crée pas d'effet d'éviction sur les autres programmes puisqu'elle a été imaginée et conçue comme telle avec Bercy, ça c'est une réalité d'où les longs débats sur 413 et suivants je recommence pas parce que pour le coup là inévitablement à un moment donné, on commence à avoir une difficulté en tout cas l'avis défavorable. Merci alors je. Oui, monsieur le président Gontard. pour, pour répondre au président quand bon c'est vrai que j'ai j'ai déjà pas opposer les les Budgets au contraire, je m'en suis bien. Préservé. J'ai même dit que le budget et les prévisions qui étaient là étaient importantes et dans le contexte actuel, au contraire je demandais juste et et cet amendement précise justement où est-ce qu'en gros on va prendre cet argent et. Et effectivement ça, ça aura forcément un impact sur l'ensemble des autres Budgets et c'est toute la problématique. De fait, d'un, d'avoir un budget dédié sur sur la la question de de l'armée. On, on a quand même cette problématique-là et ça pose quand même avec le nombre de budget qui se qui se, qui s'interpose comme ça et et qui s'additionnent. Au bout du compte quelles seront les autres les autres secteurs qui seront qui seront impactées ou alors quelles ressources. Le ministre il peut nous apporter pour justement. Apporter ces nouvelles ressources. Merci monsieur le président, Laurent. je partage ce que vient de dire le président Gontard et j'ajoute que si on voulait pas. Organiser mettre en opposition des Budgets comme vous le dites, Monsieur le Ministre. Encore faudrait-il ne pas réserver la la programmation budgétaire à certains Budgets et pas à d'autres. Je prends 2 exemples très rapidement, nous avons eu ici, on débat pendant. De longs mois, une loi dite de programmation. De l'aide au développement, dont la grande caractéristique et qu'elle n'a jamais été une loi de programmation budgétaire. Puisque toute programmation budgétaire sérieuse nous a été refusé. Dans ce débat budgétaire donc là par exemple nous ne savons pas comment ça va évoluer. 2ème exemple dans tout un tas de domaines de la transition écologique. J'en prends un par exemple, il n'y aura aucune reconquête du ferroviaire français dans le domaine du fret sans une réelle programmation budgétaire. Il n'y en a aucune. Donc si on veut lever ce type de débat et sécuriser les choses à ce moment-là, il faut avoir une vision de la programmation budgétaire qui ne se réduisent pas uniquement au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense. Il faut avoir un débat plus large sur ces questions et à ce moment-là on pourra discuter des arbitrages réels qui sont rendus mais là en vérité les Budgets ne sont pas à égalité, même quand il s'agit de budget stratégique et même quand il s'agit de budget qui ont besoin de la programmation sur longue période. Merci. Alors je mets aux voix donc l'amendement 191 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient et donc pas adopté l'amendement 192 président Gontard. madame, madame la présidente. L'amendement que nous proposons a été travaillé avec Icahn France qui est le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires et il vise à s'assurer que l'investissement dans la dissuasion nucléaire ne dépasse pas 13% du montant global de la LPM. La dissuasion nucléaire représente selon les mots exprimé à plusieurs reprises par monsieur le le ministre 13% du montant global de la LPM, soit 53,69 milliards d'euros. Nulle part. Pourtant dans cette loi ce montant ou même ce pourcentage est inscrit contrairement aux dépenses liées aux dépenses liées à de très nombreux Bram d'armement et contrairement aux précédentes LPM. Il est donc nécessaire de maîtriser les dépenses en matière de dissuasion nucléaire pour ne pas pénaliser les autres programmes et objectif de cette LPM. Certes, notre modèle d'armée repose largement sur la dissuasion qui peut contribuer à préserver la stabilité et à éviter les conflits majeurs entre les États dotés de l'arme nucléaire et peut constituer un moyen essentiel de garantir la sécurité nationale et de protéger les intérêts vitaux. Mais d'une d'une l'effort en matière de dissuasion grève largement d'autres efforts notamment en matière de renforcement des moyens de notre armée de terre et contribue largement échantillonnage de notre armée et de de la dissuasion ne nous évite pas un conflit militaire indirect avec une puissance nucléaire. Et nous nous permet pas de faire l'économie d'un armement conventionnel. Enfin un surinvestissement ce domaine pourrait nous conduire au delà de la doctrine de stricte suffisance et créer une spirale dangereuse de prolifération nucléaire. Pour toutes ces raisons, il nous apparaît indispensable de plafonner les dépenses relatives à la dissuasion nucléaire pour s'assurer qu'elles respectent les engagements de la France et pour ne pas qu'elle morte sur le reste des besoins de l'armée. Merci. Merci l'avis de la commission, monsieur le président. dans le travail de la commission de de de revenir sur ce point, néanmoins la rédaction de cet amendement n'est pas acceptable et je dirais que par les temps que nous connaissons de très grande menace, tout ce qui concerne à la fois le renouvellement et la modernisation de notre dissuasion nucléaire qui est notre assurance ultime ne peut pas être négligée. Donc c'est un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Bon avis, avis défavorable. Pierre Messmer avait une très jolie formule il disait à propos de la dissuasion nucléaire dans les dans les textes financiers, économiques et financiers enfin budgétaire un certain secret militaire, il fallait aussi y adjoindre une forme de discrétion budgétaire. Et de fait. Pour désormais de l'autre côté de la barrière, la structuration même des crédits. Il y a la dissuasion disent des choses sur notre dissuasion. Voilà

donner un peu plus de transparence sur la dissuasion nucléaire très vite vous donner à voir au contenu des programmes de modernisation et en fonction de ce que vous dites sur le degré de modernisation de la dissuasion, vous envoyez donc aussi autant donner directement un certain nombre de secrets à nos compétiteurs. C'est ce qui explique. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Président.

J'ai regardé ce qui était communicables au Parlement, j'ai dit 13% après vous faites un amendement pour expliquer faut capé à 13% je vous explique que non, déjà pour des raisons de détail mais je pourrais aussi dire et si ça faisait 15%. En quoi ça serait grave après on revient à un débat de fond, vous êtes contre la dissuasion. Ce que je respecte mais je ne partage pas. la. À la question. Pourquoi je donne un chiffre, parce que vous m'avez posé la question. Alors je peux vous aussi vous dire pourquoi vous avez pris mon film dans un amendement pour le cap et donc voilà, donc c'est un peu sans fin, c'est la poule et l'oeuf. En tout cas la dissuasion, c'est la clé de voûte de notre défense pour la protection de nos intérêts vitaux et comme vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois en commission mais je le redis ici, vous avez tous les 20 ou 25 ans, des efforts de modernisation qui sont un cap sur par exemple SNLE ou sur les avions ou sur les missiles ou sur d'autres aspects, plus critique, qui tiennent évidemment tête et que donc, par définition, vous avez des pics et ça je m'en étais aussi expliquer par rapport à la chronique budgétaire qui fait que la dissuasion va connaître énormément de modernisation entre 2028 29 jusqu'en 2035. Je forme le voeu que les majorités qui viendront et les président de la République qui suivront défendront la dissuasion nucléaire mais parce qu'en fait, entre le moment où vous décidez un programme et le moment où il s'exécute en crédits de paiement ça prend du temps. on vit sous l'empire de la dissuasion globalement décidée par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Vous avez inertie très très forte évidemment que vous retrouvez aussi sur les crédits de paiement c'est aussi évidemment c'est quelque chose qui est propre à ce modèle. Merci alors je mets. Aux voix l'amendement 192 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté l'amendement 237 du gouvernement, Monsieur le Ministre défendu. Merci l'avis de la commission, monsieur le président. La commission aura un avis défavorable. Parce que cet amendement vise. Par ses explications laconiques il a supprimé un excellent amendement du sénateur de Lège, rapporteur de la commission des finances. Qui vise les cas où la France procède à des cessions de matériels militaires à d'autres pays, c'est-à-dire des exportations de matériel d'occasion. La moindre des choses c'est quand on cède un Rafale à la Grèce ou à la Croatie ou d'autres pays car nous sommes tous toujours plutôt favorable. Il convient de le remplacer et pour le remplacer. Si vous touchez le produit d'un d'une vente d'occasion. Vous êtes obligés de compléter, pour acheter un avion 9 on achète pas d'avions d'occasion. Donc je pense que l'amendement de Dominique, de lait, j'étais un amendement tout à fait est important et donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre, à votre amendement. Merci alors je mets aux voix donc l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission, c'est l'amendement 237 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils ne vont pas adopté 2 amendements en discussion commune le 149 monsieur le président, Laurent. c'est c'est un amendement d'appel et je vais m'adresser aux particuliers à Monsieur le Ministre, enfin ou Madame la Ministre. Puisque la commission a pris la peine de préciser dans cette. Phrase rajoutée que. Le la LPM 2 financerait en aucun cas le service national universel, c'est la première fois dans le texte qui les mentions du. Du service national universel et on retrouvera cette référence à différents endroits du texte. Donc la question moi que je pose, parce qu'on a eu des versions différentes. La dernière en date c'est l'interview que vous avez donné. Dans Le Figaro. mais on a eu plusieurs versions de. De ce dispositif et on ne comprend toujours pas explicitement qu'elle quel est son lien à la loi de programmation militaire, puisqu'il figure à plusieurs endroits de ce texte. Donc y a-t-il un lien entre le SNU et la loi de programmation militaire. Lequel. Parce que sinon on ne voit pas pourquoi ce dispositif figure. D'une manière ou d'une autre dans le projet de loi. Quel est ce dispositif. Est-ce que c'est un dispositif de formation militaire qui va s'adresser, puisque c'est lundi le dernier dispositif annoncé à des jeunes de 14 ans pendant des séjours de 12 jours sur le temps scolaire. Si ça n'est pas le cas. Quel est son rapport avec la loi de programmation militaire nous on veut comprendre quelle est la nature de ce dispositif et je le répète, pas seulement en général mais dans son lien à la loi de programmation militaire. Sinon toute référence au SNU n'a rien à y faire, d'autant plus que la commission dit. La la LPM ne financera en aucun cas le le SNU. Si l'amendement 194 monsieur le président Gontard.

sur la question du du SNU. Effectivement, il est dans cette, dans cette LPM et il apparaît dans cette thèmes MPM et donc il nous paraissait important de préciser. Puisque l'objectif de ça, du moment et de clarifier que le service national universel SNU restera entièrement volontaire puisqu'il ne peut être établi sous la contrainte car le lien entre la nation et l'armée doit continuer à être fondée sur un engagement volontaire et donc pour lever toute ambiguïté, il est proposé de le dénommé service national ça nous paraît aussi aller dans le sens. De Madame la Ministre qui nous avait indiqué que le service national universel était justement volontaire et donc comme il est inscrit dans ce texte autant préciser justement son comme son caractère. Volontaire. Merci l'avis de la commission, monsieur le président. Merci madame la présidente. C'est une position constante de la commission de d'avoir dit depuis que le projet de SNU Madame la Ministre et a été lancée par le président de la République avec l'intérêt que le Sénat peut bien évidemment y porter mais c'est une position constante de la commission de dire que le SNU ne peut pas être financé par la LPM je prends juste un exemple, si nous étions en année pleine pour une classe d'âge c'est une dépense de l'Ordre de 3 milliards. Alors vous voyez ce les conséquences que ça. Oui donc, bien évidemment c'était un, un avis défavorable sur l'amendement de notre collègue Pierre Laurent. Hé bien évidemment en ce qui concerne la transformation du SNU en service volontaire là aussi la la loi de programmation militaire n'est absolument pas le bon véhicule pour débat du SNU. Nous sommes à la disposition de la ministre. Je suis heureux qu'elle soit ici pour l'entendre et pour développer ce projet. R si si l'avis du gouvernement. Madame la Ministre. Merci beaucoup madame la présidente, monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs pour faire peut être un point assez. Assez globale sur le service national universel aujourd'hui le projet est totalement volontaire il a si demain la modalité devait changer évidemment ce serait avec une proposition avec un projet de loi qui devrait être débattue évidemment dans nos, dans les deux chambres et ce serait évidemment votre décision définitive qui devrait l'emporter pour apporter de la clarté sur le nouveau projet du service national universel sur le temps scolaire. Ça c'est le projet volontaire d'établissement et de classe qui choisissent la forme d'engagement en réalité notion pédagogique plus que nécessaire. Pourquoi le service national universel et cité dans le rapport annexé dans la forme du texte présenté par le gouvernement pour une raison toute simple, il y a dans le service national universel dans son ADN même et dans son projet pédagogique. Le renforcement du civisme de la citoyenneté et en réalité également du lien armée jeunesse puisque il y a la journée défense mémoire qui, évidemment, vous le savez, est présenté par un certain nombre. Hé bien de nos armées puisque elle est portée par la direction. L'ADSL J. la direction de la jeunesse du ministère des Armées. Au-delà de ça, évidemment il y a la phase de puisque nous parlions là de exclusivement du séjour de cohésion. Donc la phase d'internat et le séjour volontaire d'engagement des jeunes qui a la mission d'intérêt général peut prendre plusieurs formes. Et vous, vous en connaissez un certain nombre, les cadets de la gendarmerie. Les escadrilles hier jeunesse ou encore des engagements civil ça peut être service civique. Engagement associatif dans un Epad hé bien divers engagements donc pour répondre à votre, à votre question. La réalité c'est que non, il n'y a pas de financement dans le cadre de la LPM et nous nous sommes totalement en phase avec le président de la commission qui a apporté une une réponse extrêmement clair. Donc c'est un avis défavorable pour les amendements 149 monsieur le président et l'amendement monsieur le présent 194 également, remercié. Monsieur le président, Laurent. Le. Oui, moi je voudrais m'associer aux remarques de mes 2 collègues qui d'ailleurs disent que ce sont des amendements d'appel, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dans l'article 3 alinéa 10 ans la première partie c'est-à-dire ce qu'a répété le président quand bon tout à l'heure les ressources ne comprennent pas le financement du SNU. Mais ce que je ne comprends plus et que Suède SNU. Il est inscrit va disposer de financements Haddock. Mais qu'est-ce que c'est des financements où allez-vous trouver ces financements Haddock. Autre chose, excusez-moi, vous allez dire que je pose des Budgets de l'État. J'espère que ce ne sont pas des financements liés à l'éducation nationale, parce que ça avait été évoqué et parce que Madame la Ministre vos propos diverses et variées à travers la presse nous inquiète et ne nous rassure pas du tout sur ce point. Vous parlez de prendre le SNU sur le temps scolaire. Vous dites que les voyages scolaires vont être assimilés enfin c'est à peu près la même chose donc je n'oppose pas des Budgets. Je veux simplement vous dire notre inquiétude et vous dire aussi que ce passage en force du SNU sans faire le bilan de quoique ce soit nous exaspère beaucoup. Merci sur le président Laurent. sérieux et d'ailleurs nous avons fait adopter un amendement qui a été retenu par la commission. Pour appeler à ce débat national, mais les formules actuelles qui sont avancés les unes après les autres du SNU ne répondent pas à cette question, hein, et ne peuvent pas s'adresser qu'à des jeunes de 14 ans en seconde. Donc nous avons besoin d'un débat national sur cette question, qui n'existe pas pour le moment et ça fait des années que la question est posée la question du volontariat. Elle est toujours pas réglé. J'entends ce que vous dites mais c'est le volontariat de qui, des établissements. De professeurs avec leur classe, des élèves et de leurs parents, parce que là on parle d'enfants de 14 secondes hein 13, 14 15 ans. Donc il est volontaire, c'est, ça n'est pas clair. Et comme en plus, il s'agit d'une période de 12 jours sur ton scolaire donc on ne parle pas d'un d'un problème mineur dont le parcours scolaire des enfants, surtout à cet âge-là. Donc je pense que le dispositif n'est pas clair. nécessaire sur le lien armée jeunesse fait défaut et il faudra l'ouvrir un jour de manière sérieuse et transparente avec le pays. Et enfin je retiens je vais retirer mon amendement parce que je suis d'accord avec la formule c'était je l'ai dit un amendement d'appel la LPM n'a pas à financer en l'état le SNU. Mais ça veut dire que nous devrons retirer le SNU par exemple quand il figure dans des énumérations plus tard dans la loi, au même titre que la réserve opérationnelle. Monsieur le président. Non. Non. Rapidement parce que je rejoins tout ce qu'il a tout ce qui a été dit mais c'est vrai que sur le SNU en fait beaucoup de choses sont dites hein et on vous écoute sur à la fois son son organisation. Le fait qu'ils soient volontaires et cetera mais rien n'est jamais inscrit quoi et donc à un moment donné il va peut-être falloir préciser là on vous en donne l'occasion en tout cas sur l'aspect volontaire, vous nous dites que c'est volontaire. S'il est inscrit dans la loi et ben autant inscrire très clairement qu'il est volontaire. Et puis c'est vrai que si on nous dit qu'il ne doit pas être dans la loi. Ben en tout cas il faut le faire, il faut le qu'on puisse l'enlever. En tout cas de toutes. Et les les mentions qui peuvent être faire tout au long de de ce texte.

en réalité ce sur la base du volontariat. Aujourd'hui, c'est demain, ça devait évoluer, il y aurait un débat, un débat parlementaire et madame la sénatrice pour vous rassurer, le budget du service national universel est un budget autonome qui ne touche ni à l'Éducation nationale, ni aux armées, c'est un budget qui est une ligne qui s'appelle la 163 c'est jeunesse vie associative et en réalité, son budget a toujours été autonome puisque j'ai été moi-même parlementaire quand il a été créé, il en avait la charge et j'avais une seule inquiétude et tout à fait légitime, c'était que ça vienne piocher dans d'autres Budgets que cela affaiblisse d'autres projets jeunesse et c'est pour ça qu'elle est sanctuarisé, elle a augmenté proportionnellement aux engagements et peut être monsieur le sénateur, pour compléter. Aujourd'hui, le SNU continue à évoluer bien sûr mais il a trouvé une, il a trouvé en tout cas une aspiration au sein de la jeunesse. Il y a plus d'. Ministre qui a la parole. Et pour conclure et revenir sur les propos essentiel. Aujourd'hui, le projet n'est n'a pas vocation à être débattue dans la LPM mais je suis à la disposition des parlementaires évidemment et des sénateurs pour entrer dans le détail du projet. Merci alors je mets aux voix l'amendement 194 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient et donc pas adoptée, je mets voix l'article 3 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est donc adopté. Alors après l'article 3 L'amendement 69 Monsieur Féraud. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Si nous avons choisi avec. Décidé avec. Collègues du groupe. Socialiste de présenter cet amendement, c'est parce que. Dans. La discussion de cette LPM. Il ne nous paraît pas possible de discuter exclusivement des dépenses sans aborder aussi la question des recettes. On le voit d'ailleurs bien avec l'ensemble du débat que nous venons d'avoir sur report de charges marge frictionnel la réalité des moyens que nous nous donnons et donc nous avons proposé un amendement pour lever des recettes supplémentaires afin de financer les investissements et les dépenses considérables dont nous avons besoin pour protéger notre pays nos compatriotes dans les années qui viennent, qui concerne la loi de programmation militaire. Je pense qu'il y a d'ailleurs là un vrai parallèle avec les travaux, notamment, de Jean Pisani-Ferry sur le financement de la transition énergétique, comment nous le finançons comment nous faisons en sorte que ce financement pèse de manière raisonnable sur la dette publique que le financement soit socialement juste. Donc notre amendement propose. De lever une taxe sur les placements d'assurance-vie à partir d'un certain montant pour que cela ne pèse pas sur la la classe moyenne ou les classes populaires. Si le dispositif d'ailleurs ne me paraît pas pertinent à la majorité sénatoriale ou au gouvernement, il en existe d'autres possibles sur le Patrimoine. On s'est battu en vain ces derniers mois pour une taxe sur les superprofits. Nous sommes toujours favorables à des dispositifs de cette nature qui permettent de. Trouver les financements nécessaires au considérables dépenses publiques dont nous avons besoin. Donc voilà, nous avons voulu élargir le débat sur la LPM avec cet amendement, en parlant des recettes nécessaires pour les dépenses. J'espère que cela pourra intéresser notre assemblée quelques si l'avis de la commission, monsieur le président. Président hein présidente cet amendement vise simplement à augmenter la pression fiscale sur les ménages. Avec cette originalité c'est que. Il n'est pas précisé qu'ils financent les dépenses militaires donc c'est évidemment un avis tout à fait négatif. Merci

Prises de parole de monsieur Olivier si le de Gaulle dit. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à ce stade de la discussion, nous souhaitons apporter de point de précision avant l'examen de l'article 4 et les deux amendements du gouvernement. Nous avons modifié en commission cet article pour prévoir que le financement interministériel des surcoûts liés aux OPEX et aux missions intérieur ne souffrirait pas d'exceptions liées, je cite, à des circonstances exceptionnelles qui justifieraient que la mission Défense contribue au-delà de sa proportion dans le budget de l'État. Cela ne nous paraît pas judicieux. Monsieur le Ministre vous demander un effort qui est volontiers qualifiée d'historique à la nation. Cet effort et est là pour préparer notre ou nos troupes à la haute intensité et à l'engagement majeur pouvoir constituer une poire pour la soif. Dans un contexte budgétaire déjà dégradé et enfin 2ème point à cet article. Nous avons également ajouté la présentation annuelle par vous, Monsieur le Ministre du bilan détaillé des OPEX. Et d'missions intérieur il sera leur temps de débat de la contribution de la mission Défense à leur financement. Merci. Merci. Alors passons à l'amendement 238 monsieur le ministre. Un amendement du gouvernement. Monsieur le Ministre, pardonnez-moi, voilà la présidente je je me je suis distrait. Le 200. Les deux sont défendus. J'insisterai bien volontiers sur le 238 pour essayer de, de comprendre sur le je reviens pas sur circonstances exceptionnelles bon sur les JO. C'est un amendement au fond qui est un amendement d'appel pour comprendre ce que vous avez vous souhaité faire en, en, en commission, structure évidemment OPEX et ce qu'on appelle mi-sainte mission intérieur. Mais je suis intérieur évidemment sentinelle. On y reviendra plus tard évidemment harpies. Parce qu'on dit sur le territoire national et c'est pas une mission facile pour les forces armées on pourra être revenir et puis il y a une mission. Ponctuelle spécifique aux forces armées, que sont les Jeux olympiques sur des missions qui sont celles des forces armées. Posture permanente. De sûreté de l'espace aérien lutte anti-drone. Renforcement de la sécurité d'un certain nombre d'emprises militaires dans Paris pour soulager les forces de sécurité intérieure mais on reste dans le cadre. Et donc la copie que je vous avez présenté initialement. Hein. Évidemment, prenez en en compte ce que le ministère des Armées doit pour le volet. JO, ce qui a été documenté par les états majors et qui nous semble sincère. Bon ça a été raboté un tout petit peu en commission, je sais pas pour quelle raison parce que, au fond, il y a deux cas de figure. Enfin non il y a 2 éléments d'information. Vous devez avoir en tête le 1er c'est que le chiffre est telle qu'il est présenté, il correspond bien à des missions militaires sur les jeux. Sur les Donc c'est logique de faire de mettre une provision pour se faire et s'il veut inquiétude c'est que y'un dépassement. On est bien dans ce tableau dans les logiques de et donc c'était évidemment le financement interministériel qui seraient sollicités. Si nous devions aller au-delà de la provision. Donc j'insiste peut-être plus lourdement. Même si je sais que les avis des commissions sont déjà faits enfin je je je je prône le rétablissement de la provision initiale parce qu'en terme de sincérité budgétaire, elle correspond à l'argent qui est documenté par les États-Majors pour réussir les missions qui lui sont dévolues aux forces armées sur sur les Jeux olympiques 239. Vous êtes revenu, il est défendu. Merci. L'avis de la commission, monsieur le président. Sur ces deux amendements. qui avait été votée par nos collègues socialistes qui a été adopté en commission et qui prévoyait que le financement des Jeux olympiques était exclusivement inter-ministériel et ne s'imputer donc pas la provision annuelle au titre des OPEX et des missiles. C'est ce qui avait conduit, Monsieur le Ministre à la diminution de 50 millions d'euros. Alors nous sommes tout à fait d'accord pour que les militaires participent à la sécurisation du territoire pendant les Jeux olympiques, on est un petit peu moins d'accord pour que le ministère des films désarmer finance intégralement cette dépense. Et donc c'est pour ça que nous donnons un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Avis défavorable aussi sur le 239 sur la réintroduction de la possibilité d'une contribution plus que proportionnelle de la mission Défense pour les mêmes raisons. Donc. Il n'est pas question de revenir sur le principe qu'on a évoqué, avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. c'est le. Vous voyez ma tristesse à ne pas avoir été, avec vous en commission pour pouvoir expliquer les choses. Et. Oh ben m'écouter n'est pas une infraction à la séparation des pouvoirs. Non sur le 238 de bonne foi les provisions telles qu'elles sont construites sont bien sûr les missions militaires. Lutte anti-drone, c'est le boulot des forces armées, l'armée de l'air en l'espèce. La posture permanente dans le ciel qu'on va durcir pendant les JO. Et donc il est logique, enfin on, on sera en insincérité budgétaire. Si on ne l'avait. et là vous l'avez diminué un peu mais en fait. Mais en fait. C'est normal de prendre sur la la la part qui correspond à à l'activité des forces en temps normal, enfin ça ne viendrait pas à l'esprit de rebasculer l'ensemble de la posture permanente de sûreté du ciel en interministériel. Enfin, le système fonctionne parce que le président Madame la présidente, il il il est fait de telle sorte ou si ça dépasse, ça ça part en en interministériel. Mais il faut quand même que ça corresponde à la réalité des missions militaires tels qu'on les imagine en tout cas là je trouve qu'on va abîmer un tout petit peu la la la structure des choses pour 2024. Je tiens vraiment à le dire pour le, pour le Sénat. En revanche, je m'engage. Si on devait avoir des éléments. Qui serait nouveau dans ce qu'on demanderait aux forces armées pour les JO. Bon il est évident que là, on repart en interministériel. Voilà je voulais quand même le dire parce que c'est un point important me semble-t-il. Merci. Alors je vais mettre aux voix donc l'amendement 238 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre un qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'amendement 239. Même avis même vote. aux voix l'article 4 qui est pour. Contre qui s'abstient. Il est donc adopté à l'article 5. Monsieur Olivier Cigolotti a demandé la parole. Monsieur le Ministre, nous on l'a abordé dans cet article 5. La problématique des carburants opérationnels. Nous avons souhaité ajouter le même type de garantie. Si les cours chutent en dessous de 85 dollars par baril cours utilisé comme hypothèse de construction de la LPM, hé bien la mission Défense ne sera pas fonctionner ceci vise à ce que. Un pari à la baisse ne soit pas tenté en gestion et qu'ainsi Nigel ni mise en réserve ne puissent être décidé sur la base d'une prévision baissière des cours des énergies opérationnel des à-coups qui seraient générés nuirait grandement à notre sens à la bonne exécution de cette LPM Merci. Alors l'amendement 195. Président Gontard. Et qu'un rapport soit remis au Parlement sur les moyens pour nos armées de limiter leur consommation de carburant. Plus précisément, nous souhaitons que ce rapport inclut également une réflexion sur les possibilités de rationalisation de l'utilisation de carburant en dehors de théâtres d'opération mais aussi sur les possibilités d'éco-conception d'équipements militaires, notamment des véhicules. L'armée possède beaucoup d'équipements très polluant. Si elle a longtemps été exempté de tout objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, il lui faut aujourd'hui prendre sa part à l'effort national lorsque le contexte le permet. Mais c'est aussi un enjeu stratégique important la dépendance de nos armées aux énergies fossiles, pose des questions sur la capacité de nos armées à opérer efficacement la fluctuation des prix du pétrole et d'autres les énergies fossiles, ainsi que leur déclin prévisible à long terme est une problématique. Il faut à tout prix prendre au sérieux. De plus, c'est un enjeu financier nos armées dépense près d'un milliard d'euros en carburant soit aujourd'hui plus de 2% de leur budget. La volatilité des prix du carburant, faisant peser une incertitude sur notamment la trajectoire même de cette LPM. Face, donc à un environnement énergétique en constante évolution. Il nous faut renforcer la durabilité et la résilience de nos armées. Il ne s'agit pas ici de contraindre les militaires sur un théâtre d'opération mais bien de réfléchir à une nouvelle génération de véhicules qui en ne consommant pas ou peu de carburant fossile pourrait gagner en durée de route de vol et en capacité opérationnelle il ça aussi sans contrainte excessive de porter une attention accrue à l'économie des carburants en dehors des théâtres d'opérations qu'il s'agisse de la logistique militaire ou des exercices donc nécessaire de réaffirmer notre engagement pour la transition vers une économie à faible émission de carbone. Non seulement pour lutter contre le changement climatique mais également pour garantir notre sécurité et notre dépendance. Madame la présidente, tout ce qui concourt à diminuer l'empreinte carbone de nos activités militaires va dans le bon sens et ce rapport viendra effectivement étayer les travaux qui sont faits dans ce domaine la Commission et demi à il a émis un avis favorable. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui merci mais à présent il y a le fond et la forme, sur le fond. Évidemment, ça va dans le bon sens. Sur la forme demandées aux armées de produire un rapport uniquement sur ce sujet. Me semble. On va dire. Non mais c'est un homme fichu, sauf que vous avez par ailleurs adopté sous le contrôle du président. Évidemment le bilan annuel de la LPM à l'article 8. Donc moi ce que je vous propose, c'est juste une affaire de méthode. C'est que on peut obliger et ça je m'y engage à ce que dans le rapport annuel de la LPM. On est tout un chapitre du Mans documenté sur cet aspect des choses mais un rapport dédié

Mais pas je dirais par le petit bout de la lorgnette et qu'on aura une réflexion sur l'ensemble. Je je peux retirer l'amendement. Et et je fais confiance. Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup dans un je m'y engage pour la mémoire des débats et de je vous l'écris comme ça, ça cadre les choses et de fait, je trouve ça bien de le traiter dans le tout parce que. Le ce qui fera aussi avancer le combat, c'est de le traiter comme étant un paramètre naturels basée ce clé dans la politique publique quand on le fait à côté. S'il y a toujours un tout petit bon moi y compris, donc merci en tout cas pour le retrait et ancien. Merci. Alors je mets aux voix l'article 5 qui est pour un contre qui s'abstient. Il est donc adopté à l'article 6, j'ai une demande de prise de parole de monsieur Marc Laménie. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre sur le président de la commission. Défense, Affaires étrangères forces armées en saluant aussi tout le travail qui a été fait sur sur ce texte important puisque l'objectif 400 milliards d'euros ont loi de programmation militaire et concernant ce cet article. 6. Ben j'associerai aussi à mes propos, ma collègue sénatrice des Ardennes. Elle se Joseph puisque je dirais. Dans les Ardennes, on a la chance, vous connaissez bien notre département. Monsieur le Ministre, n'a la chance de voir un régiment, le 3ème régiment du génie. Et et là cet article si ce sont les moyens humains, les effectifs. Donc je crois que c'est réellement particulièrement. Importants et malheureusement. On regrette souvent que beaucoup de départements non plus de militaires dans dans les départements et. L'évolution des effectifs. Ce serait l'objectif de 175.000. Et qui Valenton plein en 2030. Alors la question c'est quand même comment susciter les vocations. Même si on annonce vous annoncez, monsieur le ministre, une progression forte de la réserve opérationnelle. Comment susciter les vocations. Les difficultés de recrutement. Bon c'est c'est souvent rappelé et puis aussi, il a certes la la JDC le service national universel dont nous accueillons les Ardennes régulièrement. Je dirais des des jeunes de 15 17 ans le service militaire volontaire et puis aussi le lien avec l'éducation nationale les classes défense dans des collèges dans des lycées, donc il y a un lien aussi important. Alors pour et puis aussi fidéliser les effectifs parce que je dirais dont le SNU et aussi beaucoup de dévouement aussi des encadrants et je crois que c'est mérite d'être souligné. Mais c'est surtout fidéliser et susciter les vocations. Voilà je voterai cet article, merci. Merci. Monsieur Philippe Folliot. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le président. De la commission. Mes chers collègues effectivement cet article si ce concerne la manoeuvre RH et c'est. Un élément important. Nous sommes quelques-uns à avoir en mémoire un temps finalement pas si lointain où. Le seul ministère des de de la Défense supporter les 2 tiers des baisses d'effectifs dans. La fonction publique et donc le fait qu'il y a une augmentation nette hein. Telle que proposée dans le cadre de cet article est un élément éminemment positif dont nous ne pouvons que nous réjouir. Monsieur le Ministre, je voulais juste vous. Interpeller sur pour être logique et en cohérence avec. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si vous vous être difficile, je le comprends bien de, de nous dire à ce stade là. Où vont aller ces augmentations d'effectifs. Mais est-ce que en fait il y aura un objectif en ce qui vous quoi hein. D'essayer de faire de telle sorte par rapport à ces enjeux que j'ai développé tout à l'heure relatives forces de souveraineté qu'il puisse y avoir. Un, j'allais dire. Un petit peu. De d'orientation dans ce cadre-là et puis ensuite le 2ème point. Et comme l'a dit notre collègue tout à l'heure fort justement il y a un entre éléments qui est très important par rapport à la manoeuvre. Effectif. C'est la fidélisation donc de celles et ceux qui font le choix des armes parce que nous sommes dans une situation qui dans certains bassins d'emploi se rapproche du plein emploi et que donc dans ce cadre-là, il est important de faire de telle sorte que celles et ceux qui signent un contrat puisse rester rester le plus longtemps possible tout au moins le temps où ils auront profité de leur formation et c'est un enjeu qui est un enjeu important pour la suite. Merci. Alors, nous passons à l'amendement 98 de même Carlotti. Oui merci madame la présidente. Le projet de loi de programmation militaire vient interrompre la trajectoire d'augmentation des effectifs qui était prévus par la précédente loi de programmation militaire. Elle réduit le nombre de d'embauche en 2024 et en 2025 puisqu'on est passé de 1500 équivalents temps plein prévue pour 2024 prévue pour 2025 et on passe à 700 en 2024 et 700 en 2025. Donc je trouve que la montée en puissance des recrutements et repousser là aussi un peu comme pour la la trajectoire financière est repoussée à la fin du mandat du président de la République est ce qu'on a le droit d'attendre autant de temps et de perdre autant de temps pour doter nos armées d'effectifs suffisants afin de faire face, comme vous le dites souvent à la, à une guerre doit intensité je sais pas on perd beaucoup de temps dans le recrutement des effectifs. C'est pourquoi nous procès nous proposons dans cet amendement de reprendre les objectifs de l'ancienne loi de programmation militaire

il nous apparaît que cette trajectoire. Et n'est pas cohérente avec la trajectoire budgétaire qui a été adopté par la commission et. Et donc il nous semble que la cette nouvelle trajectoire. Pour la création de postes dans le périmètre du ministère des Armées. N'est pas la bonne, donc je propose un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui merci beaucoup madame la présidente, madame la ministre, Je pense que c'est un amendement d'appel en tant que telle parce que par définition la structuration du tableau. Fait que ce ce n'est pas évidemment complètement faisable. Je pense que l'urgence si un combat, c'était dit par le sénateur Folio si un combat à mener, c'est évidemment la fidélisation. On est un. Grand ministère employeur et dans lequel le solde entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent doit rester évidemment un solde positif et ça évidemment c'est pas tant l'attractivité pour embaucher la capacité a gardé un certain nombre. De de de de personnel et de cible particulière de personnel, pardon de le dire de manière un peu technique. Ça m'amène à deux public qui mérite à mon avis attention assez particulière. La première, c'est celle d'une sous-officiers qui constituent la la structure quand même du modèle d'armée et en fait on le voit bien ou au fur et à mesure des années, les revalorisations. Du SMIC et du point d'indice font qu'il y a eu un tassement entre les soldes de la troupe et évidemment les 1er grade de sous-officier sergent ou second maître sergent-chef et évidemment ce déséquilibre. On le retrouve dans l'ensemble de la pyramide des grades. Donc ça c'est le 1er combat si j'ose dire à mener. Vous avez pris des amendements en commission qui vont dans le bon sens qui correspond, cet engagement-là je pense que pour ces le ceux qui suivent les débats avant de parler des chiffres et nos armées regarde le débat, je pense qu'il faut renvoyer ce message important. Le 2ème, type de métier sur lequel il y a un enjeu important en matière de fidélisation. Et d'ouvertures de postes nouveaux, là on commence à avoir la jonction des deux c'est évidemment ce ne sont pas évidemment les métiers autour du cyber. Qui sont évidemment des métiers particulièrement chassés par le privé et ça vaut aussi d'ailleurs pour la DGSE dans lequel vous avez de jeunes gens qui commencent leur formation qui sont embauchés. Au sein des structures différentes structures cyber du ministère et qui au bout de 4 ou 5 ans pour des enjeux de fidélisation salariales mais pas qu'eux aussi de mobilité enfin bref. Le problème est complexe, sont amenés malheureusement a quitté le ministère. Donc ça, c'est de les, de les de combats. Vraiment, absolument clé de la réussite de la programmation militaire. Ensuite il y a une courbe effectivement d'augmentation de de TP alors. C'est là où on ne peut pas comparer la LPM entre elles parce qu'après tout. Jadis, il s'agissait d'augmenter les structures de combat quand je dis jadis dit il y a longtemps. Par exemple sur des régiments d'infanterie. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est pas tellement sûr l'infanterie de mêler que nous sommes attendus que plutôt justement sur la guerre électronique ou sur la transformation cyber de l'armée de terre. Donc on a une trajectoire qui correspond aussi aux besoins des employeurs. Et à la réalité aussi des capacités, embauché et surtout la capacité à fidéliser parce que sinon on remplira jamais évidemment les différents objectifs qui sont assignés de par de par la loi, donc avis défavorable aux demandes de retrait plutôt parce que c'est un, un amendement d'appel. Et je pense qu'au fond dans le bilan annuel de la LPM, à chaque fois devant vous, j'essayerai de justifier chaque année en tout cas. Où mon successeur ma successeure comment on est arrivé à remplir l'objectif ou pourquoi on lui ait pas arrivé et surtout vous donner des éléments analytique parce qu'au fond le remplir sur la troupe, c'est pas la même chose que de le remplir. Sur la DGSE qui n'est même pas la même chose que de le remplir sur les fonctions de soutien et ça aussi j'amènerai pour les réserves mais c'est l'approche qualitative évidemment de la de la. Pardon d'avoir été long mais ça me semblait important d'être complet, la ministre. Oui madame Carlotti. Oui, merci Monsieur le Ministre, oui je vais retirer cet amendement et sachez que sur les deux combat que vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure nous avons déposé des amendements, notamment sur l'mis des bornes pour l'évolution indiciaire parce que je crois que c'est très important et deuxièmement sur les, la question de la fidélisation beaucoup d'amendements de notre commission répondent à ce souci et donc je réponds moi au président Cambon et je lui dis qu'effectivement au regard de la trajectoire que nous avons. Adopté à l'article 3 donc je retire cet amendement. Merci. Alors 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 197. Monsieur le Président compta. Comme le précédent au sujet du du SNU puisqu'on retrouve. La mention et l'indication du SNU dans cet article 6 et donc on voulait ajouter la mode, la notion de de volontaires. Voilà bon je pense que je peux je vais le le retirer puisqu'on a eu on a eu les débats tout à l'heure, mais en tout cas voilà il y a un un quand même un problème de cohérence puisque le SNU, on le retrouve tout au long de de ce texte. Merci. Alors le 97. Madame Carlotti. Alors le 97, il est en 2 parties sur l'alinéa 4, j'avais fait une reformulation que je trouvais plus clair, plus incisive pour dire qu'effectivement, mais on l'a dit tout à l'heure que la loi de programmation militaire ne prévoit pas la mobilisation des ressources humaines désarmées pour la mise en place du disciple positif du SNU. c'est dedans. Donc moi je préférais ma formule mais celle adoptée par la Commission me convient très bien. Et deuxièmement, je remercie le ministre de s'associer et de soutenir l'amendement socialiste à l'alinéa 6 puisque vous proposez comme moi, la suppression de la référence c'est.

et rajoute le fait que ce n'est pas dedans donc ça revient à peu près avant ajoute une phrase dans un cas eux donc. Sagesse sur votre amendement évidemment enfin je non je je redonne juste la lecture quand même pour le, le Sénat. Sur la réserve à ses effectifs s'ajoutera enfin l'augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire et du service national universel portée à 80.000 en 2030 puis à 105.000 et etc donc ça, je le redis, même s'il y a eu des velléités parfois par certains services de mon ministère, de se dire que si jamais le SNU peut-être que moi je ne rentre pas là dedans, je donne mon engagement auprès du Parlement. Le SNU n'est pas dans la LPM. Et il n'y a pas de lien entre le service national universel et les augmentations des cibles de réserve sauf évidemment à ce que des jeunes de même volontaire au SNU deviennent volontairement réservistes mais ça ça tombe tellement sous le sens qu'il a pas besoin de le, de L'eau mouille et le feu brûle bon donc. Vraiment je défends cet amendement farouchement parce que sans quoi, ça veut dire qu'on se retrouve avec le SMI dans la programmation militaire. C'est tout l'inverse de ce qu'on se dit donc voilà non mais je, je sais que les services ont pu produire des choses. Il y a un ministre dans un ministère et c'est lui qui est responsable devant le Parlement. Donc c'est la constitution et rien que la Constitution le SNU n'est pas dans la loi de programmation militaire et par définition, il n'a pas de lien entre le SNU et les et les réserves en tout cas moi je souhaite qu'il puisse y avoir une clarification donc favorable même amendement même Carlotti si l'amendement du gouvernement n'était pas de. C'est l'inverse. L'avis de la commission, monsieur le président. Alors le 197 a été retiré le 90 le 97. Nous proposons. Un retrait puisque ça cet amendement était satisfait par les modifications qui a été ont qui ont été apportées en commission au projet de loi. Alors en ce qui concerne l'amendement 240, monsieur. Effectivement nous nous sommes basés dans un une proposition d'avis défavorable sur le fait que votre cabinet a écrit noir sur blanc qu'il fallait rajouter. Pour bien comprendre le chiffre de 80.015, 1000 en 2030 comptabilisés dans les effectifs d'augmentation de la réserve. Montée en puissance des volontaires du SNU. Bon, alors vous nous apporter une précision. Ça veut donc dire que vous engagez ici a atteint le chiffre de 80.100 les les effectifs du SNU. C'est bien ce qu'on doit comprendre. Auquel cas, dans ce cas-là l'avis de la commission est favorable. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement 97. Qui a reçu un une demande de retrait de la commission et un avis favorable du gouvernement. N'est pas retirée même Carlotti non donc je mets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mets aux voix l'amendement du gouvernement 240 qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est donc adopté. Le 241. Monsieur le Ministre, amendement du gouvernement. Oui madame. La présidente. Alors le gouvernement s'il a le droit de faire des amendements d'appel. Je je n'arrive pas à comprendre la la trajectoire telle qu'elle est proposée par la Commission sur les réserves. Pour plusieurs raisons. Enfin première question déjà. Celles et ceux qui ont introduit la disposition. Comment l'avez-vous calculé sur quelle documentation et quels besoins en matière de ressources parce que là on a une division d'un objectif linéaire. Or, pour le coup je vous reste persuadé que. Le combat pour les réserves. C'est un combat qui doit se mener. Je, c'est un combat qui sera très enfin qui a beaucoup d'aléas, évidemment parce que on est pas sur une politique salariale classique, la réserve un engagement individuel. Il y a une géographie déjà des réservistes et puis accessoirement. C'est pas complètement la même chose entre officiers sous-officiers et hommes du rang. Que c'est pas complètement la même chose entre Marine nationale Ahmed Terre et armée de l'air que c'est pas complètement la même chose entre. Territoires d'outre-mer et l'Hexagone que d'ailleurs si on avait une approche des réserves d'un point de vue purement militaire. Je pense qu'il faudrait davantage regarder les priorités par unité. Plutôt que par chiffre. Donne 2 exemples très concrets, délégation générale pour l'armement et évidemment, service de santé des armées sur lequel le besoin réservistes. C'est très important. Donc moi je questionne le Sénat. Pourquoi on a cette chronique qui déjà ne semble pas réaliste pour être complètement transparent et surtout s'éloigne, me semble-t-il des besoins militaires mais je, j'ai besoin de le comprendre. 2ème des choses, pourquoi. Plus de 25.000. Soit 65.000 ont tout. C'est-à-dire en clair, on est à moins que l'ambition initiale. Je vous rappelle que on est sur 80.000 autour de 80.000, là aussi faut, enfin c'est pas scolaire comme débat dans une programmation autour de 80.000 réservistes, en 2030. Autour de 100.000. C'est une idée du ratio qui compte, c'est ça qui est intéressant politiquement dans le format d'armée on à 200.000 soldats d'active. On a donc à terme, l'objectif d'avoir 100.000 réservistes et c'est donc un modèle d'armée dans lequel j'espère qu'un jour on pourra dire, nous avons 300.000 militaires, dont 200.000 d'active et 100.000 réservistes, c'est ça l'esprit. Mais vous auriez droit de me dire mais pourquoi pas 95.000 ou 105.000. Vous avez bien raison de me le dire, ça se trouve, d'ailleurs ça sera comme ça à la fin mais ce n'est pas grave, c'est le ratio qui compte en tout cas là sur la chronique telle qu'elle est proposée on a. Une chronique de réserve qui est plus faible que ce que le gouvernement avait, avait proposé. Et je ne comprends pas pourquoi au fond il y a une proposition de réduire l'ambition d'ou l'amendement 241, porté par le gouvernement pour revenir évidemment la chronique sachant que. si à la rigueur vous souhaiter une chronique. Moi ce que j'avais demandé aux états majors, mais attention ça sera toujours une chronique indicatives et elle ne saurait être contraignante. C'est pas une chronique capacitaire pour acheter. C'est pas une chronique budgétaire pour avoir des ressources. On est sur une politique fondamentalement humaine là je pense qu'on serait détachée de toute forme de réalités de la vie des forces si on était dans une prescription donc il faut que ce soit un objectif mou bienveillant parce que sans quoi il sera pas compris par les états majors et par les forces si on devait être sur une chronique

je ne suis pas en commission. C'est bien dommage. Et non mais je. Je je ne sais pas ce que a voulu faire le Sénat en commission donc je pose la question moi je peux je peux évidemment sous-amender, si il y a une demande parce que je veux montrer ma ma bonne volonté à à une Oui voilà j'allais dire une condition de bon sens et que celles et ceux qui regarderont la loi en 2029 ou 30, on sera plus là de de dire. Ne pas dire aux états majors, à ce moment-là vous n'avez pas rempli la cible et cetera parce que ça doit rester quelque chose qui crée une chronique avec la même transparence. J'ai demandé aussi à ce qu'on commence à réfléchir à des objectifs par territoire parce que quand le délégué militaire départemental de la Vendée au hasard aura des objectifs. Ça lui permettra évidemment d'être un peu plus motivé pour arriver à les remplir. Donc je pense que ces affaires, de chroniques peuvent être regardés de différentes manières. Merci. L'avis de la commission, monsieur le président. Monsieur le Ministre, j'ai, je vais vous expliquer comment nous avons procédé alors effectivement votre amendement vise à supprimer cette trajectoire des hausse annuelle des effectifs de la réserve opérationnelle donc nous il nous paraissait que ses objectifs étaient trop flous puisqu'il y avait en fait 2 jalons de rendez vous, 2030 et 2035, c'est-à-dire sept, ans et 12 ans après le vote de la loi, c'est quand même un petit peu incomplet. Alors on a demandé des précisions à vos service et j'ai ici le texte de la commission

il y a un rattrapage des femmes 15.000 du SNU, qui ont disparu dans la bataille. Donc. On on s'est vraiment basé sur les renseignements que vous nous donnez il y a un petit problème de méthodologie si une réponse écrite que j'ai. vous si vous rectifiez les chiffres on devient voir notre position mais sinon on donné un avis défavorable, parce que on souhaite préciser cette montée en puissance des effectifs de la réserve opérationnelle. Merci, monsieur le Ministre. Une fois de plus. Dans notre Constitution. Tous les questionnaires ne remplis ne remplaceront jamais le ministre et je pense que c'est important de le redire. Et là, telle qu'on a cette rédaction on a bien une diminution de l'ambition Je je leur redis donc moi je suis prêt à à à déposer un sous-amendement ou un autre un nouvel amendement. Le problème c'est qu'il faut suspendre j'imagine, pour ça puisqu'il s'agit quand même de produire un tableau. Chiffré. Pardon. Là ça fait un peu juste. De fait, après, ça peut aussi un engagement du ministre ici à avec une chronique puisque de toute façon dans une part aussi indicatif comme je le disais et donc je la mémoire des débats le compte rendu faisant foi. Le Parlement est ainsi éclairé des objectifs que veut remplir le gouvernement en la matière, sachant qu'une fois de plus, même le jalon à 2032 1035. Il est pas si grave. J'ai envie de dire le vrai sujet c'est par armée par service et pourquoi pas même par grade parce qu'au fond quand on dit augmentation du nombre de réservistes. Il y aura aussi une réflexion sur le pyramidal. Si c'est une armée d'officiers de réserve. La belle affaire. Il faudra aussi quand même qu'on ait des sous-officiers qu'on est des hommes du donc de toute façon il y a peut-être une approche globale, après je peux aussi. Si vous le souhaitez, produire ou imaginer un rapport aussi au Parlement sur le les réserves ou dans le cadre d'audition spécifique du ministre venir présenter aussi la politique des réserves en tout cas moi je me dérobe pas parce que je suis transparent avec vous, pour réussir cet objectif je vais avoir besoin de vous également parce que c'est une affaire aussi humaine de mobilisation de la nation pour que les gens s'engage et donc ce n'est pas que prescripteur. Ça doit être aussi un élément de motivation. Monsieur le Président, je voudrais je vous donne la parole et de nous éclairer un peu sur ce que vous souhaitez faire à ce stade. Allez-y, monsieur le président. comme on est très fâché que votre cabinet nous donnent des réponses qui ne sont pas les vôtres. Donc, je me réserve ça pour la va s'expliquer. D'ici là donc pour l'instant, garde un avis défavorable. J'entends vos explications mais sincèrement dites à votre cabinet de. De contrôler les informations qui nous donne. C'est difficile pour la Commission de travailler. On vous a déposé un questionnaire de 82 question justement pour éclairer le Sénat et si les réponses ne sont pas les vôtres c'est un peu compliqué donc rendez-vous à la CMP sur cet amendement. Mercier même Carlotti

dans le travail de la commission c'est ne pas de mettre un carcan. Vous disiez tout à l'heure je vous ai écouté, pas de carcan. C'est pas un carcan s'est c'est donner une vision donner quelque chose dont moi je je. S'il avait eu la possibilité que vous posiez un amendement en séance en ce qui nous concerne, notre groupe l'aurait accepté hein parce que à ce stade. C'est compliqué de, de voter favorablement. Votre nous ça sera défavorable à moins que vous puissiez faire un amendement mais j'ai écouté le président Cambon. Merci vous voulez reprendre la parole monsieur le ministre. Puisque nous sommes éclairés. Si l'amendement de toute façon devait être adopté, il y aura une suppression pure et simple de la chronique, ce qui, pour la CMP priverait me semble-t-il si je me trompe pas une discussion puisque le tableau disparaîtrait. Donc, puisque nous travaillons en bonne Intelligence. Moi ce que je vous propose c'est, je retire l'amendement du gouvernement comme ça le tableau reste. En l'état, il vous fait une accroche pour travailler avec. Vos collègues parlementaires et en revanche on n'en reste pas à cette chronique de chiffres on la complète peut être aussi qu'on peut le tableau pour aussi. Rendre plus. D'écrire la politique publique de la réserve grade service etc pour montrer qu'on est sur une cible complètement indicative et non pas prescriptives en tout cas c'est le le voeu que je forme en le faisant comme ça donc amendement retiré. Merci Monsieur le Ministre. Mais je vous redonne tout de suite la parole pour défendre votre amendement 292. Oui il est défendu madame la présidente. Pour éclairer le Sénat. Donc il s'agit de de de recompléter le l'Linea. Il se trouve que c'est une souplesse. Que vous avez supprimé en commission mais qui fonctionne bien dans la vie quotidienne du MIN armes avec. Avec Bercy pour être très clair. Et que globalement. Cette Cette capacité à avoir de la souplesse dans la gestion des ETP est globalement très attendue des états majors pour être très Direct. Et que jusqu'à présent, ça a bien fonctionné avec. Avec l'interministérielle. Se priver de cette souplesse et nous renvoyer à la rigidité. De comment dire de l'organisation des ETP et à mon avis, ça ne va pas dans le bon sens. Donc. Je je. Pour le ministère, je je je recommande. Enfin vraiment chaleureusement et fortement le fait de revenir à la rédaction initiale. si l'avis de la commission, monsieur le président. Alors. Je je je vous suggère Monsieur le Ministre de de convaincre d'abord le conseil d'état parce que sur cet alinéa que nous avons supprimé dans son avis du 30 mars 2023, il a rendu un avis, considérant que ces dispose de cet alinéa était obscur. Et donc nous l'avons supprimée pour 2 raisons, d'abord parce que sa portée normative n'est pas établi par. N'est pas établie par le ministère et par ailleurs on considère que les recrutements du ministère de la Défense ne doivent dépendre que de vos besoins opérationnels exprime par les armées, ce qui nous sommes tout à fait recevable et qui n'est pas souhaitable de les faire dépendre de la situation du marché du travail, donc à ce stade, nous rendons un avis défavorable. Merci monsieur le ministre. Oui, il est peut-être obscur pour le Conseil d'État mais il est bien utile pour les armées, donc puisque vous voulez défendre. Le ministère des Armées. Ce que vous m'avez dit plusieurs fois Monsieur le Président commission. C'est un dispositif de souplesse qui aide les employeurs militaire quand on parle de situation sur le marché du travail, c'est évidemment le dumping dont je pouvais parler tout à l'heure sur les métiers du cyber d'aménager justement l'architecture des postes parfois les systèmes de rémunération. Donc là on est en train, enfin Qui n'est pas profitable aux armées françaises donc je, je le redis avec la même chaleur et la même engagement que le président Retailleau tout à l'heure, on est en train de priver le ministère des Armées d'un bon outil pour les armées. Même si vous voulez faire plaisir au Conseil d'État, je le note donc je je j'appelle véritablement le Sénat a voté l'amendement du gouvernement, non pas parce qu'il viendrait du gouvernement mais parce qu'il est bon pour les armées. Je ne peux pas dire mieux. Merci Madame Carlotti. Monsieur le Ministre, encore un amendement de souplesse encore une rédaction souple. Non, on ne veut pas faire plaisir au Conseil d'État. Il, c'est vrai qu'il est confus, cet amendement, nous on a on a décidé au sein de laquelle de ne pas de ne pas l'accepter parce que il laisse entendre que les recrutements des ressources humaines se ferait en fonction du marché du travail plutôt que dans l'intérêt des armées et donc ça va à l'encontre avec ce que vous avez dit tout à l'heure et que nous défendons ensemble, c'est-à-dire la fidélisation l'attractivité. Donc nous on l'a compris, comme ça, ça veut dire qu'il est pas très clair. Merci. Alors Monsieur le Président Cambon. Nous, féministes, j'entends bien, j'entends bien vos observations. Donc ce que je vous propose c'est de rerédigé cet amendement d'ici la CMP, on verra si notre position peut évoluer mais pour l'instant je maintiens la position de la commission. Merci monsieur le ministre. Là pour le coup je maintiens vraiment l'amendement du gouvernement parce que. C'est en fonction de la situation du marché du travail que le ministère des Armées à de la souplesse avec Bercy pour pour discuter et adaptée chaque année les choses, vous avez une programmation militaire et derrière, vous avez évidemment des tensions qui peuvent apparaître ici ou là, soit par bassin. Surtout par métier. En fait, c'est surtout ça la finalité et qui permet à l'employeur de militaires de garder au fond ces ETP et de les redistribuer sur un autre besoin et ça c'est vraiment le boulot des majors généraux des 3 armées la DGA fonctionne un peu différemment et le service de santé des armées aussi et en fait c'est sur la base de ce qui est écrit là que le ministère des Armées peut le faire dans le dialogue avec Bercy si c'est supprimé, ça ne sera plus possible, et une fois de plus, je le redis parce que je ne prends personne en traître. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le ministère des Armées. Vous voyez même l'interministériel m'a autorisé déposé l'amendement. C'est dire si c'est quand même quelque chose auquel je tiens donc voilà je, je, j'insiste, je pense qu'il faut adopter cet amendement du gouvernement pour le bien du ministère des Armées. Merci alors je mets aux voix l'amendement 292 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est donc pas adoptée, je mets aux voix l'article 6 qui est pour. Contre qui s'abstient. Il est donc adopté à l'article 7 l'amendement 61 monsieur Oui madame la présidente, monsieur Miss c'est un monument qui a pour objectif de garantir la mise en oeuvre de que la mise en oeuvre de la programmation se fera dans le respect des villes la dignité humaine et vise à renforcer les principes éthiques et les droits fondamentaux qui doivent guider toute action militaire dans le cadre de cette loi. Pas de préjudice avéré causés aux à la dignité humaine des mécanismes de réparation appropriée devront être mis en place. Mises en place pardon pour assurer une protection adéquate des personnes affectées. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le. Président. Président, on est évidemment très sensible à la dimension éthique et au respect du droit international humanitaire la France se tient ces notions pour tout à fait fondamental mais cet amendement n'a absolument pas sa place à l'article 7 puisque l'article 7 concerne les conditions d'actualisation de la programmation militaire. Donc je pense que le plus simple c'est peut-être. Sans ça, un avis défavorable. Merci monsieur le ministre-président même avis monsieur Bono je le retire. Merci. Alors 2 amendements en discussion commune le 242. Monsieur le Ministre, pour le gouvernement. Oui merci. Mais la présence. C'est un moment d'appel là aussi sur le Livre blanc bon je suis au fond. Ni pour ni compte comme dirait l'autre, bien au contraire. Je ne peux pas ne pas voir quand même que les exercices des livres blancs et dans la mémoire et dans l'impression rétinienne des forces armées sur les deux derniers exercices ce ce, ces livres blancs ont été quand même imaginer pour malheureusement faire endosser techniquement une légitimité qui permettait d'erreurs de diminuer les crédits militaires, c'est comme ça que c'est vécu au sein du ministère des Armées et c'est une réalité. Bon 2ème des choses et ce qu'il faut à l'avenir imaginé des comitologie qui permette de réfléchir tous ensemble. La réponse est oui c'est mal un peu ouvert le débat. Lors de la DG enfin la discussion générale tout à l'heure la prison comme on l'a dit, jamais une LPM n'a été autant travaillé chacun de l'a fait à sa manière, moi je. Vraiment je vous le redis, mais l'ensemble des contributions des parlementaires par les nombreux rapports qui sont produits par les commissions ont largement été intégrée ce que d'ailleurs trop souvent ce n'était pas le cas dans le livre blanc parce que telle ou telle think tank ou lobbies d'intérêts étaient parfois beaucoup plus sonore et beaucoup plus vocale que un rapport parlementaire. Non mais. Or si on est honnête, la loi se construit quand même avec le Parlement et dans la démocratie représentative, c'est quand même bien de commencer par là. vraiment et je pense que là pour le coup c'était le PM elle elle puisse à son le nombre d'amendements, déjà à l'Assemblée, au Sénat, la manière dont on le fait c'est bon et puis si j'ose dire Monsieur le sénateur es mal votre article 1er plus votre discussion générale vous avez brossé globalement toutes les menaces. Il y a que le mot Iran que vous n'avez pas cité sinon tu. Vaut déjà tous les livres blancs. Donc, donc moi je, je ne me battrai pas. Sur cet amendement, là, à la différence du précédent qui était vraiment une mauvaise nouvelle pour le ministère des Armées. Autant que celui-ci. Je pense qu'il doit redéfinir un cadre, au revoir. Moi j'ai une conviction et je dit à à la tribune. Il faut davantage repartir des orientations politiques des parlementaires. Moi je préfère le président Laurent. Qui. Vient avec ses convictions et la sénatrice homme. je reviendrai plus tard dans la, dans la discussion sur la dissuasion nucléaire sur le temps, je ne suis pas d'accord avec vous mais ça me semble bien mieux que d'aller parfois capter ici ou là. Différents groupes d'intérêts je vous le dis comme je le pense qui ont parfois des intérêts a poussé un certain nombre d'amendements ou de préconisations dans un livre blanc. Et pardon je m'arrêterai là, mais je peux refaire la chronique du dernier qui a quand même montré aussi de sérieuses limites et et de sérieuses difficultés en tout cas moi je suis favorable à ce qu'on continue de réfléchir à une méthodologie pour l'avenir, ça, ça participe évidemment à la construction de la loi. Merci la maman 76

d'accord. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre bon cet amendement vise à renforcer le dispositif prévu visant à mettre en place une commission chargée d'un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et s'assurer que cet engagement sera effectivement proposé sera effectif en proposant que cette commission devrait être mises en place avant le 30 juin 2028. Alors que la LPM qui succédera à la LPM 2024 2030 devra être votée dans le courant de l'année 2029. Alors pour rappel quand même un livre blanc est chargé. Monsieur le Ministre, de définir une stratégie globale aussi de défense et de sécurité, c'est également l'occasion de donner une certaine visibilité nécessaire à l'ensemble des acteurs chargés de notre sécurité allant de ce qui bien évidemment produisent les matériels militaires à ceux qui les utilisent, c'est-à-dire nos militaires en passant par celles et ceux qui votent les Budgets c'est-à-dire les parlementaires en fait pour nous c'est autant le document qui est important puisqu'il sert de référence pour définir des objectifs et une vision stratégique dont nous avons besoin que l'exercice de concertation qui a quand même cruellement manqué au texte que nous examinons. Je ne partage pas d'ailleurs forcément votre avis que le seul objectif d'un livre blanc serait de limiter les le budget. Alors vous l'avez compris, nous sommes attachés à la concertation au travail approfondi et sérieux de réflexion qui, pour un sujet aussi régaliens que celui de la Défense nationale demande je crois un engagement de toutes et de tous. Il y va de notre sécurité et de la paix à laquelle nous sommes. À laquelle nous aspirons voilà donc le Sénat entend. Jouer pleinement son rôle dans cet exercice de concertation que le livre blanc propose, je vous remercie. Merci monsieur le président. L'avis de la commission. Oui, cet amendement qui a été déposée par. Nos collègues du groupe socialiste est un petit peu le résultat de la frustration que nous avons ressentie lors de la préparation de cette LPM où il nous a été communiqué communiqué une revue stratégique qui a été rédigé excessivement rapidement et qui n'a pas véritablement associer le Parlement à sa à sa conception, comme ça avait été le cas précédemment donc. nous soutenons cette demande, c'est de toute façon c'est pour la prochaine LPM sont c'est que c'est aux alentours de 2028, on a encore le temps d'y réfléchir et bien évidemment le second amendement, nous donnons un avis favorable puisque il faudra constituer la commission préparatoire à ce livre blanc donc avis défavorable sur l'amendement du gouvernement est favorable sur l'amendement du groupe. Merci, monsieur le Ministre oui défavorable. Oui. Alors Monsieur le Président. Laurent, vous aviez demandé la parole. Oui je crois que ce ce débat sur le Livre blanc il témoigne. De ce que j'ai essayé moi même de dire dans la question préalable, quelles que soient les débats sur le fond une très grande frustration partagée du Parlement sur la préparation stratégique de de la LPM et je pense que, quoi qu'on dise les uns et les autres ici. Ce, ce manque de conception partagée. Nous allons le ressentir. Au fur à mesure des évolutions désormais extrêmement rapide de la situation internationale et des gens et des enjeux. De défense. Donc je pense que. Le texte actuel. Amendé par la commission renvoie encore très loin ce travail. Donc moi je, je vais soutenir l'amendement. Socialiste parce que au moins il se donne une perspective. Plus. Parce que ce travail est indispensable. Il n'a pas été menée dans le dans la préparation de cette LPM il restera indispensable et le repousser à la fin de cette LPM je pense c'est trop tard. Nous n'avons pas eu de débat sur l'actualisation du LPM. Nous avons raté la la la préparation de celle-là. Se dire qu'on va rediscuter de tout ça. Dans 7 ans c'est trop loin à la vitesse à laquelle évoluent les choses, donc il faut des échéances. Plus sérieuse et plus rapide, donc en l'état avec toute la frustration ça. Signifie pour moi et pour mon groupe mais on votera quand même l'amendement socialiste parce que c'est celui qui nous rapproche le plus d'un travail collectif et national absolument indispensable. C'était mal. Merci à la prison. Monsieur le Ministre, vous évoquez le la question du Livre blanc et du passé. J'ai envie de vous dire que je pensais qu'avec le nouveau monde. Il y aurait justement avec la même chose mieux mais ça c'est Moi je ne vois pas en quoi en. Enlève serait un problème, je pense que c'est, vous l'avez dit, la façon d'associer l'ensemble des parlementaires. Mais je voudrais élargir un peu l'espace du débat parce que. D'abord ça serait bien d'avoir les parlementaires le Parlement dedans mais évidemment la question des Français même plus largement puisque et on le voit d'ailleurs sur la question. En Ukraine, on voit bien que la population qui a mon et ce sont aussi concernés par sa propre sécurité peut être associée et c'est vrai qu'en France. Assez peu le Parlement déjà mais encore moins les Français, nous avons un débat dans notre pays sur les questions de défense. Donc moi je pense qu'à mon et je ne dis pas que là on n'a pas d'amendement. En l'espèce à ce stade, mais peut-être qu'il faudrait aussi dans la prochaine phase. S'il devait avoir une nouvelle. Loi de programmation militaire poste. Celle que nous sommes en train de voter, je crois que la question de la, de l'association des Français plus largement non me semble essentiel parce que si on veut encore une fois que la question de la défense soit partagé autant que les Français soient aussi associés en amont et puis il y a, je crois que vous avez su vous-même d'ailleurs par le passé, faire des grands débats ou autre, on pourrait imaginer différentes formules. Je crois que c'est un des sujets qui sera quand même devant nous. Malgré tout, Madame après cette LPM. Monsieur le ministre. Je dirais même plus, les élites aussi puisque je l'ai suffisamment dit ici au micro. Au pupitre, enfin la Tribune pardonnez-moi quand on voit un certain nombre de commentateurs. Qui place la France dans la même position que l'Ukraine en disant ben vous voyez. On peut tenir uniquement un front de 80 kilomètres pendant 15 jours et cetera ça veut dire qu'on a quand même des élites qui sur des plateaux de télévision. Non, absolument rien compris à ce que notre modèle l'armée. Sont-ils des élus. La question est posée donc par définition, il est clair que je suis pas certain que la la pour moi livre blanc ça correspond à 2 exercices normé. qui d'ailleurs n'associait pas la population sur les zones non mais je je donc. Quand on emploie le mot Livre blanc désormais. Vous, vous n'échapperez pas au fait que une partie de de notre écosystème. Politico-militaire renverra aux exercices du passé. Non mais vous diriez que à un moment donné enfin qu'il faille imaginer des des débats avec la nation mais je je sors de cette séquence et Ukraine. Et même sur ce que vous avez fait avec le le bon débat sur l'Afrique que nous avons eu ou au fond. Mais pourquoi nos militaires sont morts c'est c'était quoi Barkhane, à quoi ça servait et et même si je puis me permettre, madame la sénatrice tout à l'heure j'ai quand même un peu bondi sur sur mon banc lorsque vous avez comparé le nombre de chars Leclerc avec le nombre de chars russes. Mais nous ne sommes pas une armée d'agression. Nous sommes dans un modèle purement défensif et que précisément parce que nous avons notre dissuasion nucléaire, nous n'avons pas complètement les mêmes besoins sur le le le terrain conventionnelle et de fait vous avez si vous voulez supprimer la dissuasion nucléaire. Il faut plutôt faire des amendements d'urgence de cibles à 1000 chars parce que pour le coup on reviendrait dans une autre technique de défense donc. Les modèles sont ainsi mais je pense monsieur le président, Laurent. C'est pas vrai de dire que le travail n'a pas été fait. Il a été fait. Il a abouti sur un résultat que vous ne partagez pas. Mais il a été fait, pardon, par nos états. Il a été fait devant vous en commission. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans l'appeler mais. J'ai pas j'ai répondu davantage à des questions sur les marges frictionnel avec un succès limité, je le note. Que de parler justement du rôle de la France dans l'OTAN comme le sénateur tu es mal la fait tout à l'heure et pour le coup le débat à l'Assemblée nationale nous a permis de le faire pendant 15 jours. Seule. Les militaires sont justement prêts à avoir le débat y compris sur la dissuasion nucléaire c'est quoi le débat au Parlement sur la loi de programmation militaire, si ce n'est pas aussi un débat sur la défense nationale et je le disais ce matin dans les colonnes d'un quotidien. Moi en tant que citoyen, j'aurais préféré qu'aux élections législatives. Lors de l'Alliance dite NUPES qui ne concerne pas forcément cet intergroupe ici mais il y est pas du tout qu'il lui est une clarification sur le positionnement des 4 formations politiques qui forme la NUPES aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'étais bien en difficulté comme ministre au banc à l'assemblée de me retrouver dans une situation dans lequel tout le monde avait un avis différent sur le porte-avions la dissuasion les coopérations européennes l'OTAN donc de fait le débat avec la nation. Il est important et moi je souhaite aussi que lors des élections législatives ou présidentielles, on parle peut-être aussi davantage de défense nationale à ce moment-là en tout cas moi je retiens que la technique du Livre blanc telle qu'on la connue, je pense que malheureusement elle est à réinventer. Donc peut-être dans le cadre de la, de la CMP si il y a une rédaction que vous êtes capable de de d'imaginer qu'il ouvre à une manière d'associer mais aussi les élus locaux, les correspondants défense dans les collectivités locales les on parle de dualité, les entreprises qui ne sont pas dans la BITD mais qui peuvent être sollicités dans un schéma de résilience. Je pense que là pour le coup, moi je partage complètement cette cette vue, il est important d'embarquer la nation mais je pense qu'il faut qu'on soit imaginatif pour le faire parce que sans quoi, malheureusement on, on passera à côté en tout cas cela analyse stratégique. Elle a été faite elle produit une copie et on reviendra monsieur le sénateur, c'est mal promis sur France et autant parce que les interpellations que vous avez fait, sont très importante pour comprendre une partie de la structuration de la copie. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement du gouvernement numéro 242 qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ils ne ont pas adopté, je mets aux voix l'amendement 76 qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour, contre qui s'abstient et des donc adopté l'amendement 234 le président Gontard. Oui merci merci madame la présidente. Il s'agit d'un amendement qui vise à ce qu'un débat parlementaire sur la dissuasion nucléaire soit organisé avant la fin de cette loi de programmation militaire. C'est évidemment un à un amendement plutôt plutôt d'appel mais qui fait écho à ce que, à ce que vient de dire monsieur le monsieur le ministre, je pense qu'effectivement on a besoin d'avoir cette réflexion, on a besoin d'avoir ce ce débat. Et notamment sur la question de la dissuasion puisque on parle de dissuasion comme un fait un fait accompli. Je pense qu'on a besoin de de vraiment ouvrir le débat et de l'ouvrir même plus largement avec l'ensemble de nos, de nos concitoyens. La question la la dissuasion, vous m'avez dit monsieur le Ministre qu'on était contre la dissuasion. Je ne pense pas avoir dit ça. Aucun moment. Et à aucun moment dans mon intervention, je dis qu'on se poser des questions sur la question de la dissuasion et je pense qu'on a, on a raison de se poser des questions, comme vous dites, c'est entre 13 et 15% ça LPM. Ce n'est pas rien. Et qu'on a besoin aussi de se projeter sur cette dissuasion notamment dans l'évolution à la fois du du contexte géopolitique mais aussi du contexte technologique et qu'on a évidemment besoin d'avoir cette d'avoir cette réflexion et puis quand on parle de dissuasion. On n'est pas forcément sur la dissuasion nucléaire il y a aussi d'autres types de dissuasion et donc en tout cas tous tous ces éléments-là doivent s'ouvrir et dont on doit avoir cette réflexion là et donc voilà je pense que, encore une fois, il me semble qu'on a besoin de poser ce débat là, on a besoin de pouvoir l'ouvrir et également avec l'ensemble de nos concitoyens parce que c'est vrai que la dissuasion. Je pense que beaucoup quand on en parle, c'est vraiment pas quelque chose qui est totalement compris est totalement je dirais intégré. À la fois dans son fonctionnement et la foi dans ses projections. Donc voilà c'était plus à un amendement d'appel mais en tout cas je pense qu'on a réellement besoin d'avoir ce débat. Merci. Alors l'avis de la commission, monsieur le président. Je note avec intérêt que le groupe du président Gontard n'est pas totalement hostile à la dissuasion avec cette subtilité. Dissuasion dissuasion nucléaire, enfin pour nous quand on parle de dissuasion. C'est à peu près à quoi on pense bien évidemment la commission ne cesse de travailler sur la dissuasion avec ses rapporteurs avec ses commissaires avec nos auditions et donc nous nous nous poursuivrons ce travail. J'entends bien votre appel en revanche dans votre amendement il y a quelque chose. Qui n'était pas acceptable, c'est que le par le le le débat parlementaire que vous proposiez incluait l'audition d'une ONG en séance dans l'hémicycle. Donc ça je pense que. C'est pas vraiment souhaitable. Et donc je vous propose de retirer votre amendement on a bien attendu cet appel et on continuera bien évidemment au sein de la commission de travailler sur ce sujet. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Alors absolument contre non pas le débat. Mais le fait qu'il ait lieu plus tard c'est la loi de programmation militaire. Faut l'avoir maintenant. je vois la cavalerie aussi parce que après on reproche au gouvernement une insuffisance de préparation, la RNS, le ceci, le cela très bien là, on est là, si vous avez des questions, c'est la dissuasion. Monsieur le Président. Posez-les moi et s'il faut prendre toute la semaine et la semaine prochaine pour avoir un débat sur mais on ne peut pas aller, je veux bien la passion pour les marches la passion pour les marges frictionnel la passion pour les reports de charges au bout d'un moment j'ai j'ai formé ce voeu enneigé il y a un sujet qui est central. Si des sensibilités politiques des parlementaires ont des questions sur la dissuasion nucléaire, il faut le faire dès maintenant et avant le vote. Donc moi, si vous avez des questions, je suis, je l'ai fait à l'Assemblée, vous le savez, vous avez suivi, on est toute une nuit de débats avec les députés écologistes, les députés de la France insoumise. Essentiellement. Sur le sujet de la dissuasion et j'ai justement je n'ai pas voulu éluder en faisant face défavorable et cetera j'ai dit. Posez-moi toutes les questions et on a eu un débat de bonne tenue et de bonne qualité sur la dissuasion nucléaire ou d'ailleurs c'est là où je me suis permis de saluer pas pour donner des bons points des mauvais points, cela va sans dire, mais Fabien Roussel, le député pardonnez-moi a pris du temps pour réexpliquer la la position historique du Parti communiste c'était intéressant donc moi je je je mets un avis défavorable ou de retrait à cet amendement. Mais si vous souhaitez poser des questions sur la dissuasion. Monsieur le Président. Faites-le dès maintenant pour ne pas dans trois mois ou dans un an. Entendre dire que la LPM n'aura pas permis d'évoquer toutes les questions et qu'il aurait fallu faire un livre blanc pour le coup, c'est le moment posant des questions sur la dissuasion. Merci monsieur le président Gontard.

Aujourd'hui on a ce système de dissuasion nucléaire. Il a pas complètement dingue, je sais bien qu'on va pas l'arrêter du jour au lendemain ça il y a pas de souci. Et par contre de, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette dissuasion et quel objectif on lui donne et quelle orientation également lui donne je veux dire est-ce que c'est toujours plus de dissuasion. Est-ce que la France. Indique orientent justement sur une dénucléarisation et donne l'exemple et en tout cas réfléchi avec l'ensemble de ses partenaires. Voilà l'ensemble, l'ensemble de ces deux de ces questions. Donc effectivement sur la question de la dissuasion. Je pense qu'il y a il y a vraiment un, un débat et une réflexion, une Tout à l'heure je vous ai posé des questions, vous m'avez dit 13 115 % et je vous ai demandé justement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Est-ce que c'était justement du remplacement sur des armes liées à la dissuasion ou est-ce que c'était une évolution et ce qu'ont donné une puissance supplémentaire. Vous m'avez dit, secret défense. Donc moi je veux bien mais mais on a besoin aussi d'avoir ces éléments-là et ses orientations là donc voilà je pense qu'en tout cas le ce débat là il me semble pas inutile en tout cas je ne pense pas qu'il faut le prendre comme ça en se disant bon ben c'est bon et puis mettent des bons points et des mauvais points. Je pense que dans la population, tout le monde se pose des questions et a le droit aussi d'avoir des réponses et des réflexions en tout cas ce serait une erreur de pas réfléchir à ça. Si Monsieur le Ministre. Oui mais la présente. Moi je suis bien d'accord avec toute la dernière partie de votre intervention. Il faut avoir le débat parce que il en va de l'acceptabilité aussi. Sociétal je l'dis notamment pour les autres parlementaires qui sont vraiment pour la dissuasion nucléaire en disant, c'est comme ça, ça fonctionne circulaire. Rien à voir, ce n'est pas une bonne manière justement de défendre la dissuasion nucléaire. C'est pour ça que je je je je n'ai pas vous autoriser à me poser des questions des parlementaires, en revanche je je ne veux pas qu'on passe à côté du débat parce que sinon on ça sera pour mieux se plaindre qu'ils n'aient pas eu lieu et ça je trouve que c'est c'est c'est pas raisonnable parce que si nous ici au Sénat, on en débat pas, qui va en débattre à notre place. Très franchement, ça n'a pas de la patience. Vous m'avez posé une question précise, c'est. Au fond, 13%. Qu'est-ce que ça veut dire. Moi j'amènerai quand même plusieurs commentaires hein. Parmi les puissances dotées déclarer toutes ne sont pas des démocraties. Et donc par définition il nous faut nous comparer avec les trois démocratie nucléaire déclaré les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France, 3 pays d'ailleurs membre de l'OTAN. Laquelle France n'est pas membre de la planification nucléaire de l'OTAN. Ce qui est un des éléments aussi clé dans notre héritage évidemment. Gaullien. Parmi ces trois démocratie nucléaire je parle même pas de la Chine ou la Russie. Quel est le pays qui a la doctrine la plus lisible et la plus publique et je trouve que c'est la France. Avec cette permanence depuis le général de Gaulle le sénateur c'est mal a rappelé. Les engagements du président Mitterrand et du président Hollande, donc il y a quand même une une grande constance française non mais moi je moi j'aime l'histoire, dans sa réalité. Je l'ai fait le, ben il est pas de gauche, Jacques Chirac. Bon. Enfin. Et donc que Jacques Chirac soit dans la fidélité à ce que faisait le général de Gaulle ne semble pas surprenant sous le contrôle de celui qui fut son secrétaire général, Monsieur le Ministre, bah ce que je voulais souligner, c'est que les présidents Hollande. Et Mitterrand était aussi dans cette continuité. Ça pour le coup, c'est ce que voulait dire le le sénateur es mal tout à l'heure. Et cette doctrine qu'est ce qu'elle dit. Que par définition, on est pour défendre nos intérêts vitaux. D'une menace. Venant. D'un État. Ce qui donc déjà crée une voûte évidemment des éléments de contournement potentiel de cette voûte c'est ce que j'indiquais. En discussion générale. Que cette doctrine elle pointé du doigt le fait qu'elle était strictement défensive et suffisante. Et donc si votre question sous-jacente c'est mais c'est 13% là dans un budget global qui augmente. Est-ce que ça remet en cause le fait que notre dissuasion nucléaire et défensive et suffisante. La réponse est non monsieur le sénateur. Voilà et que donc ces crédits sont des crédits de renouvellement. De renouvellement dans des conditions opérationnelles qui change parce que évidemment les différentes menaces de l'adversaire nous conduisent à devoir faire attention je donne un exemple plein de bon sens et en sources ouvertes. L'acoustique des sous-marins. La signature acoustique d'un sous-marin mais il est évident que nous SNLE le troisième génération seront plus discrets que ceux de la 2ème génération et que, par définition, c'est un saut technologique et que, par définition, ça coûte de l'argent, c'est un exemple sur le SNLE. Ça pourrait être le cas sur d'autres sur d'autres types, donc je ne veux pas être plus long mais en tout cas il y a certes du secret défense mais il n'est pas fait pour évacuer le débat sur le fond, après on a eu un bon débat avec le parti communiste français à l'Assemblée nationale sur. Tian TNP. En quoi la France est engagée dans la non-prolifération ce qui n'est pas complètement la même chose que d'être dans une logique d'interdiction que nous combattons parce que l'interdiction, c'est le désarmement et c'est là où avec le parti communiste, on ne sait affronter entre guillemets entre désarmement multilatéral mais qui au fond dans les faits, on le sait tous est unilatérale, c'est là où Fabien Roussel a eu des propos. Évidemment intéressant parce qu'il a voulu aussi et je connais les choses. Bref, en tout cas je pense que c'est un débat qui est clé. Et si on ne l'a pas pendant la loi de programmation militaire pardon. On peut toujours renvoyer aux calendes grecques ou dans un débat spécifique, on ne leur a pas plu, ça c'est vraiment le coeur de la LPM. Hier, aujourd'hui, demain et qui permet aussi de regarder ce que la dissuasion ne couvre pas et c'est pour ça que je suis parfois un peu durs et engagé. Sur les nouvelles menaces parce que par définition une puissance dotée ces vulnérabilités, elles sont évidemment dans des espaces beaucoup plus hybride beaucoup plus sournois beaucoup plus pernicieux. Pas de face mais sur les côtés, c'est évidemment la question du cyber du spatial que j'évoquais précédemment. Merci à Monsieur le Laurent. Oui merci. Bon, c'est effectivement un débat très important. On va, on y on rebondira dans ce débat, plusieurs fois parce qu'il y a d'autres amendements dans la discussion qui nous permettront d'aborder certains aspects comme. La question de la non-prolifération et. Et du traité d'interdiction des des des armes nucléaires parce. On a fait des amendements là-dessus. Mais je pense que, au moins les chances qu'on a là a le mérite de dire que il y a besoin effectivement d'un débat national sur ces questions et la situation internationale, nous y invite. Parce qu'il faut avoir un débat avec la nation sur cette question très importante. Et vous le dites vous-même d'une certaine manière. la première réponse que vous nous avez fait tout à l'heure vous abritant derrière le secret défense. Je vous mets au défi de vous en tenir à cette question si vous étiez Fall face à une salle de 500 Français qui vous interroge là- dessus. Vous seriez obligé de rentrer dans plus de détails. Donc je ne vois pas pourquoi nous les parlementaires on devrait s'en tenir à une réponse qui dit secret de la défense, point barre, alors que nous débattons de cette question avec beaucoup de citoyens. Deuxièmement les la composante les composantes de la dissuasion ont connu des évolutions. Déjà des évolutions significatives depuis la création de la dissuasion française. Le format de notre dissuasion n'a pas toujours été le même. Il a évolué. Donc nous pouvons nous poser des questions sur le format de la dissuasion ou en tout cas demandé des débats ou avoir des débats sur ces questions là sans être. Renvoyées à des gens qui sont des irresponsables par rapport à cette question. Hein puisque ces questions là. Ces évolutions-là ont eu lieu.

Oui madame la présidente, enfin. Après, on reproche au gouvernement. Que il n'y aurait pas suffisamment de débat que les choses seraient pas suffisamment éclairée que la réflexion stratégique qui aurait présidé ou précéder la LPM aurait été bâclé donc non. s'il le faut je serai là jusqu'au bout parce que précisément. Aussi. Non non mais je le dis parce que je je je mets en cohérence aussi l'ensemble de ce que j'ai pu entendre depuis depuis six mois sur la, la, la manière dont a été imaginé cette loi de programmation militaire. Monsieur le président Laurent sur le secret défense. Les choses sont assez simples. Il y a des choses qui sont classifiés les choses qu'ils ne sont pas posez-moi toutes les questions et c'est à moi de faire le tri entre ce que j'ai le droit de dire, de ce que la loi que le Parlement a voté m'autorise à dire pour être précis. C'est pas c'est pas ma discrétion ce qui est classifié ou pas c'est c'est un moment donné tout ça une base légale, ce que j'ai le droit de dire est-ce que je n'ai pas le droit de dire et d'ailleurs objectivement on peut quand même dire beaucoup de choses, si on est honnête et si on va même au-delà je le prends cet engagement devant le président. Une séance de commission qui ne serait pas retransmise ne me permettrais pas de dévoiler des secrets défense mais me permettrait d'être encore plus à l'aise pour parler d'un certain nombre de cas pratiques ou de situation. Sur lequel je n'ai pas forcément envie de susciter une réaction de telle ou telle ambassade où vous devez l'hôtel le partenaire pour dire les choses très très clairement. Mais oui le format de la dissuasion. A évolué dans le temps. Déjà avec l'apparition puis la disparition de ce qu'on a appelé abusivement le nucléaire tactique, c'était plutôt dans sa composante armée de terre, la fermeture d'Albion dans les années 90. Et pour cause, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dissolution du Pacte de Varsovie, un certain nombre de de décisions ont été prises, la profession de l'armée de terre enfin de désarmer. En général, pardonnez-moi, qui a beaucoup touché l'armée de terre mais aussi évidemment le fait de toucher la composante et là dans la loi de programmation militaire telle que nous la proposons, vous n'avez pas de modification en tant que telle, du format de la dissuasion composante aérienne les fasse composante océanique, La Poste avec des modifications de matériel mais toujours sur les mêmes cibles quatre SNLE et une demi- composantes comme on le dit, là aussi c'est pas très élégant pour la Fanny qui peut être embarqué ou non sur le porte-avions Il y a pas de modification de la doctrine en tant que telle, elle a été réaffirmée par le président de la République à l'école de guerre lors d'un discours hein c'est un peu la tradition qui fait que chaque quinquennat au septennat, le chef de l'État, quel qu'il soit précisé les choses. Si ce n'est que le président au regard des circonstances a été amené en parler plus. Que à l'accoutumée aussi pour répondre à ce qui a été dit à l'instant sur la nécessaire compréhension et notamment des phrases comme les intérêts vitaux. Ont une dimension européenne. Ça fait 15 ans que c'est le cas et cette affiche est très clairement dans la doctrine française mais qui est un des éléments qu'on a répété à de nombreuses reprises ces derniers temps, ce qui est aussi un des moyens de répondre aux sénateurs téma donc il y a beaucoup de sujets qui sont complètement en sources ouvertes qui sont enseignées à l'école de guerre aux Chem pour les parlementaires qui ont été auditeur l'IHU ADN donc il y a pas de raison qu'on fasse moins ici mais c'est bien pour ça mais vous avez raison monsieur le sénateur, Hervé. C'est pour ça que moi je veux redire que je suis disponible pour le faire. D'ores et déjà ici et maintenant, et de ne pas le renvoyer à plus tard, sans quoi je sais aussi désormais d'expérience qu'on regrettera de pas l'avoir fait, maintenant ensuite. Merci. Alors je mets aux voix l'amendement 234 qui a reçu donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contrat qui s'abstient. Il n'est donc pas adopté l'article 7 je le mets aux voix qui est pour, contre qui s'abstient. Il est donc adopté hier, mes chers collègues. Je vais suspendre la séance. Hein et elle sera reprise à 21h 30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.